La séance est reprise. Alors la parole est à monsieur André Gattolin pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci beaucoup madame la présidente. Oui, je voudrais dire que lors du scrutin numéro public numéro 120. Mon collègue Didier Rambaud souhaitaient voter pour et mon collègue Alain Richard souhaitaient voter contre les votes avaient été inversés, je vous remercie. Acte est donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. Mes chers collègues. Par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 16 février matin et éventuellement l'après-midi après l'examen de la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture sous réserve de leur dépôt acte et donner de cette demande. Le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixée au mercredi 15 février à 15h, y a-t-il des observations. Il en est ainsi décidé. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple. Durant la première guerre mondiale. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un espace réservé au groupe écologiste solidarité et territoires qui ne se poursuivra pas au-delà de 16h 10. dans la discussion générale. Nous sommes parvenus à l'intervention de Monsieur Guillaume Gontard, un rapporteur de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour 10 minutes. madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 10 mars 1915. Les poilus de la 21ème compagnie du 336ème régiment d'infanterie. Refuse de courir à une mort certaine. Pour reprendre une position au nord du village de soins. 24 d'entre eux sont tirés au sort arbitrairement et comparaissent devant le conseil de guerre. Quatre caporaux sont condamnés à mort. Ils sont fusillés le 17 mars par leurs camarades. Quelques heures avant que ne parvienne le résultat du recours en grâce commuant leur peine en travaux forcés. 14 juin 1915 après s'être fait soigner d'une blessure. Joseph Gabrielli. Ne parlons pas, ne parlant que le Corse ne parvient pas à rejoindre sa compagnie. Il est condamné à mort pour abandon de poste et fusillé le jour même. 21 mai 1916. 4 soldats sont condamnés à mort à Russie quelques jours plus tôt, ils avaient retardé d'une heure le départ de leur compagnie. Initialement, condamnée à 8 jours de prison. Leur peine a été modifiée en condamnations à mort. Pour faire un exemple. Des récits semblable. Glaçant confondant d'injustice et confinant parfois à l'absurde. Les historiens de la Grande Guerre. On ne. Des centaines. Pour avoir refusé de courir devant la mort ou pour l'avoir laissé penser des centaines de poilus ont été fusillés pour l'exemple. Les conseils de guerre spéciaux instaurés par le décret du 6 septembre 1914 ont donné droit de vie ou de mort haut gradé sur les soldats. Même sans conseil de guerre, les officiers pouvait exécuté sommairement soldat dont il jugeait la conduite dangereuse. En France, plus encore que dans les autres nations belligérantes la justice militaire était implacable et chercher à faire des exemples pour maintenir les soldats dans la peur. Ils nous ont laissé le choix qu'entre la mort certaine et la mort probable. Les condamnés n'avait pas les moyens de se défendre était parfois tirés au sort dans un groupe d'accuser et abattus par leurs pairs devant leurs pairs. Celui qui refusaient de tirer sur son camarade était condamné à prendre sa place. Dès le 20 août 1914, de pouvoir politique par la plume du Ministre de la guerre, Adolf Messi mis en 2, cette responsabilité en reconnaissant que cette justice d'exception n'a pas tant vocation à punir des coupables qu'à faire des exemples. Les historiens, notamment ceux du groupe de travail dirigé par l'illustre Antoine pro dont le rapport fait autorité. On dénombrait environ 740 soldats, fusillés au cours de la guerre. À la demande de l'ancien secrétaire d'État Kader Arif, le service historique de la Défense a établi une liste de 639 personnes fusillées pour désobéissance militaire auxquels s'ajoutent 141 fusillés pour des faits de droit commun et 126 pour espionnage. La présente, proposition de loi vise à réhabiliter ses 639 soldats. Je précise au passage pour lever certaines inquiétudes que si ce nom ne figure pas dans le corps de l'article il est explicitement mentionné dans l'exposé des motifs et que l'intention du législateur et sans ambiguïté. Ces sodas sont-ils morts pour la France comme le considère les dizaines de maires qui ont porté leurs noms sur les monuments aux morts de leurs communes, et comme nous sommes nombreux à le croire. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été qu'ils ont Chers collègues. Ce n'est pas réécrire l'histoire que d'admettre cette froide vérité. C'est au contraire accepter notre histoire dans toute sa complexité reconnaître qu'assailli pris à la gorge. La République a commis une lourde faute en confiant la mission régalienne primordial de rendre justice à des conseils de guerre spéciaux. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement de valeur sur des faits vieux de plus d'un siècle avec les yeux du présent. Comment le pourrions-nous il le séchait pas ici de blâmer les gouvernements républicains qui ont officié durant le conflit, chacun peut entrevoir l'extrême complexité que de gouverner un pays assailli, a fortiori quand l'armée ennemie est aux portes de Paris. Il ne s'agit pas non plus de blâmer une armée qui avait ah mission vitale de protéger la nation et dont le fonctionnement, notamment le droit militaire était très largement héritée de la période impériale. Il s'agit simplement de reconnaître que dans des circonstances d'une extrême gravité. Des centaines d'hommes ont été victimes d'un déni de justice tellement grave qu'il entache la mémoire collective de la Grande Guerre depuis plus d'un siècle. Car le problème qui s'est abattue injustement sur la plupart de ses soldats s'est abattue sur leur famille parfois sur toutes leurs communes. Et a traversé des générations, ce sont ces familles qui un siècle après demande encore la réhabilitation de leurs aïeuls. Qu'est-ce qui différencie un soldat tiré au sort pour être fusillés de son camarade du même bataillon qui a également refusé de monter au front, une nouvelle fois mais qui a échappé aux hasards du destin. Le nom du second figurent sur un monument aux morts sous la mention Mort pour la France et sa mémoire est honorée depuis un siècle la réhabilitation du premier est envisagée, alors que la guerre fait encore rage. Mais le Parlement tiraillée entre la compta cette constatation désolée des exactions manifeste et la nécessité de préserver l'union sacrée n'engage pas ce combat. Il supprime néammoins en 1916, les conseils de guerre spéciaux. Cette mesure va drastiquement faire diminuer les exécutions. Ainsi en 1900, cette année, des grandes mutineries, seule une trentaine de soldats et condamné à mort. De fait, l'essentiel des fusillés l'ont été en 1914 et 1915. Les travaux d'Éric Viot, ont montré que nombre d'entre eux ont été victimes de quelques officiers zélé qui dans chaque division par laquelle il passe accroissent le nombre de fusiller. Certains ont heureusement été désavoué et relevé par leur général comme les officiers qui ont condamné à mort les 6 fusillés de Russie. Au lendemain de la guerre, la réhabilitation des fusillés est assez consensuelle. Les soldats revenus du front AIC avant tout les embusqués et les profiteurs mais pas ceux qui avaient combattu à leurs côtés. Dans l'entre-deux guerres, le Parlement tente autant que possible de réparer l'erreur de 19.114, avec l'adoption très large, voire unanime de plusieurs textes lois d'amnistie du 29 avril 1921, plusieurs lois pour faciliter les procédures de réhabilitation loi ouvrant la possibilité de procédure devant la Cour de cassation. Réforme du code de justice militaire en 1928. Création même d'une cour spéciale de justice militaire qui siège entre 1932 et 1935 pour examiner certains dossiers. Au total, environ 10 pour % des soldats, fusillés sont réhabilités. C'est peu. Les réhabilitations furent aléatoire, il fallait qu'il y ait des témoins survivants que les familles s'impliquent elles et des relations bien placées et que la demande soit prise en j'en charge par une à une association comme par exemple la Ligue des droits de l'homme pour nombre de familles modestes d'ouvriers de paysans, ces voies de recours était inaccessible. Poursuivent les réhabilitations au cas par cas serait naturellement le chemin idéal mais ce chemin n'existe pas. Le général bac historien du ministère des Armées la montrer. Il manque de 20 à 25% des dossiers et beaucoup d'autres sont vides ou si incomplet, qu'il est impossible d'en rien tiré la réhabilitation ne peut être que collective. Il serait de toute façon inconcevable de rejuger aujourd'hui des faits vieux de plus d'un siècle, le temps de la justice est passée, celui des historiens qui ont désormais exploiter l'essentiel des archives aussi vient désormais le temps du politique qui doit se prononcer non pas sur l'histoire mais sur la mémoire de la nation. Un 1er pas important a été accompli au sommet de l'État Lionel Jospin le 1er en 98 à Khan a souhaité que les fusillés pour l'exemple, réintègrent pleinement notre mémoire collective nationale. Nicolas Sarkozy ensuite dans un discours fort à Douaumont en 2008 a tenu à les rétablir dans leur honneur, puis sur l'Arc de Triomphe en 2009 a évoqué ces fusillés qui attendent encore qu'on leur rende justice en 2014 pour le centenaire, sous la présidence de François Hollande un espace a été aménagé en leur mémoire au sein du Musée des armées. Localement, près de 2000 communes. 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux dont beaucoup de territoires marqués par les les stigmates de la Grande Guerre ont adopté des voeux pour réhabiliter les fusillés des monuments ont été érigés en leur mémoire comme le magnifique monument de Chauny dans l'Aisne où les associations locales d'anciens combattants leur rendent également hommage jusqu'à présent je n'ai, je crois qu'exposé des faits que personne ne conteste. Reste à conclure ce chapitre notre assemblée s'est prononcée une première fois sur une proposition de loi similaire de nos collègues communistes emmenés par Guy Fischer. Elle est amenée aujourd'hui à se prononcer sur cette proposition de loi de notre collègue Bastien Lachaud que je salue, adopté à l'Assemblée nationale. La commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées après un riche et vibrant débat s'est prononcé à une très courte majorité contre ce texte, cette majorité a notamment estimé que la réhabilitation. De personnes condamnées par décision de justice posait un problème juridique et que seuls des réhabilitations individuelles était légitime. Certains ont également craint que le Parlement ne s'engage dans une réécriture dommageable de l'histoire qui ne relevait pas de ses prérogatives, mais uniquement de celles des historiens à titre personnel je considère au contraire que le Parlement doit conclure ce qu'il a commencé en 1916. Alors que la guerre de tranchées que l'on croyait appartenir aux vestiges du passé, ressurgit à quelques milliers de kilomètres de nous en Ukraine. Le Sénat tout entier peut choisir aujourd'hui de lever l'opprobre et d'affirmer que nul n'aurait dû et ne devrait jamais être condamnés à mort sommairement parce qu'il a comme tout soldat. Eu un moment de doute ou d'effroi face à l'atrocité indicible d'une bataille d'infanterie. Je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Tout d'abord il m'apparaît toujours délicat de regarder l'histoire avec les yeux les connaissances et les mentalités d'aujourd'hui. Comment nos propres actions de responsables politiques seront-elles jugé dans un siècle ou 2. Nul ne le sait, et nous agissons tous avec les critères et usage de notre époque. Qui paraîtront peut être inapproprié. Aux générations futures. Ensuite, je rappelle le contexte de la période 14 18, la guerre et mondiale totale. Chaque parti, joue sa survie. Des millions d'hommes dont la plupart étaient de simples civils se battre sur plusieurs fronts. L'ennemi de la France n'est pas n'importe qui. Il s'agit de l'Allemagne et de ses alliés, c'est-à-dire une puissance économique industrielle et militaire considérable. Le traumatisme de 1870, habite les esprits. Une nouvelle défaite de la France aurait signifié la fin de la France. Les soldats mobilisés quant au cours des combats étaient confrontés à un niveau de violence inouïe et inédit dans une guerre véritablement industriels qui utilisent pour la première fois en masse des armes très meurtrières terrorisante. Les conditions de vie étaient particulièrement rude comme nous le laisse entrevoir actuellement la guerre de tranchées en Ukraine. Nous le savons aujourd'hui beaucoup de vies ont été sacrifiés en 14 18 dans des offensives inutiles ou en raison d'erreurs de commandement. La période 1914 1915 et celle des combats les plus meurtriers et probablement les moins bien préparés qui donne lieu à de nombreux faits de désobéissance militaire entraînant de multiples condamnations, comme le rappelait le rapport Probst en À côté des blessures physiques des soldats. Étaient souvent ils étaient souvent pardon atteint de troubles psychiques qu'on appelle désormais syndrome post-traumatique qui altère le jugement et annihile la volonté. Pour autant, la France ne pouvait se payer le luxe de perdre du terrain ni de voir la troupe gagnées par des actes de de désobéissance et une démoralisation générale face à un ennemi coriace. Des mesures radicales c'est vrai ont été prises et conformes à l'esprit de l'époque et à la situation de guerre. Tous les belligérants ont d'ailleurs prononcé des condamnations à mort dans leurs rangs. Signe des temps, des procès hâtifs ont été tenus et dans lesquelles les droits de la défense était limité. Il faut souligner et enseigner cette réalité qui fait partie de notre histoire collective. Il me paraît néanmoins inapproprié de mettre sur un même plan ceux qui épuisés et eux aussi probablement la peur au ventre ont néanmoins accompli jusqu'au bout leurs devoirs face à l'ennemi. Il est 100 souvent la vie et ceux qui pour des raisons que l'on peut peut-être être entendre n'ont pas voulu se battre, je me garderais bien de juger ces derniers. Les tribunaux l'ont déjà fait et des réhabilitations ont eu lieu dès les années 20. Mais comme le rappelait là aussi le rapport Probst imaginer qu'on puisse aujourd'hui établir une vérité sur la plupart des cas de fusiller est une pure illusion. Et si comme notre commission je n'approuve pas cette PPL elle offre néanmoins l'occasion de rappeler la mémoire de tous les soldats de cette guerre épouvantable qui a brisé les corps, les esprits durablement affaibli l'Europe, mais néanmoins je n'approuverai pas cette PPL je vous remercie. Merci la parole est à Madame, Colette Mélot pour le groupe les indépendants et pour quatre minutes. Madame le président, madame la ministre. Mes chers collègues. La jeunesse du XXIe siècle a connu les confinements celle du début du XXe siècle connaissait les tranchées, les gaz les charges à la baïonnette, le feu roulant et les shrapnel. Siècles. Le monde a évidemment changé. À tel point que nous avons du mal à nous représenter l'horreur des combats. Nous avons reçu un héritage de précieux témoignages. Celui de nos anciens. Tout d'abord à travers des lettres et quelques rares discussions. Des écrivains nous ont aussi laissé. Une trace mémorable de ce qu'ils ont vécu comme Maurice Genevoix Roland Dorgelès ou encore ainsi Unger tous ces récits sont difficiles choquant. Et marquant mais ils ne sont que des récits. Ils ne peuvent transmettre la mémoire de la peau, celle de ceux qui ont vécu cette apocalypse. Celle-ci s'est éteinte en 2008 avec la disparition de Lazare Ponticelli. Le dernier poilu, il nous appartient désormais de maintenir allumé la flamme du souvenir. Les monuments au bord de nos communes retiennent les noms de ceux qui se sont battus pour défendre la patrie des Ardennes aux Dardanelles. Il s'agit de leurs fondamentaux de lieux fondamentaux pour notre République et pour notre nation. La première guerre mondiale a fait plus de 4 millions de blessés parmi les militaires de notre pays. Elle a tué près d'un million et demi de soldats français. Aujourd'hui, même avec ces chiffres en tête, on peine à se représenter l'ampleur du massacre. Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. Certains d'entre eux cependant, sont morts sous les balles françaises. Condamné à mort par une justice de guerre. Une justice qui n'offrait pas de procès équitable à l'accusé. Elle a exécuté des déserteurs comme des soldats tirer au sort mais aussi des fous. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à réhabiliter l'ensemble des militaires condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilations volontaires par les conseils de guerre spéciaux, c'est-à-dire 639 soldats. Ainsi qu'il a été rappelé dès 1916. Le parlement français a décidé de mettre fin à ces tribunaux spéciaux. Il reconnaissait ainsi que ces procédures n'avait pas grand chose à voir avec la justice. Dans les années qui ont suivi la guerre plusieurs vagues de réhabilitation ont eu lieu. Il demeure cependant 639 nous. L'examen individuel n'est pas envisageable pour bon nombre d'entre eux. Dans la mesure où leurs dossiers sont parfois manquant ou bien inexploitables. Nous sommes tous soucieux de la mémoire de ces hommes tous soucieux également de la cohésion de la nation. La réhabilitation générale est ardemment souhaitée par certains tandis que d'autres craignent qu'elle ne soit porteuse de divisions. Le rapporteur évoquent des moments de faiblesse pour convaincre que ces condamnations étaient injustes. À la guerre, les moments de faiblesse n'ont-ils pas toujours des conséquences tragiques pour les camarades comme pour la patrie. Que serait-il advenu si tous nos soldats avaient cédé à des moments de faiblesse. Ces exécutions était injuste parce que nul ne devrait être condamné à la peine de mort. Qui peut aujourd'hui juger des actions et des décisions qui ont eu lieu il y a plus d'un siècle. Nous sommes face à notre conscience, chacun des membres de notre groupe votera conformément à la sienne. Merci. La parole est à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires et pour quatre minutes.

Madame la présidente. Madame la Ministre, c'est le rapporteur, Charles Guillaume, chers collègues. On retrouva aujourd'hui pour étudier une loi de justice. Une loi qui permet de revenir sur le déni d'une justice militaire arbitraire bafoue le droit de la défense. Une loi qui permet de rendre leur honneur à certains combattants tombés sous les balles d'un tribunal militaire exécutés après avoir été parfois tirés au sort une loi qui plus que d'autres dépasse tout clivage partisan. De nombreuses associations. Ont fait du devoir de réhabilitation juste combat monsieur Gosselin député des républicains de la moche ah lors de la discussion à l'Assemblée nationale, évoquer la statutaire Théophile Maupas. Des caporaux de soins dans le cas avait été défendue avec acharnement par sa veuve blanche pour pas en lien étroit avec la LDH et que seule une cour spéciale de révision en 1932 réhabilite monsieur Nicolas Sarkozy, a reconnu que ses soldats je cite ne s'étaient pas déshonorés car ils étaient allés jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. N'oublions pas que cette grande guerre a décidé d'au village les monuments aux morts dans l'ensemble de nos territoires, nous rappelle le coup Hubei de la guerre. La souffrance des familles. De nombreux conseils municipaux des conseils départementaux des conseils régionaux. Conscient de cette blessure en eux aussi demander justice pour ces fusillés pour l'exemple pour parfois n'avoir pas entendu hein, d'ordre car il ne parlait pas le français ou pour désertion alors qu'ils étaient en fait blessés. C'est cette reconnaissance tardive mais nécessaire que ce texte propose la réparation leur est dû. Je remercie d'ailleurs le rapporteur pour la qualité de ses travaux et pour avoir permis de mettre à jour combien cette réhabilitation et d'SSR et sous cette forme. L'examen au cas par cas, alors que près de 20% des archives ont désormais disparu ajouterait de la justice à la justice. Comment instruire de tels dossiers. Son témoignage. La liste des fusillés pour l'exemple. Ces personnes en fait dès Yacoubi aucun Crime ni de droit commun, ni d'espionnage fait consensus au niveau des historiens comme au niveau de l'administration du ministère des Armées. Ces personnes, ces soldats au début de Kofi si terrible et meurtriers ont été accusé le plus souvent de mutilations volontaires d'abandons de poste ou de refus d'obéissance en présence de l'ennemi. L'auteur de la présente PPL que nous saluons ici rappeler que dès 1925, médecin légiste démontra qu'il n'était pas possible de déterminer si une blessure était tous dans le résultat d'une mutilation volontaire ce qui aurait dû entraîner la réhabilitation de tous les condamnés pour ce motif mairie Bettel deux fut pas le cas. J'entends les réticences de certains qui voient dans cette loi une réécriture de l'histoire, il n'en est rien, c'est une loi de réhabilitation. Il ne s'agit pas de regarder le passé avec les yeux du présent dès 1916 l'armée suite à l'intervention de députés s'est posé la question de ce simulacre de justice militaire et à supprimer ses conseils de guerre spéciaux rendant possible de rétablir les circonstances atténuantes et de permettre les recours en révision. Cette réhabilitation passe aussi par la juste reconnaissance de ces 639 martyrs de l'armée. Il est de notre devoir de reconnaître et réparer les injustices réparées tant que faire se peut, car pas leurs biens de jeune homme de 18 20 ans parfois ayant payé de leur vie. La dérive de ses conseils de guerre spéciaux dans les règles étaient déjà dépassé. Une inscription aux monuments aux morts va dans le sens de la justice pour ses soldats et officiers notre rapporteur l'indiquer il revient après les historiens après les juges à la représentation nationale de se prononcer dans pas sur l'histoire mais sur la mémoire de la nation. Mes chers collègues, ils sont bien rares. Les textes qui peuvent et doivent nous unir tellement ils sont juste et essentielle à d'autres pays merci. C'est pourquoi dans le groupe geste vous propose ce texte, qui rend enfin justice à ses soldats et créer les conditions de notre devoir mémoire envers leurs vies inutilement sacrifié. Merci cher collègue. La parole est à monsieur André Gattolin pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et pour quatre minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues comme tout texte législatif à dimension mémorielle. La proposition que que nous discutons aujourd'hui est particulièrement sensible sur le fond la question ici posée est de savoir quel statut doit en plus d'un siècle après les faits, accordé à 639 militaires de l'armée française qui ont été condamné pour désobéissance militaire par un conseil de guerre entre 1914 et 1918 et qui n'ont pas fait l'objet d'un procès en réhabilitation durant les années qui ont suivi la première guerre mondiale. Ces 639 militaires exécutés, disons-le clairement, et avec des mots crus ne sont par leurs actes ni des héros ni des salauds. Ce ne sont pas des héros. Car si d'une certaine manière ils sont morts par la France, il ne saurait être cependant considéré comme des morts pour la France une acceptation clairement codifié dans notre droit. Ce ne sont pas non plus des salauds, car aucun d'entre eux dans cette longue liste n'a été condamné pour des faits d'espionnage ou de ralliement à l'ennemi. Il s'agissait tout simplement de soldats engagés dans un combat combat d'une férocité inouïe et qui, dans des circonstances extrêmes ont refusé d'obéir aux ordres de rejoindre leur bataillon ou encore se sont gravement mutilé en vue d'être démobilisés ou garder à l'arrière du front. En l'état et en dépit des déclarations et des gestes successivement engagé par le 1er ministre Lionel Jospin, puis par les présidents Sarkozy et Hollande de morts aujourd'hui encore des parias de la nation et cela, à mon sens comme à celui de nombre d'entre nous n'est pas admissible. Le problème qui se pose c'est que le texte qui nous est proposé ici après son peu d'options à l'Assemblée nationale est entâchée de nombreuses imperfections et même je le crains de vices de constitutionnalité alors qu'il vise à restaurer leur dignité aux militaires qui ont été exécutés, il déborde largement de ce cadre en instruisant une sorte de procès des autorités politiques, militaires et judiciaires de l'époque. Historien de formation j'appréhende toujours avec beaucoup de précaution et parfois même de méfiance, les lois mémorielles qu'elle émane du gouvernement ou du parlement. Je rappelle que nous sommes tous ici des législateurs. Ce qui nous enjoint d'être soucieux de la conformité de nos lois avec la Constitution. À ce titre, il est dommage que ce texte n'ait pas été soumis à un avis préalable du Conseil d'État comme cela. RFI est possible depuis la réforme constitutionnelle de 2008 ont plus gros doutes concernent l'habilitation juridique du Parlement a procédé de son seul fait à une réhabilitation je cite général collective civique et moral des militaires fusillés. L'acte de réhabilitation dans notre droit, relève d'une procédure judiciaire qui ne peut être procédé que par un juge. Il passe par la réouverture des dossiers individuels de chacun des cas concernés. de l'importance du sujet. J'ai donc déposé un amendement visant à réécrire l'article 1. Cette proposition et non pas à réécrire l'histoire en substituant notamment la notion de réinscription des militaires fusillés dans la mémoire nationale à celle à mon sens très discutable de réhabilitation collective une approche plus juste et plus conforme aux principes fondamentaux de notre droit. J'ai proposé aussi. Dotés de ce texte certaines scories qui à mon sens les maillets, ah si je suis si je suis favorable à l'érection d'un monument national en mémoire d'assez fusillés je trouve inapproprié de préciser, ici, dans la lignée de que ce monument leur rendent hommage. Mon amendement, je dois dire a été rejeté à une très forte majorité, par la commission. Je regrette qu'aucun de mes collègues qui eux aussi ont constaté des insuffisances dans ce texte n'est proposé d'amendement, ce qu'ils recherchent. Sans doute aurait permis de clarifier leur avis à ce sujet, je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, madame la Ministre, Monsieur le Président notre commission monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, fusillés pour l'exemple. Cette seule est terrible expression peut faire froid dans le dos, particulièrement en temps de paix. Mais l'histoire nous enseigne et malheureusement l'actualité du présent également que toute guerre livre ses propres horreur et laisse très peu de place au sentiment d'humanité. Du meilleur comme du pire. Ainsi l'humain serait-il fait. Lorsque les militaires sont au combat pour défendre une nation un territoire parfois liés à une philosophie de l'existence. Nous savons que la discipline collective fait partie intégrante de leur engagement. Mais mes chers collègues. Ce n'est pas vraiment de cela dont il s'agit aujourd'hui lorsque nous évoquons les fusillés pour l'exemple. Ils avaient 18 ou 20 ans. Combattaient dans des conditions atroces. Le seul fait de gagner quelques mètres entre de trancher et de ne pas en perdre pouvait entraîner la mort de plusieurs dizaines de soldats, l'espace d'un seul instant. Nous pourrions penser de ce fait que les fusillés pour l'exemple était ceux qui refusaient ce combat peu rationnel, où seule la discipline était l'Alpha et l'oméga de l'engagement. Mais non ce n'est même pas très majoritairement de ce dont il s'agit c'est le confusion ne peut exister. Les condamnés Le Fur principalement en retrait de la ligne de front et particulièrement en 1914 et 1915, ils n'ont donc rien à voir avec les mutins de 1917 lorsqu'un soldat a été déclaré couple able d'indiscipline la sentence tombait aucune possibilité de se défendre. Pas de contradictoire devant ses cours martiales particulièrement expéditive et arbitraire certains fusillés pour l'exemple, furent même tiré soeur que dire. De ce soldats refusant de porter le pantalon souillé de sang de son camarade. Jugé le jour même de ce refus, il est condamné à mort il est fusillé le lendemain matin. Face à ces effrayant constat dès 1916, les députés et ce, à l'unanimité votent la fin de cette justice d'exception et restaure le même jour le droit de grâce, utilisée par le président Poincaré. De sorte que dès 1916 95% des condamnés à mort furent graciés. Une forme de réhabilitation était déjà en marche. Souvenons-nous, mes chers collègues, de cette période noire de notre histoire et des familles de fusillés pour l'exemple qu'subissait l'opprobre et la honte dans nos villes, c'est le village. Souvenons-nous que la facture de la balle qui les avait exécuté des poteaux qui les avaient soutenus étaient envoyés aux familles. Souvenons-nous de cette inhumanité là. Oui, comme le souligne Erik Orsena la mémoire c'est la santé du monde ce devoir de mémoire s'impose à nous tous. Ce devoir de compassion et de réparation doit s'inscrire au tableau d'honneur de notre haute assemblée observons et reconnaissons volontiers et admirons combien les généraux et officiers de nos 3 armées que nous rencontrons fréquemment dans le cadre de nos fonctions de parlementaires sont particulièrement soucieux de nos jours de préserver la vie et la santé des soldats qui commandent et dirigent et hommage doit leur être rendu pour cela c'était moins le cas, nous le savons, des 2 premières années de cette guerre. 14 18. Mes chers collègues. De nombreux historiens se sont penchés sur ce délicat sujet des fusillés pour l'exemple afin de déterminer qui était coupable de trahison qui était coupable de mutilations volontaires pour échapper aux combats. Fier du cas par cas, été juridiquement logique idéal. Ils ont cependant conclu que c'était impossible du fait des disparitions d'archives eux-mêmes ont indiqué qu'il était préférable de procéder à une réhabilitation générale excepté pour les traîtres et les crimes de droit commun. La proposition de loi de ce jour, indique précisément condamné pour désobéissance militaire ou mutilations volontaires du service historique du ministère des Armées ont estimé formellement qu'il y a 639 fusillés pour l'exemple, qui ne sont ni des traîtres Didier droit commun et c'est essentiellement à ces 639 que s'adresse la réhabilitation proposé aujourd'hui. De nombreuses avancées ont permis depuis 1914 1915, de reconnaître les choses les fautes commises et ceci dès 1916 comme je l'évoquais précédemment depuis sous différents gouvernements ça été rappelé de droite et de gauche avec Lionel Jospin puis Nicolas Sarkozy et François Hollande de véritable reconnaissance ce ton se sont mises en oeuvre. Jean Marc tôt défini notre collègue, alors secrétaire d'État rappeler en 2016 que désormais les fusillés pour l'exemple sont intégrés aux espaces muséographiques du musée de l'armée consacré à la première guerre mondiale, à l'Hôtel des invalides. Ainsi au coeur de l'institution militaire leur mémoire tient la place qui leur est dû. Dans le prolongement de ces différentes évolutions. Nous devons aujourd'hui compte tenu des précisions apportées franchir une nouvelle et dernière étape, celle d'une réhabilitation, à la fois précise et général cette démarche sera l'honneur de notre République. Elle serait le point final tant attendu est le prolongement logique des prises en considération successives des erreurs et fautes juridique commise. Mes chers collègues, à la fin de mon propos, je songe à ces très jeunes gens fusillés pour l'exemple et à leurs familles humiliées, rendant leur honneur et fierté d'être dans une communauté nationale dont la grandeur et de reconnaître ses erreurs en ce moment je pense aussi à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc j'imagine aisément qu'elle approuverait notre démarche. Après presque plus d'un siècle même faire cela ce serait pour notre Sénat signe de sagesse et de hauteur de vue, ce serait aussi mettre en évidence après tout ce temps que notre nation la France n'est pas seulement le pays de la déclaration des droits de l'homme mais qu'elle ambitionne véritablement d'être le pays des droits de l'homme. Merci. La parole est à madame Michelle Gréaume pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour quatre minutes, chers collègues. Madame la ministre, madame la présidente, mes chers collègues. Dans un monde en feu où les grandes puissances se sont affrontés pour le partage des marchés et des ressources pour la reconquête de colonies pour la restructuration de leur sphère d'influence. La guerre de 14 18 fut une accumulé une accumulation d'horreur pour les soldats, comme pour les civils. Durant ce conflit des soldats français et immigrés furent exécutés dans le cadre de conseil de guerre improvisé pour cause d'indiscipline militaire refus d'obéissance abandon de poste désertion à l'ennemi, tandis que d'autres furent abattus au détour d'une tranchée par un officier. À bout portant pour rébellion soit et je tiens à le rappeler avec émotion pour appartenance connue à des organisations ouvrières militant contre la guerre. La réhabilitation des fusillés pour l'exemple nous Charles coeur et j'en profite pour rendre hommage à notre ancien collègue Guy Fischer. Qui avait porté avec brio cette question dans l'hémicycle. Notre groupe avait déposé en 2013 une proposition de loi visant à répondre à la demande juridique et mémorielles au sujet de la réhabilitation. Celle-ci reposer sur une approche globale car nous considérions qu'il n'était pas possible de faire le tri. Plus de 100 ans après, entre les soldats, fusillés à tort, victime de condamnations arbitraires ou abusive et ceux dont l'exécution aurait été justifié. Le parti pris du texte ce qui nous est présentée aujourd'hui est différent. C'est un regret. Il nous semble toutefois essentiel de soutenir le principe qui anime. À savoir la réhabilitation d'hommes exécutés pourra. Lors de la Grande Guerre. Conscient également que ce sujet reste encore sensible. Nous avons fait le choix dans un esprit de conciliation positive de ne pas amender ce texte car cette réhabilitation ah siècles plus tard, et toujours sujette. À controverse. Déjà parce qu'elle touche à des destins individuels poignant à la Star du sous-, lieutenant Chapelon fusillé attachée sur son brancard ou encore celui du soldat Lucia berceau condamnés puis exécutés pour avoir refusé de portes de porter le pantalon taché de de son, de de son, de son frère d'armes. Je profite de ces exemples, pour saluer le travail et l'engagement des associations dans leur combat pour la réhabilitation des fusillés comme l'Association républicaine des anciens combattants. Le mouvement de la paix l'Union pacifiste de France ou encore la Libre pensée. Le sujet divise également les tenants d'une discipline garant de l'intégrité nationale justifiant une sévérité exemplaire, ainsi que l'absence d'une quelconque remise en question de celle-ci et se défendant une lecture humaniste qui considère que ses soldats n'étaient ni des lâches ni des traites, mais des hommes qui avaient fait leur devoir usé par la guerre et la violence physique et psychologique. Des combats. Des soldats qui étaient allés au bout de ce qu'un homme pouvait endurer. Qu'il ne comprenait pas au plus les objectifs et le sens de ces combats et de la mort certaine vers laquelle on les envoyer. Il ne méritait certainement pas la mort. La dignité dont ils sont encore aujourd'hui frappée doit être lavé. En tant que communiste et républicaine, je suis absolument convaincu que l'adoption de ce texte serait un acte de fraternité pour la mémoire de ces hommes qui furent jetés dans l'arène meurtrière des tranchées et qui fut cul par l'épuisement. Certains collègues nous ont dit vouloir des réhabilitations individuelles plutôt qu'une réhabilitation collective. Pourtant les historiens sont unanimes. Cela n'est pas possible. Âpre avec près de 20% des dossiers disparus, la possibilité d'enquêter, l'absence de témoins encore vivants. Accéder à une telle demande reviendrait à repousser toute réhabilitation. D'autres de nos collègues ça qui assure jusqu'à l'air déchirant écrivant de la réhabilitation collective au sein de notre pays. Merci. Le groupe hier tu sais assez votera pour ce texte. Merci. La parole est à monsieur Olivier Cigolotti pour l'Union centriste et pour six minutes. Madame le président, madame la ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. La question des fusillés pour l'exemple constitue un volet particulièrement douloureux de la première guerre mondiale et n'est pas sans soulever émotion et des bas historique. Preuve en sont les différents échanges que nous avons pu avoir lors de nos travaux ça notre commission et les témoignages parfois très fort. À ce titre je souhaite saluer le travail précis et documenté de notre rapporteur Guillaume Gontard, dont les travaux ont permis de débattre avec respect de ce sujet particulièrement sensible. La présente, proposition de loi pour objet de réhabiliter les 639 fusillés pour désobéissance militaire. En 1914 et 1915. Ces exécutions concernaient essentiellement des actes individuels tels que la désertion l'abandon de poste les mutilations volontaires ou encore le recul pendant l'assaut. Autant d'actes qui mettait en péril la mobilisation totale et l'engagement de nos régiment d'artilleurs pour défendre notre pays. Comme a pu le préciser. L'historien Antoine Prost dans le rapport qu'il a remis à Kader Arif en septembre 2013. Si beaucoup de fusiller l'ont été dans des conditions inacceptables. D'autres l'ont été pour des raisons sérieuses. La question de la reconnaissance de ses hommes fusillés pour l'exemple, il n'est pas nouvelle. Avant même la fin de la première guerre mondiale, des associations de droits de l'homme et d'anciens combattants ou encore d'élus, toutes tendances confondues se sont mobilisés à ce sujet. Les lois d'amnistie de 1919 et d'avril 1921 qui instaure un recours contre les condamnations prononcées par les conseils de guerre spéciaux au bénéfice des conjoints ascendants et descendants jusqu'au 4ème degré ont été voté à l'unanimité des députés. Outre ces 2 lois d'amnistie, d'autres dispositions ont été voter le plus souvent de manière, de manière transpartisane. La loi du 9 août 1924, permettant la réhabilitation de soldats exécutés sans jugement. Une nouvelle loi d'amnistie votée le 3 janvier 1925, instaurant une procédure exceptionnelle devant la Cour de cassation ou encore la loi du 9 mars 1932 créant une cour spéciale de justice militaire composée de magistrats et d'anciens combattants et compétente pour réviser l'ensemble des jugements rendus par les conseils de guerre. Les travaux menés durant cette période, ont permis la réhabilitation d'une quarantaine de cas, je pense par exemple aux fusillés de 20 degrés. D'autres gestes politiques bien plus récents ont permis d'encourager la reconnaissance de ses soldats. En 1998, Lionel Jospin a été le 1er à rendre hommage aux fusillés pour l'exemple. Dans un discours prononcé à Crown lors des commémorations de l'armistice de 1918. Nicolas Sarkozy a rendu un hommage similaire le 11 novembre 2008 lors de la commémoration de l'armistice de l'Armistice au mémorial de Douaumont. Les travaux menés lors des commémorations du centenaire de la Grande Guerre ont abouti à la création d'un espace consacré aux fusillés au musée de l'Armée aux invalides, ainsi que la numérisation et la mise en ligne des dossiers des conseils de guerre sur le site Mémoire des hommes. Nous saluons l'ensemble de ces démarches et de ces avancées. Le travail historique et judiciaire déjà accompli a permis durant plus d'un siècle de revenir en profondeur sur ces réalités de la Grande Guerre. Mais également, me semble-t-il d'apporter un regard indispensable sur certaines injustices qui ont pu être commises. Aujourd'hui il est question d'aller encore plus loin en proposant une réhabilitation collective et générale. Cependant si nous décidons de réhabiliter ces soldats cela en sous-entend que leurs condamnations ont été prononcées à tort dans la totalité des procédures. Nous ne pouvons pas aujourd'hui établir cette réalité historique. C'est pourquoi la réhabilitation collective et générale proposée par ce texte ne nous paraît pas être une solution satisfaisante. Une réhabilitation doit être le résultat d'une décision judiciaire est le fruit d'une procédure individuelle et non la résultante d'un texte de portée généralisée. Elle apparaît à la fois politiquement inadapté à la situation et à la limite des principes de constitutionnalité. Pour toutes ces raisons, le groupe Union centriste votera dans sa grande majorité contre cette proposition de loi, je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur André Guillaume pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. Madame la présidente. Madame la ministre. Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur et chers collègues. Examiner ce texte visant à réhabiliter les militaires fusée fusillés pour l'exemple, c'est nous replonger dans le sens d'une certaine émotion dans un des épisodes les plus tragiques de la première guerre mondiale. En effet en filigrane de ce texte nous apparaît une certaine histoire celle du quotidien brutale et atroce des soldats dans les tranchées dans la boue sous la mitraille ennemie, la faim et la peur au ventre. C'est l'histoire touchante de ceux de 14. Comme les années dénommé Maurice Genevoix d'insérer ici rapporté au front de vers de. Le poilu André Fribourg l'écrivain de à 1915 au journal l'Opinion. Voilà près de moi que je ne me suis ni déshabiller ni des chaussées. Je me suis lavé deux fois. Dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché matelas, j'ai passé toutes mes nuits par terre. La nation a toujours salué le courage et les sacrifices consentis par tous ces hommes réduits à se battre dans des conditions insoutenables au nom de la patrie de la liberté et à en mourir pour beaucoup d'entre eux. Cependant, dans le tableau de l'honneur de la France subsiste une ombre, celle des fusillés pour l'exemple. Ce sont ces militaires qui nous occupe aujourd'hui. Seulement, il faut le préciser qui nous, qui n'ont pas été exécutés pour des crimes ou des droits de droit commun ou pour espionnage naturellement dans ce type de débat la question du rôle du législateur face à l'histoire et bien souvent posé. Pour la majorité des membres de mon groupe, il s'agit de ce con de pas. Ne s'agit pas de se conduire un historien. Le travail a été fait et je dirais même bien fait, notamment par l'historien Antoine Prost et ça a été dit tout à l'heure qui a rendu en 2013 un rapport au gouvernement sur les conditions de réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Il s'agit donc avant tout d'endosser la responsabilité de la justice au regard du trouble tester est largement reconnu puisque dans les discours présidentiel depuis Lionel Jospin sur ce régime exceptionnel des fusillés pour la France. Sur ces 639 soldats visés par le projet de réhabilitation collective. On sait que l'injustice et l'arbitraire ont concerné une majorité d'entre eux. Notre émotion face au sort de ces soldats de ces jeunes soldats sans droit à la défense serait-elle anachronique. Je ne le crois pas dès 2016. En plein conflit le régime des fusillés pour l'exemple, a été mis en question par la suppression des cours martiales et l'ouverture du droit au recours. Cela démontre le malaise que la méthode avait suscité dès l'époque et cela explique aussi la concentration des exécutions sur les années 1914 et 1915 comme cela été souligné notre collègue rapporteur a rappelé que certains officiers avaient également été relevés par leurs supérieurs, suite à des exécutions. Certes, on pourrait opposer qu'en temps de guerre. La faiblesse n'a pas sa place et que la discipline doit être implacable. Mais il est ici question de situations compliquées d'interprétations erronées. Quant à l'attitude de certains soldats pris au piège de l'enfer des tranchées et bien entendu à l'absence de droit élémentaire à la défense. Je pense aussi à ceux qui ont tenu le fusil à ces jeunes gens qui ont dû tué souvent l'ampleur, la boule au ventre leurs camarades. Et leurs frères de combat quel traumatisme irréparable. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, l'histoire, c'est l'étude et l'écriture des faits. La réhabilitation, c'est rendre estime public. Il s'agit donc de faire rentrer dans la mémoire collective si tu veux que ce qui aurait été exclues sans ménagement ici se rencontrent la justice et la discipline militaire. Tout notre discernement discernement doit être mobilisés. En tant qu'élu de la République. Nous devons contribuer à construire une société plus apaisée. Ne sommes-nous pas dépositaire d'une Frattini faire éternité bienveillante soucieux d'honorer cette valeur la majorité de mes collègues du RDSE approuveront la proposition de loi, je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains et pour trois minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Parmi les événements historiques qui jalonnent le passé de notre nation, pas un a plus profondément façonné le territoire et la société de mon département de laine que la Grande Guerre, notre département. Madame la présidente. Dans la commune de Fontenoy, berceau de ma famille paternelle, il y a une histoire qui se transmettait de génération en génération et qui m'avait glacé le sang lorsque j'étais enfant, celle du soldat Lucien berceau un jet de 33 ans, évoquée par nos collègues et Vaugrenard et qui avait été mobilisés au 60ème régiment d'infanterie puis envoyé sur le front de laine dès l'hiver 1914. En février 1915, le jeune militaire. Toujours le même pantalon de toile et blanc qui lui avait été remis à la mobilisation grelottant de froid dans les tranchées, il demanda l'autorisation de recevoir un nouveau pantalon de laine identique à celui de ses camarades le sergent Fourrier exécute à la demande en lui remettant un pantalon déchirés et maculés de sang. Récupérée sur le cadavre d'un soldat français français récemment tué. Berceau refusa de le porter. Il fut condamné d'abord à huit jours de cachot puis trouvant que la peine était trop clément que le lieutenant-colonel le fit comparaître devant le tribunal de guerre puis condamné à mort pour refus d'obéissance, il fut fusillé pour l'exemple. Le 13 février 1915. Si le soldat berceau fut réhabilité par la Cour de cassation en juillet 1922, aucun texte de loi ni aucun artifice ne sera jamais panser les plaies de ces quatre années meurtrières ni amender les décisions prises dans le contexte d'une six exceptionnelle violence que celui de la guerre, la politique c'est déjà fendu par le passé d'initiative tendant à la reconnaissance de l'injustice de leur sort. En déplacement à Crozon dans l'aine en novembre 1998 le 1er ministre Lionel Jospin à plat la réintégration des fusillés pour l'exemple dans notre mémoire collective. Tout comme le fit François Hollande en 2017 à Cerny en Lanois toujours dans l'aine. Nous comprenons la volonté des sénatrices et sénateurs porteurs de cette proposition qui résulte d'une intention hautement honorable je tiens par ailleurs à saluer le travail de notre rapporteure le président Gontard sur ce sujet particulièrement douloureux de notre histoire. Mais il n'appartient pas selon moi au législateur de réécrire l'histoire à la lumière de la lecture qui souhaiteraient en faire il lui revient néanmoins de consacrer l'histoire en tant que phénomène disant quelque chose de son époque et de sa société bien évidemment ces condamnations paraissent aujourd'hui être des actes juridiques entaché d'une cruauté sans nom. Mais quelle est la valeur de l'histoire, si nous ne consentons pas à la lire sous le prisme de sa propres. Contemporanéité. Le législateur n'a pas n'est pas un historien et l'historien n'est pas législateur le législateur est un créateur de droit et ne peut se permettre l'erreur de créer du droit avec du sentiment réhabiliter collectivement, c'est prendre le risque de mettre sous un seul et même drapeau déserteurs innocent traître mutilés volontaire si la justice est individuelle, y compris dans ses erreurs. L'amnistie elle aussi doit doit être individuel de nouvelles réhabilitation au cas par cas sont sans doute encore possible et même nécessaire. Chers collègues, connaître et comprendre l'histoire des fusils est essentiel, il est heureux que depuis 25 ans leur sort et dans toute sa complexité très largement réintégrer la mémoire nationale de la Grande Guerre. Je vous remercie. La parole est à monsieur Marc la Mini pour le groupe Les Républicains pour trois minutes, chers collègues. Oui merci madame la présidente, madame la ministre sur le président de la commission des affaires étrangères et Défense. Monsieur le rapporteur, président Gontard. Chers collègues et je souci aussi la présidente madame Guy Days. Puisqu'on a. Au sein du Sénat, Groupe d'études du monde de combattants qui aussi. Réfléchit à elle intervient aussi dans beaucoup de domaines. Dans le cas du devoir de mémoire en particulier et merci également à nos collègues du groupe geste. Dans leur espace réservé d'avoir consacré du temps pour cette proposition de loi. Adoptée présentée par différents. Plusieurs députés de différents groupes. Et qui a été adoptée le 13 janvier 2022 à l'Assemblée nationale et qui vise à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple, durant la première guerre mondiale, mondiale. Sujet particulièrement sensible historiques comme cela été rappelé par monsieur le rapporteur. Et puis un certain nombre de collègues qui sont intervenues précédemment. Sujet hautement sensible et il convient aussi de replacer les faits dans le contexte le la première guerre. Mondiale qui a mobilisé. Des dizaines de millions d'hommes dans le monde. Et malheureusement aussi des millions de morts des deux blessés et plusieurs centaines de milliers de veuves orphelins et. Mutilé. Ferait référence aussi. Dans le cas du devoir de mémoire. Et puis je. En tant que rapporteur de la loi de finances. Lien avec la nation, mémoire. Monde combattant. Référence aussi à la Mission du centenaire. 2014 2018 où là aussi il y a eu un travail important dans nos territoires et départements respectifs. Et je crois que là, ce travail a été particulièrement important. Avec tous les participants et les représentants des associations patriotiques de mémoire Proposition de loi réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Donc au nombre de 639. Soldats. Et c'est vrai que dans le département des Ardennes que je représente. Avec ma collègue sénatrice, j'ai pu, on a pu aussi rencontré un certain nombre de. D'associations de collectifs a ordonné notamment la Ligue des droits de l'homme. Et différentes associations. Que nous avons rencontrés il y a un an environ. La notion de devoir de mémoire, de respect, de reconnaissance l'été largement. Rappelé depuis de nombreuses. Années il y a aussi de différentes actions qui ont été rappelés rappelés avec les plus hautes autorités de l'État qui sont aussi intervenu et aussi différents veut qui ont été. Déposées par des collectifs dans au niveau des collectivités territoriales, je comprends la position respecte la poussière sa coalition de Madame la Ministre mais à titre personnel, je voterai cette proposition de loi. de loi. Madame la ministre, vous avez demandé la parole. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la présidente. J'ai entendu dire que les balles. Et le poteau d'exécution été facturé aux familles. Enfin soyons sérieux. C'est faux et vous le savez. Les bâtons, des faits pas des idées reçues. Les frais de justice qui existe toujours d'ailleurs et sont mis à la charge de la partie condamné, vous le savez. Ensuite. Chacun des orateurs qui a dénoncé les conditions dans lesquelles cette justice de guerre a été rendu à raison. Je l'ai dit. Ce constat ne fait plus débat. Il nous rassemble. Ce n'est plus de cela dont nous discutons. Pas plus que des fusillés qui avaient été tiré au sort, car cela je l'ai dit dans mon discours ont été réhabilités. Les nombreux exemples cités à la tribune vers les orateurs sont tous bien connus. Et tout aussi révoltants. Mais ce qui nous divise ici. C'est seulement la méthode. Pour achever de réintégrer notre mémoire. Le sort de ces hommes. Il ne peut y avoir. De réhabilitation collective. Je vous remercie. la discussion générale est Close. La commission n'ayant pas élaboré de texte nous passons la discussion des articles. Que de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et à l'article premier j'ai plusieurs prises de parole, monsieur le président, Christian Cambon. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, avant que s'engage la discussion générale suivie suivi de. Du vote. Je voudrais tout d'abord me féliciter qu'un débat aussi dramatiquement sensible, puissent intervenir dans des conditions de dignité qui font honneur à cet hémicycle et je voudrais remercier les orateurs, quelles que soient les les positions qui ont été prises. Nous avons examiné ce texte en commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées le vote vous le savez a été négatif, c'est-à-dire que cette proposition a été refusée par 20 voix contre 17. Ce ne. Cela ne signifie pas que la position des sénateurs qui se sont exprimés contre ce texte est un rejet ou une manifestation d'un mépris car tout le monde est bien conscient que cette épouvantable affaire qui recouvre certainement des injustices. Effrayante. Doit être. Prise en compte mais effectivement. Comme le gouvernement l'a rappelé, comme un certain nombre d'entre vous l'ont rappelé. Nous ne pensons pas que cette méthode qui vise à à revisiter s'entend après. Par une assemblée. Parlementaire règle un problème qui certes relève de l'histoire, même si bien évidemment ils mettent aussi en cause ces événements. Donc je voulais simplement. Dire que dans ce débat, c'est le signe que nous sommes ici dans au Sénat en mesure d'évoquer des problèmes aussi douloureux que ceux qui. Ont marqué notre histoire sans que. La tenue du débat rails et je voulais remercier chacune et chacun, et je pense que cette attitude nous conduira jusqu'au vote final. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à monsieur Tissot. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais m'adresser à mes collègues les plus réticents à voter cette proposition de loi de réhabilitation en insistant sur le, sur ce qu'elle n'est pas cette proposition de loi ne vise pas réhabiliter des traîtres, des espions ou des déserteurs c'est ceci ne figure pas sur la liste des 639 fusillés pour l'exemple de la première guerre mondiale. Beaucoup de ces condamnés pour refus d'obéissance ou abandon de poste on en réalité commis des actes bien compréhensible comme s'endormir à son poste se replier parce qu'on a plus de munitions méconnaître à Nord qu'on n'a pas entendu ou pas compris il y a 2 ans nous commémorons dans mon département la Loire la réhabilitation des six martyrs de 20 gré aux côtés du maire dans bière les des descendants de 2 d'entre eux. Natif de cette commune engagée en 14 dans la défense du village de Vatry Ils ont été fusillés bon pour abandon de poste parce qu'ils avaient obéi à l'Ordre de repli de leurs sous-, lieutenant si les fusillés de 20 gris ont été réhabilités en 1921 639, à une famille attend toujours que cette marque d'infamie puisse être enfin effacer cette proposition de loi ne vise pas à réécrire l'histoire. Monsieur Antoine Prost, président du conseil scientifique de la Mission du centenaire là parfaitement écrit dans son rapport je cite l'histoire des fusillés de 14 18 ne réserve à nos yeux aucun mystère. Mais la question posée est celle de la mémoire on veut conserver la nation, c'est à elle de s'en saisir et c'est exactement ce que nous faisons avec ce texte et propositions de loi ne vise pas à ternir l'histoire de notre pays et de son armée, tous les protagonistes de cette guerre, ont prononcé des sentences de mort dans des conditions similaires. Nos alliés néo-zélandais canadiens et anglais ont réalisé de travail que nous engageons aujourd'hui en amnistiant ou réhabilitant leur fusillés notre pays, s'honorerait lui aussi à tourner cette page de son histoire. Enfin et c'est peut-être le plus important. Cette proposition de loi ne ternira en rien la mémoire des soldats honorés chaque 11 novembre, comme nous l'indique encore Antoine Prost. Les soldats revenus nous du front. C'est avant tout ce qu'ils appelaient les embusqués des planqués et les profiteurs pas ce qu'il avait subies à leurs côtés de grands massacres en tant que législateurs, nous avons la possibilité aujourd'hui de réunir enfin dans notre mémoire collective et sur nos monuments, ces hommes qui ont combattu côte à côte mais et qui ont perdu la vie. Cher. Merci la parole est à monsieur. Merci madame la présidente. Je m'exprime évidemment en tant que sénateur mais aussi en tant qu'agrégé d'histoire et citoyens Picard à ce que l'Aisne, l'Oise et la Somme ont été particulièrement meurtrie par ces combats mais la France entière a été meurtri n'a, n'est pas une seule famille dans notre pays qui n'a été touché, soit parce que ces ces perd ses fils ont été mobilisés, blessés, tués. C'est un débat effectivement particulièrement douloureux, personne ici ne peut accepter le déni de justice qu'a constitué. Ces punitions collectives. Une punition collective et par définition aveugle. Or sur les 639 cas évoqué chaque cas étaient particuliers. Avec certains héros qui ont été fusillés. cet homme de ces hommes n'étaient ni des traîtres, ni des lâches. C'était des conscrits ce n'était pas des militaires de carrière. Alors effectivement. Nous avons envie de tous les voir réhabiliter mais. Autant la punition collective est injuste. Autant la réhabilitation collective qui met sur le même stade. Certains héros qui ont été ignoblement. J'ai un cas dans l'Oise, l'officier, plan qui a été fusillé a crapaud Mesnil. Sur son brancard. La punition collective est injuste la réhabilitation collective en mettant sur le même plan. Ceux qui ont trahi et ceux qui ont été trahis, n'est pas la solution. Alors quelle est la seule solution. La seule solution. Mais si vous aimez les. C'est. Que nous avons des étudiants en histoire. Qu'on doit faire travailler sur tous ces cas et qu'individuellement, nous pouvons les réhabiliter encourageons nos universités nos directeur de recherches à faire des recherches sur chacun des 639 cas fair-play réhabilitons individuellement. La parole est à monsieur Dantec. On doit écoutez merci hein. Madame la présidente. Je je pense que nous sommes en train de faire fausse route. Vous imaginez qu'on est en train de dire que parce que dans les six ans il y en avait peut-être quelques-uns qui était coupable. Je ne sais pas si c'était Coupable de la peine de mort, on ne peut réhabiliter personne. C'est ce que vous défendez depuis. Le début de cet après-midi c'est profondément injuste profondément injuste puisque nous savons que nous n'avons plus de possibilités de d'examiner les les 600 cas surtout je pense que nous faisons fausse route sur le fait que ils ont été fusillés pour l'exemple. Ça je crois que personne ne le remet en cause par une décision politique. Parce qu'il fallait éviter effectivement que l'armée française recule. Ils ont donc été fusillés pour la France, c'est pour la France qu'ils ont été fusillés. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie comme ce qu'on a envoyé prendre des tranchées infranchissable. Ils ont été fusillés par ce qu'il fallait gagner la guerre et ils ont payé de leur sang. Le fait qu'il fallait gagner cette guerre les réhabiliter. Aujourd'hui ça n'est pas regarder des cas individuels, c'est regarder la décision prise par l'armée et l'État français qui a considéré que face au risque d'effondrement du front, il fallait faire des exemples. Les réhabiliter aujourd'hui c'est aussi réhabiliter finalement la décision de l'armée française et de l'État français qui a considéré que dans le moment que nous vivions à ce moment-là, il fallait des exemples et ils ont payé de leur sang pour la France le fait que l'État et l'armée a considéré qu'il fallait effectivement ces exemples les réhabiliter. C'est donc réhabiliter aussi l'armée française et pas seulement travailler sur des injustices individuelles. Merci. La parole est à monsieur t'es mal. Merci madame présente mes chers collègues. Moi je voudrais aborder 2 points le 1er c'est sur les 639. En fait, les 130 hommes ne sort pas du chapeau comme ceux-là, c'est le rapport du service historique des armées qui dit très clairement. 639 fusillés pour l'exemple. Et les autres, ceux qui sont les traites. C'est un autre cas ceux qui ont collaboré, enfin qui ont refusé et etc. Donc en fait on est sur une chose très cadré. J'ai envie de dire, on se base sur un document du service historique des armées. Donc je veux bien qu'on ait tout débat mais j'chers collègues c'est c'était bien si rentres plein donc, je crois là dessus il y a pas de fausse polémique. À voir, on est pour les comptes, mais ne jouons pas sur une ce pseudo-incompréhension, ça c'est le vrai point 2ème point c'est pour un sujet de cohérence. Je l'avais dit en commission. Certains disent il ne faut pas il ne revient pas au Parlement d'écrire l'histoire.

Pour ceux qui voteront chers collègues tu ne la votera pas je la voter, qui évoque des jeux aussi dans d'autres pays. Qui de fait, fait que le Parlement français, écrit l'histoire, mais dans d'autres pays mais bizarrement refuserait à chaque fois d'ouvrir l'histoire dans notre pays. Donc il faut qu'on ne soit cohérent. Si nous refusons d'ouvrir et c'était le débat d'ailleurs sur ce qui avait été évoqué sur le 17 octobre 61. Et sur aussi une proposition sur le 5 juillet sont de notre collègue Boyer ne veut pas dire à la fois là on a on a grand refuse de de les traiter et puis quand il s'agit d'autres pays étrangers, là par contre on écrit leur propre histoire. Donc j'invite à la cohérence. C'est pour ça que moi en étant cohérent je voterai c'est toi là comme je voterai celle de la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci la parole est au président Patriat. Ah ben oui bien entendu, mais là on était dans les prises de parole sur l'article. D'accord.

Excusez-moi, Monsieur Patriat, madame la présidente. Je voudrais essayer de répondre aux principales réserves voire désaccords que j'ai entendu et qui sont entendable. Non il est pas question ici de se substituer aux historiens, les travaux de ceux-ci sont consensuels sur ces fusillés pour les en l'exemple et encore plus nettement avec l'oeuvre de synthèse. Antoine Prost a effectué à l'occasion du centenaire. On n'a donc pas prétendre ici à départager différentes lectures historique mais plutôt à en prendre acte. Depuis le 1er ministre Lionel Jospin jusqu'au président Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'exécutif a fait avancer la démarche qui donne dans notre mémoire collective nationale la place qui est dû à ces centaines de fusiller donc après que l'exécutif a fait sa part il revient au Parlement de conclure d'une certaine façon ce qu'il avait entamé dès 1916 en mettant résolument en cause les modalités de ces conseils de guerre spéciaux bien plus napoléonien que républicain. Alors oui réhabiliter tous ceux qui ont subi sommairement le choix désastreux des autorités. D'alors d'en passer par cette forme injustifiable de justice expéditive destinée à impressionner la masse bien plus qu'à sanctionner chacun en connaissance de cause. Alors bien sûr cette réhabilitation s'interprétera de façon souple, nous n'allons pas formellement invalidés les quelque 639 décisions de justice et c'est justement là à mon sens, la force de cette proposition de loi son profit évident. Hé oui parce que, puisqu'il s'agit de mémoire nationale elle pèsera je crois avant tout comme message à la jeunesse, la mienne ma jeunesse, elle a été marquée, elle a été révoltée par les sentiers de la gloire. Ce film qui a dû attendre, rappelons-nous 18 ans pour être projeté en France. Je crois qu'il faut permettre aux jeunes générations de mieux saisir combien la nation, la République va parler au fait par les valeurs mais aussi par la reconnaissance des zones d'ombres. Merci. Alors je pense que là, nous pouvons passer donc à l'amendement numéro un. Et Monsieur le Président Patria. Je pense que là vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame Hennis, messieurs, mes chers collègues. Oui c'est vrai vous l'avez évoqué tous avec talent avec émotion. Je crois que ce sujet est un sujet douloureux qui nous interrogent tous et j'ai bien entendu de part et d'autre, quels étaient les arguments les éléments. Qui permettait de vous prononcer à l'issue de notre débat. Je comprends moi néanmoins pourquoi la solution de compromis que nous avons proposé. À Rossi, un accueil aussi méprisable. Je ne comprends pas parce que à l'issue de nos échanges avec les historiens et les associations. Notre groupe a souhaité défendre un amendement de réécriture de l'article 1. Cet amendement propose une réintégration dans la mémoire nationale des 639 fusillés dont nous parlons aujourd'hui plutôt qu'une réhabilitation collective et générale qui se heurterait à des obstacles à la fois historique et juridique. Donc les 639 monsieur es mal, ils sont bien pris en compte dans notre amendement il propose également qu'un monument national soit érigée à leur mémoire. nous aussi nous avons pensé que par cet amendement. Ne ce texte pouvait suivre son chemin et habite et aboutir à une forme de réhabilitation de ces gens qui ont été injustement fusillés. Mais force est de constater, mes chers collègues.

fin de non-recevoir, force est de constater que cet amendement de compromis a été massivement rejeté en coupe en commission sans qu'aucun groupe aucun mes chers collègues. Ne prenne la peine d'expliquer les raisons de ce rejet, alors j'ai compris, a compris que ce mot d'amendements avait peu de chances d'aboutir. et qu'à la fin de la discussion générale, il n'y aura aucune majorité qui se dégage pour le faire adopter. C'est la raison pour laquelle, alors que ce notre amendement permettait d'avancer je remets, je retire notre amendement, regrettant que ce texte ne puissent pas aller plus loin, je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix donc l'article 1er, si cet article n'était pas adopté, je considérerais que le vote est le même pour l'article 2 qui est un gage. En conséquence, c'est l'article 1er, n'était pas adopté. N'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi dans la mesure où les 2 articles qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble. j'ai été donc saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'article 1er. Ah oui pardon. Oui bien sûr je suis désolée.

fort un sujet lourd. Oui il y a de l'émotion. Mais je pense comment on peut pas avoir d'émotion à travers les descriptions qui a pu qu'il ait pu avoir. Mais c'est un débat qui a eu le lieu à la fois en commission à la fois de manière oui, on sait tous ce respecter dans dans nos choix et en tout cas dans notre manière d'aborder cette ce sujet cette et cette question. De avec sérénité et donc moi je trouve que ça montre justement qu'on peut aborder ce sujet. 100 ans après. Justement, on voit bien que ça ne réouvre pas des des brèches au contraire et qu'on a besoin aussi de clôturer. Et je pense que c'est un petit peu le le sujet qui est devant nous et avant de voter. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait par des historiens. Un travail approfondi et je dirais nombreux. Et ses 639 ils ne viennent pas de nulle part et c'est justement ce travail des historiens et l'historien nous le disent, on a fait notre travail, maintenant à vous de politique, de faire le vôtre et de je dirais conclure peut-être de tourner la page parce qu'on sait aussi que ce texte qui a été. De Bastien Lachaud qui a été votée à l'Assemblée nationale. Si on ne le vote pas aujourd'hui si on ne le vote pas conforme. On sait très bien qu'on repoussera et que ce sujet, on ne le reverra plus et derrière ben c'est 639 personnes qui. Effectivement leurs familles qui attendent quand même cette réhabilitation donc voilà j'entends que en tant que rapporteur de de ce texte. J'entends l'avis de la commission. Les débats qui a eu, on les a. Très bien très bien décrit, mais je pense qu'on a un moment assez fort pour effectivement marqué peut-être un point un terme à cette. Cette histoire importante de notre pays. Voilà, merci. Merci monsieur Vaugrenard. Merci madame la présidente, je ai simplement. Rajouter par rapport à l'intervention de notre collègue François Patriat que l'amendement. N'a pas été défendue par tout le monde. Il a été argumenter sur le fait que voter compte parce que c'était un artifice, nous le savons bien de procédure. Parce qu'à partir du moment où le texte été modifié. Ça signifie qu'il repartait à l'Assemblée nationale et qu'on en repartait probablement pour plusieurs années. C'était ça le fond de la question. Donc nous avons émis un avis défavorable par rapport à l'artifice qui étaient proposés et chacun le sait. Sur la réhabilitation pour l'exemple. J'essaie de, de m'imaginer ce que peut penser notre jeunesse d'aujourd'hui par rapport à nos j'ai changé à nos débats. Je me félicite, comme le président de la commission là j'ai rappelé tout à l'heure que ce débat en commission a été de haute tenue extrêmement intéressant et que chacun a pu en tirer des des des bénéfices. Je veux simplement dire que concrètement aujourd'hui lorsqu'il y a des dépôts de gerbe. Le 11 novembre, notamment en particulier dans l'ouest de la France. Eh bien il y a des dépôts de gerbes, qui sont faits par les responsables du Souvenir français. Et des dépôts de gerbes, qui sont faits ensuite par les associations qui défendent la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Voilà concrètement ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et j'essaie d'imaginer aujourd'hui ce les enseignements que pourrait tirer notre jeunesse le jour J 18, 20 25 ans. Alors les historiens ont fait leur travail, ça a été rappelé. Ils l'ont bien fait, parfois ils sont en désaccord. Non seulement par rapport aux propos qui ont été tenus tout à l'heure mais eux-mêmes, disent que la réhabilitation au cas par cas juridiquement n'est plus possible. Parce que nous n'avons pas d'éléments de preuve. Et donc il s'agit manifestement d'une décision politique par rapport à notre histoire et nous dans notre pays comme dans d'autres pays, hé bien nous avons parfois fait des erreurs

quand je dis merci, c'est que c'est fini monsieur. Franck Renard madame Gréaume. Ben si si justement Monsieur Vaugrenard, est-ce que vous pouvez penser aux autres collègues qui attendent le texte suivant, je je vous demande ça merci et c'est moi qui décide. Merci. Même Gréaume, c'est à vous l'. Merci madame la présidente. Nous sénatrices et sénateurs. Nous avons l'occasion unique aujourd'hui de clore un chapitre douloureux de notre histoire. Au-delà de nos différences et nos sensibilités soyons unis, pour être aux côtés de ces fusillés pour l'exemple. Vous savez très bien comme moi qui a plus de témoins. C'est plus de 100 ans après la guerre et que 20% seulement des dossiers ont été retrouvés. Donc. Pensez à tous ces gens, tous ces gens qui ont vécu dans des situations excessives ces moments et qu'ils ont été jusqu'au bout, d'eux-mêmes. Hé ben ces gens-là il faut les réhabiliter et si on veut du cas par cas. Vous savez comme moi qu'on réhabilite 3 personnes. Et là, on en prendra la responsabilité. Merci, cher collègue, Monsieur t'es mal. Merci madame, je voudrais répondre un peu à mon à mon cher ami le président Patriat. Moi j'entends de venir là et dire. Mon amendement n'a pas été pris en commission, c'est du mépris non c'est c'est un vote donc c'est pas du mépris peu tiens petite de je le retire mais en fait quand la loi est adoptée à l'Assemblée contre la montée du gouvernement. On aurait pu attendre même encore après l'inscription aussi que le gouvernement ne dise voilà, ne faites pas ce texte là. Mais je vous fasse une, je fais une autre proposition.

c'est qu'il y ait une vraie proposition de madame la ministre, en disant voilà j'ai entendu ce que vous dites, voilà ce que je peux faire mais nous savons aujourd'hui tous ensemble que la réputation individuelle parce qu'il a pu dossier n'impossible on la seule chance que nous avions c'est nous appuyer sur un travail encore une fois fait par le service historique des armées il y a refus ne prenons acte, mais franchement, ne jetez pas là ne je n'pas la faute sur les autres.

un problème juridique à l'égard de cette PPL et vous le savez et ça je le dis bah je l'ai expliqué. Alors si vous n'écoutez pas les arguments et il y a il y a une méthode le le Royaume-Uni le Royaume-Uni si je peux me permettre Monsieur mal le Royaume Uni a fait passer un texte ouvrant à la réhabilitation de plus de 300 fusillés pour l'exemple, ils ne l'ont pas fait par un acte. Je dirais parlementaire. Ils ont institué une juridiction spéciale qui a procédé à cet acte parce qu'au Royaume-Uni, comme en France il y a une distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors si on veut éviter le cas par cas fait une proposition dans ce sens j'ai ôté auteur de PPL qui ont été qui ont connu un changement un invariant sur un bout d'article en lecture à l'Assemblée nationale, hé bien je l'ai repassé conforme au Sénat. C'est le jeu parlementaire, alors arrêtez de parler d'artifices. De procédure. Ce n'est pas un artifice de procédure il est argumenté et je constate que personne lorsque j'ai présenté en commission cet amendement n'a expliqué la raison de son vote contre. Merci. Merci Monsieur Bénard Roche. Madame la ministre, après après. Merci madame la la présidente. je voudrais revenir quand même au fond du débat aujourd'hui qui n'est pas le fait que l'amendement soit un amendement. De de procédure ou pas. En fait, cet amendement, il a été rejeté par la commission, il a été rejeté par la commission. Voilà donc comme tous les amendements ici qui sont rejetés par les conditions sont pas forcément des amendements d'artifice et pour autant on ne peut pas se plaindre d'avoir été victime d'une sorte de de de d'injustice et les commissions décide des amendements qu'elle qu'elle va en tout cas elle vote pas voilà. Pour revenir sur le fond du texte. Les textes qui présente à la fois. La capacité de nous unir au sein de cette assemblée totalement d'une manière transpartisane et qui nous paraissent essentiels au rétablissement d'une certaine mémoire de notre pays sont excessivement rares ici. Nous sommes devant le texte de cet acabit. Aujourd'hui nous avons la possibilité de dire notre pays le Sénat les les parlementaires de notre pays puisque les députés leur déjà fait. Rétablisse. La le réhabilite la mémoire d'un certain nombre de condamnés dont on sait parfaitement bien qu'ils ont été condamnés pour des motifs qui étaient des motifs juste d'exemplarité. Par rapport à une situation et un contexte de guerre et qu'ils n'ont pas été condamné pour des faits réels, qu'ils ont commis. Il est impossible artifice réel c'est celui qui consiste à dire on va étudier, cas par cas. L'étude cas par cas, a déjà été fait, ça a été rappelé. Elle a été, ça a été fait et il n'est pas possible de la pousser plus loin, il n'existe plus de dossiers. Donc, dire on va étudier, cas par cas consiste à dire on ne réhabilite a jamais aucun de ses 623 personnes c'est l'honneur de l'armée et l'honneur de la France que de réhabiliter aujourd'hui les 623 personnes dont on sait qu'ils auraient été condamné pour l'exemple. Merci madame la ministre.

Alors il y en a plus de 40 à peu près qui ont été réhabilitées, donc on n'est plus à 639 mais peu importe. Sur le fond, ce que je veux vous dire. C'est que. En l'état. Ce projet. Me semble très dangereux car il modifie des décisions de justice ce qui est probable c'est ce qui est problématique en soi. Il le fait de manière indistincte en méconnaissant la réalité concrète des décisions de justice en l'état. Il permet de réhabiliter François M.. Fusillé le 22 octobre 1915 pour désertion et abandon de poste devant l'ennemi. Il appartient à la liste des 639 dont nous parlons depuis ce matin. Évoquée par la proposition.

Qu'il pense que la meilleure des solutions en la matière législative et de ne rien faire et puis pour terminer. Vous êtes législateur. Nous ne sommes pas un tribunal. Et nous devons absolument. Continuez à respecter la séparation des 2 assemblées et de la justice. Je vous remercie. Merci. Alors je vais donc. Procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Merci. Plus personne ne demande à voter le scrutin est clos. Un nombre de votants 342 exprimés, 331 pour, 113 contre, 218 voix. Donc c'est l'article 1er rejeté. Il en est donc de même de l'article de un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a plus de texte en conséquence la proposition de loi n'est pas. Adoptez.

La séance. Prise à l'ordre du jour appelle la suite de la discussion, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Visant à protéger les logements contre l'occupation. Illicite. Dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement numéro 78 au sein de l'article 1er, ah je vais demander à tout le monde, de rejoindre sa place ou de sortir de l'hémicycle. Nous avons 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 78 à monsieur boîte. Merci madame la présidente. Cet amendement on demande tout simplement qu'il le. Est-ce que vous pouvez sortir de l'hémicycle a président Gontard. Merci. Discussion à l'extérieur. Merci monsieur Bois-d', excusez-moi. Pardon, madame. Il s'agit tout simplement dans cet amant demain on demande tout simplement nous d'instaurer, c'est un nouveau délit qu'on met en place a parfaitement inutile qui permet de lutter contres les squats, mais qui n'aura aucun effet dissuasif et dont la répression est déjà prévue par les dispositions claires équilibrée de l'article 226 IV du code pénal. Cet article. La disposition suivante choquante. Il est parti comme un inquiétant que soit envisagé la criminalisation des personnes ayant occupé légitimement un lieu d'habitation qui rencontreraient des difficultés de paiement de leur loyer. L'introduction d'une peine d'emprisonnement à Paris la situation est véritablement scandaleuse. Un projet des poursuites judiciaires. faire condamner les plus démunis d'entre nous en particulier à une amène de à une amende de Tommy 7500 euros est complètement immoral et dès 2 ans, a certainement pas amélioré la situation des plus difficiles. Permettez-moi d'ajouter le je vois mal comment un propriétaire d'ailleurs qui réclame des impayés sera aidée par la croissance avant de la dette.

Merci madame la présidente. Donc c'est cet article contient plusieurs. Dispositions notamment concernant l'entrée par effraction dans certains lieux. Alors il s'agit effectivement de situations qui peuvent. Exister mais quand même. Qu'il demeure très minoritaire dans les 17.000 expulsions exécutées en moyenne chaque année il y aurait donc 3 millions de logements vacants et 300.000 personnes sans domicile fixe. Si on fait le calcul, il y a donc 10 logements vides pour une personne SDF certes cela ne légitime ni le recours à la force ni même l'atteinte au droit de propriété mais quand 300.000 personnes sont à la rue n'est-ce pas aussi problématique, voire plus grave encore de laisser 3 millions de logements vides. Chaque année entre 500 et 600 personnes meurent de sans-abrisme. Ce sont parfois. Des enfants le plus jeune avait je le rappelle un mois en 2021. J'entends que vous voulez faire référence à des petits propriétaires ils sont minoritaires parmi les propriétaires de logements, puisque 3% des produits propriétaire possède 50% du parc locatif. Ils ont chacun au moins 5 logements, eux, ne sont pas des petits propriétaires mais profite de quelques faits divers médiatisés pour vous faire porter des lois comme celle-ci que je qualifie de rétrograde et ainsi mieux protéger l'Europe. Mais je dois dire que. Nous avons entendu, vous ne voulez pas de squatters. Moi non plus. Mais ne condamnons pas les locataires en impayés de loyers à de la prison la prison ne leur apportera rien elle ne sortira personne de la précarité, bien au contraire. Ne faisons pas ici l'amalgame entre la preuve la pauvreté et la criminalité ne créons pas un nouveau délit de vagabondage si anachronique et dramatique pour notre modèle social. Nous vous proposons donc de supprimer la peine de prison pour les personnes qui n'auraient pas payer leur loyer et qui ne quitte pas le logement de leur plein gré, je vous remercie. Monsieur Bénard Roche pour le 34. Oui madame la présidente. Nous étions prononcés pour la suppression de certains articles à qui pénalise qui criminalise les locataires dès lors qu'ils ne trouvent pas à se reloger qu'il se maintiennent dans le logement après une décision de justice d'expulsion. notre amendement n'a pas été voté donc l'article à tel qu'il se présente aujourd'hui prévoit non seulement une peine d'amende augmentée, mais il prévoit également une peine d'emprisonnement pour le délit d'occupation frauduleuse de local à usage d'habitation dans le cas de locataires qui ne peut pas payer et qui se maintient après une décision d'expulsion. Nous voulons par cet amendement dire très clairement que nous ne souhaitons pas. Que la prison pour dettes. Qui est une sanction qui est banni de la République depuis des années, qui se trouve aujourd'hui dans les oubliettes de notre justice soit rétablie pour cette dette là et uniquement pour cette dette nous supprimons donc ce par cet amendement uniquement la peine d'emprisonnement même si nous ne sommes pas d'accord sur le fond y compris avec l'augmentation des amendes. Cet amendement consiste uniquement à supprimer a minima l'emprisonnement.

monsieur Besnard Roche. Vient de le présenter pour son amendement. Il s'agit effectivement de la même demande qui est que. Si on peut envisager lorsqu'il y a effectivement, occupation d'un squat où quand il y a effectivement. Enfin voilà une réalité. Tu es qui. Pour mon sang se justifie qu'on aille jusqu'à l'emprisonnement. Il me semble que même si effectivement on doit sanctionner quand on arrive à en fin de processus fortement un locataire défaillant qui après les nombreuses années de procédure n'est toujours pas en situation effectivement d'honorer sa dette malgré la situation. Il me semble qu'effectivement je ne suis pas sûr que six mois d'emprisonnement change cette réalité et si je peux me permettre rappeler aussi que il peut arriver que des locataires défaillance quand ils sont de mauvaise foi ou quand ils ont. Effectivement accumulé un certain nombre de difficultés. Et quelquefois fois aussi dégradé leur logement et à ce moment-là on peut s'interroger effectivement sur la nature de la sanction, on peut envisager l'emprisonnement et dans ce cas particulier qui pourrait justifier peut être des sanctions plus difficile le code pénal prévoit déjà un arsenal de sanctions. Donc il me semble complètement inutile et contre-productif d'aller jusqu'à l'emprisonnement. Mais par contre maintenant la sanction financière de 7500 euros, même si je pense qu'effectivement ce sont des familles en difficulté. Il faut malgré tout à un moment donné signifier une sanction minimum et pour ma part, voilà c'est quelque chose qui trouverait un compromis entendable et pour moi, effectivement, aussi je pense que la prison pour un locataire défaillant, c'est quand même autre chose qu'effectivement s'être emparé du bien d'autrui de façon illicite totalement illicite et ça paraît encore une fois une solution. Qui paraît juste, équilibré, sans ignorer et sans être dans l'impunité. Merci. L'amendement 60. Même la présidente Assassi. Oui alors. Donc effectivement. Il est proposé ici de la prison ferme pour. Les locataires ayant reçu un jugement d'expulsion. Je voudrais simplement que vous sachiez que pour être reconnus prioritaires à un relogement otite du droit au logement opposable d'. Il faut notamment justifier d'un jugement d'expulsion. Or une fois que vous avez le jugement d'expulsion il faut plusieurs mois, nous connaissons bien ça. Partout, notamment en Seine-Saint-Denis. Monsieur le Ministre, hein. Or une fois que vous avez le jugement d'expulsion. Donc il faut plusieurs mois à la commission de médiation pour vous reconnaître prioritaire. C'est à ce moment-là que cette loi va poser problème, certains pourront être mis en prison avant même d'avoir pu faire valoir leurs droits puisque puisqu'après 2 mois à rester dans le logement, vous pourrez être enfermé en prison. prison. Quand même un problème. Une condamnation pour expulsion est déjà un gros frein. Cela a été dit pour pouvoir retrouver un logement par la suite auprès d'un bailleur c'est aussi paradoxalement une nécessité pour pouvoir être reconnus prioritaires au titre du Dalo. Nous voulons proposer donc du sursis pour les personnes qui risquerait la prison pour le maintien dans un logement en considérant notamment que c'est l'absence de propositions et la longueur des démarches. Qui mène à ce que certains restent illégalement dans le logement, mais il n'y a pas de logique, je le répète à enfermer en prison ces ménages en difficulté Sont quand même déjà bien remplie et ce n'est pas de toute façon derrière les barreaux, que les locataires pourront mieux rembourser leurs bailleurs. Le sursis pourrait pourra apparaître comme un avertissement pour les mauvais payeurs qui serait récidiviste pour la très grande majorité ce n'est pas un principe de vie de ne pas payer son loyer, mais surtout une conséquence d'une perte de revenus importante en compte, de le prendre en compte comme telle. Et de proposer du sursis, plutôt que de la prison ferme. Merci. Alors l'avis de la commission. Cette fois-ci. Monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Alors sur le 78. Nos collègues du groupe socialiste propose de supprimer l'infraction prévue pour sanctionner le maintien sans droit ni titre dans un logement. Il nous semble à la commission que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et bien encadré. L'infraction s'appliqueraient seulement après un jugement définitif d'expulsion à l'expiration de tous les délais accordés par le juge en dehors de la période hivernale et elle ne concernerait pas les locataires du parc social, vous l'avez certainement lu comme moi. Par ailleurs, nous faisons confiance au discernement des parquets qui n'engageront naturellement des poursuites que si c'est justifié au vu des circonstances. Compte tenu de toutes ces garanties. Je pense que nous pouvons conserver le dispositif voté par l'Assemblée nationale et donc rejeter cet amendement de suppression avis défavorable. Nos collègues du groupe CRCE présente un amendement qui poursuit le même objectif que l'amendement que je viens d'examiner. Il appelle donc le même avis défavorable. L'amendement. Les 2 Les 2 amendements 34 et. 82 rectifié bis sont différents. Ce sont des amendements. Qui. Tendent à supprimer la peine d'un coup d'emprisonnement encourues en cas de maintien sans droit ni titre dans un logement après une décision définitive d'expulsion pour ne maintenir qu'une peine d'amende. Je voudrais rappeler à nos collègues que les peines d'emprisonnement, d'une durée égale ou inférieure à 6 mois sont en principe toujours aménagée. Je ne crois donc pas que l'application de cet article aboutissent à envoyer beaucoup.

Je suis sensible à la dimension symbolique qui s'attache à l'existence d'une peine d'emprisonnement. J'ai entendu aussi naturellement les observations des uns et des autres et notamment des associations qui défendent. Ces personnes, beaucoup d'associations d'aide aux mal-logés perçoivent cette peine comme une forme de stigmatisation et c'est la raison pour laquelle nous donnons un avis favorable. Voilà c'est bien d'entendre hein. Bravo. De temps en temps. Le dernier. Amendement et le 60. Et là aussi, on comprend bien l'intention de nos collègues qui veulent éviter que des locataires défaillants soit envoyé en prison. Vous avez compris que l'amendement ne peut pas accepter car la prison avec sursis ne peut pas constituer une peine en soi ça n'existe pas et de toute façon il tombe comme je viens de le dire avec l'avis favorable sur les deux amendements précédents. Je vous remercie. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, bonjour. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Donc comme ça vient d'être rappelé les deux premiers amendements le 78 et le 59 vise à supprimer le délit pour un locataire qui se maintient sans droit ni titre dans un local d'habitation et les deux autres le 34 et le 82 supprime uniquement la peine de prison comme ça. Autre ici été soulignée par monsieur le rapporteur. Les débats parlementaires avaient déjà bien un améliorer le texte à, à l'Assemblée. Nationale. Pour autant, c'est vrai que ce ces délits. De d'occupation sans droit ni titre pour loyers impayés ne relève pas de ce que l'on a vu dans d'autres cas pour pour les squats. Je suis donc. Favorable. Aux amendements, 34 et 82 qui vise à supprimer la peine d'entrer d'emprisonnement. En ne gardant que la peine d'amende. Évidemment ce délit. Même si ça a été dit risquait très faiblement d'être appliqué. Je suis en revanche réservé sur sa suppression. Totale parce que comme ça a été dit. Là les garanties prises en compte tout au long du traitement devrait faire que seules des personnes. De mauvaise foi et et n'ayant pas recouru à tous les voix de de recours seraient sanctionnés mais les situations les plus précaires. Je crois, dans la mesure de des protections qui ont été mises en place ne ne serait pas sanctionné. pour conclure j'aimais donc un avis favorable sur les amendements, 34 et 82 pour le gouvernement, la suppression de la peine de prison et un avis de sagesse sur les deux premiers amendements. Visant à supprimer totalement les articles merci. Merci. Alors, Madame, Goubeli Avec la suppression de la peine de prison. Cet article ne n'a plus à ce stade l'intérêt mais. Merci madame voulez. Oui, mais président d'une minute remercier le rapporteur pour la vie qu'il a donnée sur l'article sur l'amendement numéro 34 que naturellement nous soutenons puisque c'est celui de Valérie. Pagan 82. le 34 aussi d'ailleurs. C'est le même donc il y a pas il y a pas de raison de faire de d'ostracisme pour notre ami Ben Haroche. Nous pouvons aussi soutenir son amendement, d'autant que c'est le même. Voilà. En effet, ça a été dit pendant les débats, la prison n'avait pas beaucoup de, de sens et même en avait un qui était quand même tout à fait insupportable. Et si l'on ajoute en plus la surpopulation carcérale. Franchement tout ça aurait donné une image de la Haute Assemblée. Qui m'aurait fortement déplu. Donc je trouve que cette position est une position de sagesse. C'est une position humaine et c'est une position intelligente, ça ne m'étonne pas de la assemblée. Si, alors je vais mettre aux voix, donc la maman 78 qui a eu un avis défavorable de la commission. Un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ce n'est pas adopté le 59. Même avis même vote. Or le 34 et le 82 identique. Avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc adopté et le 60 tombent. Les amendements. 11 12 13 nous ne sont pas défendus. Amendement 66 même. La présidente Assassi. Merci madame la présidente. J'entends les interventions. Parce qu'il est le le débat qui a eu lieu auparavant sur les squatters sur les petits propriétaires. Nous n'avons rien à opposer aux petits aux petits propriétaires qui sont d'une minorité, je le rappelle, et nous ne soutenons soutenons pas le squat qui ne devrait pas exister dans une société où tout le monde aurait accès à un logement digne. Cependant, la réalité c'est que les personnes en situation d'impayés de loyers sont principalement des personnes ayant connu une perte brutale de leurs revenus après un licenciement ou une fin de contrat. Quand les allocations pour le chômage tarde à être versées ou en fin de droits qu'on c'est le RSA qui tardent à être versées par exemple c'est le cas pour une dépense soudaine également imprévu sanitaire une hospitalisation, bref tout ce que l'on peut appeler un accident de la vie et parmi ces accidents, il y a souvent le départ du conjoint souvent un homme qui crée une baisse brutale dans le budget du ménage. Ce sont donc souvent les femmes qui en sont victimes, une fois de plus, en devenant parents isolés, parfois sans les ressources suffisantes. Cela s'apparente à une forme de violence économique qui est pour nous intolérable et je pense que nous pourrions nous accorder là-dessus donc notre amendement vise simplement, enfin simplement vise Entendez bien pas en les dispensant de payer ou de rembourser ce qui est du mais au moins en leur évitant de subir la fronde être condamné à de la prison ferme ou une amende. Mais du coup ça ne fonctionne plus, si j'ai bien compris. D'autres votes précédents. Merci madame la présidente. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Madame la présidente, ça. Si cet amendement près propose d'exclure du Champ d'application de l'article 1er, ah, ah les femmes qui ne peuvent régler leur loyer parce qu'ils ont subi une perte de revenus du fait du départ précipité du conjoint. Je voudrais d'abord rappeler que la sanction pénale est en cause. Seulement, après une décision définitive d'expulsion et que celle-ci intervient clairement après l'expiration de tous les délais pouvant être accordées par le juge. Dans le type de situation évoquée par nos collègues du groupe CRCE le magistrat pourra tenir compte des circonstances et naturellement accordé à la mer qui se retrouve isolé avec ses enfants les délais qui lui permettrait de retrouver un logement compatible avec le niveau de ses ressources. Il n'est, selon la Commission pas utile ni pertinent d'introduire dans la loi une exception telle que vous la proposer et si vous me le permettez. J'ajouterai volontiers qu'il, qu'il n'y a pas de raison de limiter cette exception aux seule femmes dans la perte de revenus aurait entraîné la lettre la dette locative. À la suite du départ précipité du conjoint. Je connais. Nous connaissons tous. Des hommes qui peuvent connaître aussi une perte de revenus liée au départ précipité de leur conjointe E. Conjointe. C'est la raison pour laquelle nous donnons un avis défavorable avec regret. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. je peux. Évidemment. Partager votre préoccupation sur la situation des femmes mais en l'occurrence comme vient de le dire. Le président de la commission la situation et le rapporteur pardon et est déjà prise en compte à travers les règles de protection des locataires en situation d'impayés. Mettre en place une différence qui me paraît pas tout à fait constitutionnelle en entre un homme et une femme ne paraît pas non plus relevé de de cette de cette assemblée à à ce stade et sur. Sur cet amendement. Donc ce que je vous propose, c'est soit de retirer votre amendement sinon ce sera un avis défavorable. Merci. Alors oui, madame la présidente. Qui sont exclus de leur de leur le logement et qui se retrouvent dans des situations compliquées, mais je crois qu'il faut aussi entende entende ce message sur. Le ces femmes. Qui sont souvent en charge de famille avec des enfants donc à leur charge qui se et c'est une réalité. Je pourrais vous décrire plusieurs situations donc c'est bien de de l'entendre mais j'entends vos, vos arguments à vous monsieur le rapporteur. Et à monsieur le Ministre donc je retire la la Merci. Alors je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient mais donc adopté article 1er bé j'ai deux amendements identiques de suppression le 39 Monsieur Oui merci madame la présidente. Alors cet article 1er bé a été ajouté en fait ici. Et et en en demandant la suppression, en fait, on ne demande pas ni un allégement des peines une suppression des peines au contraire on trouve que l'abondement, qui a été voté ici est un amendement qui supprime la possibilité pour le juge d'avoir la capacité à faire totalement sa fonction, c'est-à-dire à juger même s'il peut accorder ou pas des délais supplémentaires par principe, par principe, nous sommes contre les décisions qui reste Stade les pouvoirs du juge par principe nous pensons que le juge doit pouvoir exercer la totalité de ses pouvoirs qu'il s'agisse de pouvoir de paid a cru qu'il s'agisse de pouvoir de délai supplémentaire. Nous souhaitons rendre au juge cette capacité à exercer la totalité de ses pouvoirs et à juger une situation globalement et pas seulement sur un critère qui serait. Automatique et automatiquement qui déciderait à la place du juge, si l'ordre à la justice prochainement par des algorithmes. Donc nous croyons vraiment à la justice des juges de d'autres pays et c'est pour cette raison que nous demandons la suppression de cette mesure, considérant que privé le juge de sorte d'opportunités d'appréciation au cas par cas, alors que cette décision qu'il doit prendre doit tenir compte, en particulier par exemple d'enfants qui pourraient être. Pour lesquels les deux pourrait pas. De d'augmentation du délai possible mettra encore plus d'enfants et de personnes à la rue temporairement sur des décisions automatique et sans le regard du juge donc remettant le regard du juge au coeur de la machine.

Il convient de bien voir que les situations peuvent être complexes peuvent être différentes, toutes les situations ne sont pas identiques. Il n'y a donc pas de raison d'empêcher le juge d'émettre un avis. Ça nous semble être. La position de fond qu'il convient de défendre l'empêcher d'apprécier. C'est finalement nier la diversité de ces situations et c'est la raison pour laquelle nous convergents sur l'objectif de la suppression de cet amendement. Merci. Merci l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. La commission a adopté un amendement de notre collègue Catherine Procaccia qui supprime la faculté pour le juge d'accorder des délais un squatteur. Ça nous a paru légitime. Cette mesure s'inscrit dans la ligne suivie par la Commission. Une ligne de de fermeté vis-à-vis de de des squatters. Une personne qui s'est introduite frauduleusement dans un logement ne peut selon nous pas prétendre aux mêmes garanties qu'un locataire qui subit un accident de la vie, c'est la raison pour laquelle. Nous ne revenons pas nous la commission propose bien sûr de maintenir sa position et donne un avis défavorable à ces deux amendements. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. L'amendement vise donc à réintroduire la possibilité pour le juge d'octroyer des délais renouvelables aux occupants sans droit ni titre lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour ma part, je suis favorable à cet amendement les les. Occupants sans droit ni titre font d'ores et déjà l'objet d'un traitement civils plus sévères que les locataires dont le bail a été résilié. En effet, ils ne peuvent se prévaloir, ni du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en oeuvre de l'expulsion, ni vous le savez de la trêve hivernale ainsi supprimer les délais prévus par l'article L 412 3 du code des procédures civiles d'exécution. Revient à priver les occupants de leur seule garantie qui leur est accordé pour bénéficier d'un logement décent puisque. Si on ne met pas en place cette capacité de logements décents. On on ne règle pas la la situation et on risque de se retrouver à nouveau soit avec une personne ou une famille dans l'hébergement d'urgence ou dans une situation de retrouver une situation illégale donc je. Pour ces raisons j'émets un avis favorable à cet amendement de suppression. Merci. Alors je vais mettre aux voix les amendements identiques, Merci, c'est une explication de vote parce que voilà quelques jours. Quelques semaines plus exactement je suis allée à la rencontre de 50 femmes et 17 enfants qui après une expulsion était logé abriter temporairement dans un gymnase sur décision préfectorale. Dans la ville d'Angers longtemps été maire et toutes ont raconté exactement la même histoire faite de succession d'hébergement temporaire, avec des passages à la rue et de renouvellement de nouveau l'endroit où elle trouve à se loger, parfois effectivement avec des gens mal intentionnés qui les conseillent et parfois simplement parce qu'il faut s'abriter et abrité les enfants le squat n'est pas un choix, c'est souvent la dernière option possible et je remercie Monsieur le Ministre, de l'avis favorable qu'il vient de donner car toutes ces situations chers collègues vous pouvez les rencontrer lorsque vous mesurez ce que sont la vie de ces personnes qui vont d'expulsion en expulsion. Moi je remercie la commission d'avoir intégré et à l'article 1. Et à cet article. Un de mes amendements je redis ce que j'ai déjà dit, le droit au logement se loger, c'est pour tout le monde y compris pour les personnes qui habitent et quand on habite et qu'on ne peut pas récupérer son logement parce qu'on est squattée hé bien qu'on se retrouve comme certains collègues nous non et ce qui. Expliquer pendant la dans une caravane. Ou à loger ailleurs. Le droit au logement. Il est aussi pour les locataires et les propriétaires en titre, et pas simplement pour. Les personnes qui se sont approprié un logement, quelles que soient les raisons de l'appropriation du logement. C'est à l'État, dans ces cas-là de gérer et de reloger ces personnes mais pas de priver. Ces personnes de des personnes titulaires du logement. Je voterai donc contre ces amendements. Monsieur Bena Roche. Oui Madame Procaccia monsieur le rapporteur, chers collègues. L'amendement que nous défendons ne consiste pas à dire qu'on va donner plus de temps,

A la capacité de prendre une meilleure décision qu'une décision automatique, c'est tout ce que nous disons il a tous les éléments pour pouvoir décider donc il s'agit pas d'être plus laxiste. Il s'agit d'être plus juste.

alors il s'est mis dans les conditions où il ne peut pas le faire je de l'excuse pas pour autant donc comme l'État ne peut pas le faire au final c'est les squatters qui sont dans des situations précaires, c'est-à-dire les femmes et les enfants qu'on va. Excusez-moi vous lever les bras mais je ne dis pas qu'il faut être plus laxiste, je répète encore une fois. Bis répétita plaquettes donc je le répète une nouvelle fois, je ne demande pas à ce que nous soyons plus laxiste, je demande à ce que le juge puisse juger en toute connaissance de cause. C'est tout ce que nous demandons dans sept ans, sept souvent je vous ai entendu, à juste titre face au ministre de la justice défendent le fait que le juge devait pouvoir juger du avoir les moyens de juger c'est tout ce que nous demandons dans à l'automaticité. Nous n'aurons plus de justice que par automaticité algorithmes c'est pas ce que nous souhaitons dit vous Didou. Merci madame Estrosi Sassone. Non, moi je voudrais réagir par rapport à une. Un mot d'un de nos collègues en disant que le squat n'est pas un choix. Mais le squat est illégale. Donc il est pas question de dire, c'est un choix ou c'est pas un choix. On voit, il faut arrêter d'excuser l'occupation illégale de locaux à usage d'habitation comme de locaux à usage économique et encore une fois je pense. On est tous d'accord, dans cet hémicycle pour dire qu'il y a un véritable problème dans notre pays quand au niveau de la crise du logement que du mal logement. Mais ce ne sont, ce propriétaires qui ont à supporter la charge du mal-logement. C'est l'État qui doit avoir à faire face à ces situations. Je ne vois pas pourquoi parce que l'État est défaillant ou parce que l'État par exemple n'indemnise pas les propriétaires qui n'obtiennent pas le concours de la force publique comme ils devraient les indemniser. Hé bien que ça serait aujourd'hui à ses propriétaires à supporter cette charge du mal logement. Merci. Alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques à 39 et 62 qui ont reçu un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Été. Tu es contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés je mets aux voix. Oui. Les amendements suivants le 23 et le 24 ne sont pas défendus je mets donc aux voix là l'article 1er, bé qui est pour.

Nous avons évoqué, c'était mardi. Le fait que nous sommes plusieurs à regretter que des décisions de justice ne soit pas appliquée. En l'occurrence nous parlions tout à l'heure avec nos collègues de du choix du juge. Quand le juge décide une expulsion, elle n'est pas pour autant réaliser parce que le préfet peut décider qu'il y a des conditions qu'il y a des problèmes de relogement que justement. Ça peut être une famille ou qui n'a rien d'autre à proposer aux logement et des c'est donc les propriétaires. Occupants ou non dans le désarroi. Donc cet amendement a pour but de ne plus laisser de. De temps aux préfets de ne pas avoir de ne pas organiser l'expulsion à partir du moment où il y a eu une décision de justice. C'est l'article. Le l'amendement 83. Et là l'amendement 95, j'ai été surprise de découvrir et y compris dans mon département que parfois. On faisait des propositions de relogement à des squatters qui les refusait parce que ça ne leur plaisait pas ou qu'il ne voulait pas changer de ville ou parce qu'ils voulaient de salle de bain, enfin des choses quand même assez effarante et je peux vous le dire, j'en ai entendu encore récemment dans les voeux des maires. Expliquant dans la situation dans leur commune, donc cet objectif de cet amendement a pour objectif. De dire que. On offre, si c'est possible, effectivement, une proposition de relogement aux squatters. Mais s'il la refuse, hé bien dans ces cas-là, l'expulsion est prononcé et le squatteur si la un mal-logés si les mal logés, on lui propose une solution de relogement il doit l'accepter. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors sur le 83, on peut partager le souci de notre collègue Catherine Procaccia d'accélérer les procédures d'expulsion en soumettant le recours à la force publique dans un délai strict. Il est quand même a paru à la commission que ce délai était très court 72 heures et risque de faire peser sur les préfectures une contrainte excessive alors que, on le sait, nos forces de police ou de gendarmerie doivent répondre à de multiples sollicitations. Nous pensons qu'il faut laisser un peu de souplesse aux préfets pour prêter le concours de la force publique rapidement mais en ayant la possibilité d'arbitrer entre les nombreuses nous disons même trop nombreuses demandes adressées aux forces de l'ordre à l'heure actuelle. Nous observons par ailleurs qu'aucun délai n'est fixé à l'article 38 de la loi Dalo pour prêter le concours de la force publique alors que la procédure de l'article 38 se veut beaucoup plus rapide que la voie judiciaire. Il y aurait donc, selon nous un paradoxe à prévoir un délai si court en cas de décision de justice mais pas dans le cadre de la procédure administrative de l'article 38 de la loi Dalo donc avis défavorable sur le 84. Malheureusement, chers collègues, nous avons un peu de mal à comprendre véritablement là. Portée de cet amendement puisque il nous paraît être rédigée de façon trop imprécise pour pouvoir être acceptés en tant que telle. On ne sait pas, en effet, s'il s'appliquerait en cas de recours à la procédure d'évacuation forcée prévu au 38 de la loi Dalo. Auquel cas il introduirait une nouvelle obligation de relogement qui n'existe pas dans les textes à l'heure actuelle ou s'il s'appliquerait en cas de procédure judiciaire. Auquel cas, on ne voit pas bien comment il s'articule avec les délais prévus dans le cadre d'une telle procédure donc. En en en en raison de de de de de difficultés de compréhension de de cet amendement. Je me permets de formuler une demande de retrait sinon avis défavorable.

de retrait ou défavorable pour le 84. Merci. Merci Madame Procaccia. Soit mal rédigé mais on fait de la loi et donc à la demande de. De du rapporteur je le retire en sachant que c'est quand même une préoccupation. Enfin c'est quand même absolument absolument anormal qu'un squatteur puisse se permettent de refuser et surtout après le rester dans les lieux et dans les lieux pendant très longtemps, je trouve ça un peu scandaleux. C'est dommage que la commission n'ait pas voulu réécrire mon article. Pour l'article 83. Alors je vous ai expliqué monsieur le rapporteur. Quelle est l'origine de l'article 38. L'article 38. À l'origine, il était un peu plus étendu que ça mais j'ai reçu des manifestants. il y a 16 ans dans la nuit et on a décidé de le circonscrire à l'habitation principale et en 16 ans, les choses ont beaucoup évolué. Donc vous me dites c'est pas prévu dans la loi dans l'article 38 de la loi Dalo. J'avoue qu'en. En 1987, j'étais déjà suffisamment contente de faire voter cet article. Cet article devenu 38 et comme vous me dites que le délai de 72 heures et trop court. Ce que je peux concevoir mais je me mets toujours dans la position des personnes et qui attendent pour rentrer dans leur logement je le rectifie et je modifie dans un délire le des 72 heures en mettant dans un délai de 7 jours suivant la décision du juge. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. je ne peux naturellement pas interrogé la Commission puisque la rectification vient de se faire à l'instant, moi, sur cette position là je vais faire une pause, il a un avis de sagesse le le la haute assemblée choisira. J'aurai à titre personnel souhaité qu'effectivement on fasse confiance aux préfets, qui s'est naturellement. S'il est en possibilité de mobiliser ou non la force publique. Dans ce délai-là. Ou non mais. Écoutez, avis de sagesse de ma part. Merci Monsieur le Ministre, de l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, là l'avis du gouvernement reste défavorable dans la mesure où on ne sait pas, à partir de. Qu'en cours le le délai de d'être sept jours telle qu'il avait proposé, je pense qu'il faudrait. C'est. Sur l'écriture telle qu'elle existe aujourd'hui dans le texte. Merci. Merci donc je vais oui monsieur bé proche. Oui, je voulais pas rapporteur monsieur Richard, qui demandait un avis de sagesse. Donc je vais donner le mien. En fait pourquoi. j'aurais un avis défavorable sur cet amendement. Même à sept jours parce qu'il est, il n'est pas opérationnelle dans la réalité. Alors bien sûr en fixe sept jours et on est content d'avoir fixé ça jour et peut être c'est bien d'ailleurs d'abord fixé sept jours en fait dans la réalité, vous savez très bien aujourd'hui le nombre de cas. Où il y a des impératifs qui sont fixé aux préfectures au préfet qui ne peuvent pas être respectées par exemple les convocations pour les migrants qui doivent renouveler leur carte de séjour et ça donne lieu à quoi, ça donne lieu à des milliers de recours dans des tribunaux d'appel administratif donc ça encore les tribunaux d'appel administratifs et les affaires ne peuvent pas être traitées dans la réalité. Donc je veux bien qu'on essaye de faire des amendements pour faire avancer les choses mais quand on sait par avance que de toute façon, il ne sera pas opérationnel à part d'être des marqueurs d'un certain Daubres de d'éléments. Je ne pense pas que ce soit utile en plus. La réponse de Monsieur le Ministre. Il me paraît tout à fait convaincante. Il faut savoir à partir de quand ça court quoi voilà. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement 83 rectifié sur le délai qui passe de 72 heures à sept jours. Avis de sagesse. le rapporteur. La commission ne s'est pas prononcé est défavorable du gouvernement qui est pour.

madame la présidente. Alors l'amendement 37 études suppressions d'articles en l'occurrence l'article premier. Alors par cet amendement. Nous voulons marquer au fait notre opposition global à cette proposition de loi sur le fait essentiel qu'elle criminalise ou qu'elle tente de criminaliser les mal logés. Et que parallèlement, elle ne lutte pas contre le mal logement. L'aggravation de la peine encourue pour violation de domicile que propose cet article est à la fois injuste dans son principe et disproportionnée dans ses modalités, le renforcement de la répression pénale des occupations illicites contrarie la politique du logement et la lutte contre l'habitat indigne, nous tenons à rappeler comme mon collègue Daniel Breuiller, il a fait tout à l'heure que ce n'est pas par choix que des personnes sans logement choisissent d'occuper des terrains ou des immeubles inhabités, comme l'avait très bien défendu. Monsieur le ministre de la Justice, Dupond-Moretti notamment parce qu'elle se trouve sans solution de logement. Pour rappel, la France compte 4 millions de mal-logés 2000 vendeurs de l'je vois social 300.000 personnes sans abri dans 42.000 enfants. En même temps le nombre de logements vacants bat des records. Chaque année, selon l'Insee. donc les occupants sans tenir compte de ce contexte et de cette configuration, c'est en fait faire preuve d'une certaine brutalité vis-à-vis des personnes vulnérables alors que nous deux prudent pas et l'État ne prend pas les moyens de résoudre les problèmes de, de, de mal logement qui aujourd'hui deviennent préoccupants et plus que préoccupant en France. Et donc en fait, beaucoup de gens qui s'installent dans les logements vides et essentiellement des femmes et des enfants échappent par là même à une certaine violence dans la rue et vous le savez parfaitement bien on la vie dans chacune de de nos communes, surtout dans le grade commune. L'aggravation des peines est également disproportionnée et puisqu'on va demander de payer des montants qui de toute façon de seront pas. Payés par des gens qui ne seront pas sur le vin pour payer c'est beau temps et en fait cette aggravation d'a pour effet que d'essayer d'aligner les sanctions qu'encourent les squatteurs avec ça. Le concours, les propriétaires qui se font justice eux-mêmes. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Ce sera un avis défavorable. Madame la présidente. Cette mesure pour nous aura d'abord un effet dissuasif qui nous paraît bienvenue. C'est ensuite une mesure d'équité puisqu'elle aura pour effet d'aligner la peine encourue sur celle prévue lorsqu'un propriétaires expulsent Manu militari un squatteur je rappelle enfin que le Sénat a déjà voté à 2 reprises. Mesure d'abord dans la loi ASAP puis dans lors de l'examen de la proposition de loi de Dominique Estrosi Sassone il y a à peine 2 ans. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. puisqu'effectivement. La loi ASAP prenait déjà en compte. Ce renforcement. De la répression à l'encontre des ces faits de de violation. De domicile et et je crois nécessaire. À une cohérence À une cohérence entre les peines encourues par le propriétaire et et la personne qui se rendraient coupables de ce cette violation de domicile, donc l'avis du Gouvernement est défavorable. Merci. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 37 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Et pour.

c'est c'est c'est effectivement un nouveau délit là qui est, qui est proposé par cet article. Que dont nous demandons la suppression. Le délit qui est proposé par cet article vise en fait à punir. La propagande ou la publicité. Quel que soit le mode en faveur de méthodes visant à faciliter au. À squatter à domicile. Et en fait adopter ce nouveau délit telle qu'il est présenté aujourd'hui dans cet article. Conduirait à sanctionner totalement tout le monde associatif qui prend en charge une grande partie des problèmes des mal logés et des sans-logement non pas pour les laisser définitivement dans les squats, mais pour essayer de résoudre leurs problèmes. En tout cas dans des délais plus rapide que ce que de les, les, l'État n'est n'est capable de le faire et donc on se retrouve en fait à pénaliser a condamné des gens dont le but est d'aider l'État à résoudre les problèmes des mal-logement et qui trouve des solutions intermédiaires dans des squats à un certain nombre de gens qui eau iraient dans la rue, ce qui serait encore plus coûte plus cher et bien entendu moins digne pour d'autres sociétés. Donc ces ces gens-là qu'on veut sanctionner matelas. Et le Secours catholique par exemple c'est pas des révolutionnaires. Patentés c'est tabac et qui était en fait de la résurgence d'une sorte de délit de solidarité destiné à réprimer l'aide la formation l'accompagnement qu'apporte donc ces associations et ses militants bénévoles, je le rappelle aux personnes et aux familles qui, faute de mieux, trouve refuge dans des locaux vacants. Nous ne pouvons pas donc accepter que ces associations qui tous les jours faut vivre quelque part le principe de fraternité qui est cher à d'autres républiques de viande en fait des délinquants. Nous ne cesserons de rappeler tout au long de cette loi et de projets de loi qui pourrait arriver que c'est par nécessité que des personnes viennent d'occuper des logements inhabités et nous dénonçons à la fois le fait que ces gens-là de peuvent pas être plongé aujourd'hui dans des logements décents et que la surenchère répressive contre les associations et les groupes militants qui agissent pour leur venir en aide empêche ça n'apportera aucune solution au problème du mal logement et à la capacité. va elle va elle va si vous voilà monsieur Lahellec pour l'amendement 63. Merci madame la présidente, monsieur le ministre je vais prolonger le propos. Donc si vous m'y autorisez. Nous considérons que, que cet article était effectivement disproportionnée par rapport à la liberté d'expression. Il ne faudrait quand même pas que l'on instaure ici un un délit de solidarité. Au regard en tout cas de la façon dont il est rédigé parce que nous ne pensons pas que ce sont les slogans militants en faveur de la défense du droit au logement qui mène au squat. Je me rappellerai ici qu'un chiffre hein ce sont les plus de 3 millions de logements considéré comme vacant aux yeux de la loi et même s'il est possible de procéder à des réquisitions, chacun sait ici que ça ne se fait que très très rarement donc. Nous vous demandons de considérer que ce ne sont pas les slogans ou les slogans. Par des associations de solidarité des syndicats et autres qui sont responsables des squats et par conséquent n'instaurons pas ce délit dont je parlais à l'instant. Merci, merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. La commission ne ne crois pas qu'on puisse qualifier d'acte de solidarité. La mise en ligne par exemple de véritables guides du squat qui explique. Notamment comment s'introduire frauduleusement dans un logement. Comment éviter ensuite l'expulsion en abusant des garanties prévues par la législation qui n'est pas faite pour cela. C'est ce type de comportement. Si Bénard Roche. Chers collègues du groupe CRCE qu'il convient de réprimer. Et je précise enfin. Mais ça ne nous dit pas que le Sénat a déjà adopté une dispute une disposition analogue il y a. 2 ans au moment de l'adoption de la proposition de loi de Madame Dominique Estrosi Sassone donc avis défavorable à ces deux amendements. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. La la vie du du gouvernement sera aussi défavorable. Je je crois que cette incitation. Et ses explications à violé des domiciles. c'est assez insupportable. Et pour bien connaître ce genre de sujet. Elles ne sont pas faites par les associations dont dont vous parlez. Le maire, l'ex-maire de Clichy-sous-Bois peut vous dire aujourd'hui si leur cote d'intérêt national de Clichy prend du retard. C'est parce qu'on subit régulièrement des assauts dans des appartements qu'on libère. Qui sont prévues à à la démolition et et le temps que l'on prend et un certain nombre de ces personnes qui rentrent dans nos logements suivent parfaitement. Des explications qui trouve sur internet, donc vous connaissez ma modération mais je pense que cette incitation est assez insupportable donc défavorable. Merci madame Estrosi Sassone.

au détriment de locataires de bonne foi ou de personnes de bonne foi, donc véritablement c'est quelque chose qui va plus que dans le bon sens auquel nous sommes confrontés de plus en plus souvent et je crois qu'il est important aujourd'hui de marquer notre sévérité à l'endroit de tels sites qui donne des guides d'emploi comment squatter un logement et s'attaquer ainsi à de véritables réseaux organisés. Merci. Alors je vais mettre aux voix l'amendement 38 et 63. Tous 2 ont reçu donc un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 1er Bissa qui est pour un contrat qui s'abstient oui adopté je me vois l'article 1er bis qui est pour contre. Abstention. Il est donc adopté. Passons un article additionnel à moment 42 monsieur Bena Roche. Madame la présidente, puisque la tendance est plutôt à l'aggravation des peines des sanctions et des délits. Cet amendement justement vise à aggraver une peine, la peine que nous souhaitons aggravée, c'est celle qui est prévue pour les marchands de sommeil. Qui profitent de la précarité ou de la situation irrégulière de personnes pour des, pour les loger dans les logements insalubres et elle en tout cas pas grand chose n'est prévu dans ce texte pour mieux sanctionner la soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes alors que nous savons qu'il existe près de 450.000 logements occupés considérée comme indigne et que lors dénombre 78 à faire sur des immeubles en péril ou insalubres pour l'année 2020. Venant de Marseille, je décrirai pas la situation découverte à Marseille après l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne qui a donné lieu à des dizaines et des centaines de d'expulser de de de d'arrêté de péril et où on s'est rendu compte du nombre de, de gens qui étaient logés par des marchands de sommeil sans bail ou en tout cas son bail écrit et et caetera, bon bien que la loi et et renforcer l'arsenal juridique entre ses bailleurs et qu'une ordonnance parue en janvier 2021 harmonise les procédures administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne les condamnations restent excessivement faire trop rare en tout cas nous vous proposons donc dans cet amendement d'inciter le gouvernement à se doter d'une véritable politique de lutte contre le mal logement et les marchands de sommeil. Si l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors comme l'indique. D'ailleurs. Les auteurs de l'amendement eux-mêmes. Il s'agit surtout d'un amendement d'appel. Qui vise à attirer l'attention sur l'habitat indigne. Monsieur le ministre et sur le problème posé par les marchands de sommeil. Qui exploite. On l'a dit la vulnérable la vulnérabilité des plus fragiles d'entre nous. La peine encourue. À l'heure actuelle 5 ans d'emprisonnement et déjà sévère dissuasive et pour nous il ne paraît pas absolument nécessaire de l'alourdir encore l'enjeu parce qu'il y en a un et naturellement de réprimer effectivement l'infraction sur le terrain et de déférer les auteurs devant les tribunaux. Notre avis est défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, vous savez l'attachement qui est celui du du gouvernement et et le mien de lutter contre les marchands de sommeil qui sont des Thénardier des des temps modernes et et qui profitent de la misère. Et des des plus fragiles. Vous avez raison, il faut continuer à, à lutter contre ces marchands de sommeil ce ce texte, a d'ailleurs permis d'ajouter des dispositions plus plus. Vous vous souhaitez en rendre encore plus sévère pour notre part nous nous soumettons à la sagesse. De la, de l'Assemblée pour choisir cette sévérité, merci. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 42 qui a reçu un avis défavorable de la commission. Un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est donc pas adoptée article 2 amendements 41 monsieur Bena Roche. Oui c'est un amendement de suppression de l'article de. Donc je rappelle qu'il a pour but d'éteindre le délit de violation de domicile ou résidence secondaire au résidence inhabitée. Et d'État de la procédure d'expulsion administrative en 48 heures, a tout local d'habitation. Même s'il n'est pas meublé et donc pas habiter. Et donc c'est. nous pensons. Ce qui nous concerne et c'est pour ça que nous souhaitons supprimer cet article par cet amendement. Que ce délit telle qu'il est passé aujourd'hui pour protéger la vie privée de personnes en sanctionnant l'occupation de logements meublés et régulièrement habiter va dorénavant par cet article là protégé mais on a eu un long débat. Avant-hier soir là dessus. Des propriétés la propriété immobilière en tant que. Valeur absolue de la propriété immobilière en sanctionnant, en fait, l'occupation de tout local futile inhabité feu tu le vide, fut-il vacant depuis des années. C'est une extension considérable du délit de violation de logement et qu'elle est d'autant plus choquante que nous savons que actuellement en France il y a 10 fois plus de logements vacants que de personnes à la rue. En plus de révéler donc. À nouveau. Une conception absolutiste du droit à la propriété immobilière au détriment des plus précaires. Les conséquences de ce renversement de valeurs sûres dangereuse. Cet article permet l'expulsion en bois de 24h en moins de 24h, sans procédure juridictionnelle. Et 100 contradictoire de personnes qui trouvent refuge dans des locaux totalement vide et n'ayant pas vocation à être occupé ici même avant-hier soir le garde des Sceaux a bien spécifié.

à loger des personnes y compris dans des endroits qui n'ont pas vocation à être des logements et qui ne sont pas occupés depuis des années. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Nous sommes défavorables à cet amendement de suppression de l'article. Tout simplement parce que celui-ci à notre avis contient des dispositions utiles à la fois pour préciser le sens de la notion de domicile et pour renforcer la procédure d'évacuation d'évacuation forcée des squatters qui est prévu à l'article 38 de la loi Dalo. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Même avis que monsieur le rapporteur. Un avis défavorable à la suppression. Merci alors je mets aux voix l'amendement 41 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient et donc pas adopté l'amendement 64 même président Assassi. Oui merci madame la présidente selon nous cet article de étant la notion de domicile bien au-delà du bon sens. Il crée presque un don d'ubiquité puisque toute propriété sera considéré comme le domicile d'une personne comme si elle pouvait vivre à plusieurs. Jean droit en même temps je précise en mettant tout sur le même plan les logements vacants comme les logements habités. Les petits propriétaires, comme les propriétaires de quartiers entiers vous tentez donc de masquer une réalité qui est pourtant flagrante la crise du logement fait de nombreuses, de nombreuses victimes et rien n'est fait pour résoudre ce problème. Alors nous vous le disons d'ailleurs et parce que c'est une réalité, la très grande majorité des logements squattés sont des logements qui sont. C'est-à-dire qu'ils ne sont le domicile de personne, je dis bien la grande majorité, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis la grande majorité. Vous souhaitez donc changer cette réalité en faisant rimer propriété et domicile. Mais ce n'est pas en changeant la définition des mots qu'on agit sur le réel mais bon c'est, je dirais que c'est presque devenu une habitude chez certains. Vous savez, c'est comme quand certains veulent supprimer certains encore veulent supprimer des postes dans les entreprises. Ils nous parlent peu pudiquement de de plan de sauvegarde de l'emploi plutôt que de nous parler de licenciements donc désormais il n'y aura plus de logements vacants, il n'y aura que des domiciles, nous vous proposons donc de supprimer cet article en proposant une nouvelle rédaction qui rappellera ce qu'est véritablement le domicile d'une personne, c'est-à-dire un logement habité.

affirmer clairement que le domicile pouvait englober également une résidence secondaire. Merci. L'avis du gouvernement. Oui madame la présidente, comme monsieur le rapporteur. Nous allons émettre un un avis. Défavorable puisque, vous le savez. La jurisprudence considère que le domicile correspond à. Un lieu où la personne a le droit de, de se dire chez elle et et puis au-delà des des résidences secondaires pour tout un tas de raisons, le célibat géographique ou des choses comme ça, des personnes peuvent avoir de domicile, donc un avis défavorable. Merci Madame Procaccia. Oui par rapport à ce que dit Monsieur le Ministre, les gens peuvent avoir de. Domicile. Je peux vous parler effectivement de ma fille qui vit à l'étranger qui a son appartement en France à Paris. Elle vient six mois dans l'année, mais il est considéré comme résidence secondaire et donc ce n'est pas son domicile principal puisque elle, elle n'est pas salarié en France mais à l'étranger et donc, vous lui donnez un droit au fait que ben elle revienne chez sa mère et elle n'est pas le droit de retourner chez elle. Merci madame la présidente Assassi. Franchement il faut être sérieux. J'ai j'ai pas parlé de résidences secondaires. Je j'ai non je non je n'ai pas parlé de résidences secondaires, j'ai parlé, j'ai bien parlé de logements qui sont squattés. On est d'accord sur le fait que ce n'est pas bien de de squatter mais qui sont des logements Des logements vides. Bah, ce n'est pas forcément des, des résidences secondaires, excusez-moi. Ça peut être aussi des résidences secondaires mais ce ne sont pas que des résidences. Ce qu'on aime. J'ai j'ai bien précisé qu'il n'était que ce dont je les les logements de son parc n'était le domicile de personnes, donc ce n'est pas je suppose Madame Procaccia le cas de votre fille. Dont le logement à Paris et son logement ou c'est le logement de quelqu'un c'est pas le logement de personnes. Merci madame Estrosi Sassone. pour répondre à Madame la Présidente Assassi elle dit ces logements donc sur le domicile de personnes mais ils sont bien la propriété de quelqu'un. Donc à partir du moment où cet homme la propriété de quelqu'un, on respecte le droit de propriété, ce droit qui est inviolable et sacrée et pour aller plus loin dans ce que vous dites madame Assassi. Certes, on voit bien la problématique du mal-logement mais aujourd'hui justement dans cette proposition de loi on pérennise un dispositif qui jusqu'alors était un dispositif expérimental qui permet l'occupation temporaire de locaux qui sont vides mais encadré avec des sociétés avec des associations qui justement passe une convention avec le propriétaire parce que pour l'heure, il n'y a pas encore de destination de l'immeuble par exemple de bureau où il n'y a pas, il va y avoir un changement d'usage mais ça va prendre un certain temps hé bien pendant une période de 18 mois. Partir du moment où on s'adresse à ses sociétés ou à ces associations, comme la fondation Emmaüs. Eh bien ça permet quand même d'occuper ses locaux de pouvoir loger temporairement des personnes qui sont en situation de mobilité géographique professionnelle ou des ménages en difficulté mais ça a un temps bien précis et ça hein donc c'est encadré c'est pas s'introduire dans un domicile parce qu'ils seraient vides et parce qu'ils seraient vacants. Il reste la propriété de quelqu'un. Merci madame la présidente. Mes chers collègues, je pense que les, les mots ont un sens. Et le mot domicile dans l'esprit commun il atteint 100, ce qui n'est pas assimilable au propriété il y a vraiment pour moi un danger, un danger à mettre dans une même catégorie toute une typologie de Bati. On va dire où certains. Sont occupés en permanence d'autres temporairement d'autres ne sont pas occupés depuis des années et je pense que voilà on est en train de de glisser là lorsque vous prenez des exemples en général ce sont. Des. Faits divers, où l'on voit des personnes effectivement qui ont été squatté ceux qui reviennent en permanence et des personnes qui ont été squatté dans leur domicile, qui ont été absente un peu quelque temps et qui reviennent. Il y a quelqu'un chez eux, Effectivement cela. Alerte tout un chacun et tout cela et tout totalement condamnable. Par contre, mettre dans la même catégorie ah logement hein bâti qui n'a été inoccupée pendant des années et des années qu'il est vide. Eh bien je pense que ce n'est pas ce n'est pas correct et on doit faire différentes catégories. Qui est contre. Il s'abstient n'est donc pas adopté 2 amendements identiques. Alors le 17. Madame avait. Merci madame la présidente. L'amendement proposé tend à supprimer la mention du délai de 72 heures pour que le préfet saisisse l'administration fiscale à la demande du propriétaire, dont le bien est squattée et qui ne peut pas accéder à son titre de propriété. Cette faculté est en effet déjà rendu possible par la loi de mars 2007 instituant le droit au logement opposable et pourtant et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Je vous remercie. C'est le même amendement que le que que le le 17 comme ça a été dit hein à la loi Dalo impose déjà actuellement hein. Un délai de 48 heures au préfet pour instruire les demandes d'évacuation forcée de logements squattés. Il s'agit d'un délai impératif fixé par l'article 38 de la loi et dont l'importance a été rappelé auprès des services préfectoraux, par voie de circulaire par conséquent c'est bien ce délai de 48 heures qui s'impose aujourd'hui au préfet pour l'instruction des des demandes et c'est à l'intérieur de ce même délai qu'il devra, le cas échéant, consultés, les services de la DGFIP du reste les services préfectoraux ont déjà pris l'habitude de se tourner vers les services fiscaux lorsque le demandeur éprouvent des difficultés à démontrer qu'il est le propriétaire du bien occupé si par exemple il n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de de son domicile pour récupérer. Les documents y afférents. et donc, dès lors, il ne paraît pas utile que la présente, proposition de loi rajoute ce délai supplémentaire de 72 heures, pardon pour la consultation des des services fiscaux. Donc le gouvernement a déposé et donc favorable. À ces amendements. avait de la commission. Monsieur le rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques, considère Pour pouvoir mettre en oeuvre la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 38 de la loi Dalo plusieurs conditions doivent être réunies, la personne dont le domicile a squatté doit bien entendu porté plainte elle doit faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire et enfin elle doit fournir la preuve que le logement constitue bien son domicile. Il arrive. Comme vient de le dire à l'instant monsieur le Ministre que cette preuve soit difficile à fournir en raison précisément du squat, ne pouvant accéder à son logement, celui dont le domicile est squatté aura du mal à réunir les documents établissement. Établissement son droit qui sont documents souvent dans, dans Dans ce cas, la commission propose d'inscrire dans la loi que la prof et la préfecture dispose effectivement d'un délai de 72 heures pour saisir l'administration fiscale afin d'établir les droits de la personne dont le domicile a squatté. Monsieur le Ministre, ce délai de 72 heures n'est pas redondant par rapport au délai de 48 heures, prévues à l'article 38 de la loi Dalo parce que le délai de 48 heures dont vous parlez court à partir du moment où la préfecture a reçu un dossier complet. L'éventuelle saisine de l'administration fiscale se saisit en amont se situe en amont, pardon et elle vise précisément à compléter le dossier pour qu'une demande puisse être valablement adressée aux services préfectoraux fixé un délai permettra ainsi de s'assurer que la préfecture agira avec célérité dans un domaine où une intervention rapide est nécessaire afin de mettre un terme à des situations qui peuvent être humainement très difficile j'ajouterai pour tout le monde. Merci. Alors je vais mettre aux voix donc les amendements, 17 et 86 dans 86 et celui du gouvernement, avis défavorable de la commission. Donc est pour.

Merci madame la présidente. L'amendement que nous proposons supprime la réduction du délai d'exécution de l'expulsion de 48 heures à 24h. Prévues par l'article 38 de la loi Dalo. En effet le délai d'exécution de 24h pour l'expulsion par le préfet ne serait pas opérants et ne permettrait pas matériellement à l'administration de mobiliser le minimum de moyens requis pour l'expulsion. Pour garantir l'autre public et prévenir les contentieux administratifs avec les propriétaires concernés en cas de dépassements contraints de ce nouveau délai d'exécution. Nous vous proposons de conserver le délai de 48 heures, je vous remercie. Merci. L'amendement 40 monsieur Bena Roche. Oui c'est le même argument que tout à l'heure et que celui qui vient d'être développé en fait. Quand on fait des articles ou des amendements. Il faut toujours se poser la question quand même de l'opérationnalité des choses. donc là on veut faire faire aux 24h quelque chose qui est déjà compliqué en 48 heures, résultat on augmentera le nombre de recours aux tribunaux administratifs. Dans le. Merci et l'maman. 85. Monsieur le Ministre. on s'associe à à ces amendements. C'est le même amendement pour le gouvernement. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors l'avis de la commission est défavorable. Le Sénat avait déjà voté la réduction de ce délai. Lors de l'adoption de la proposition de loi de Dominique Estrosi Sassone en janvier 2021. Et nous proposons de reprendre ce ce ce délai pourquoi parce qu'il s'agit de faire preuve de célérité lorsque quelqu'un constate que son domicile a été squatté. Si alors je mets aux voix donc ces trois amendements identiques, dont celui du gouvernement et un avis défavorable de la commission. Donc qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Je me vois l'article 2 qui est pour un qui a contre qui s'abstient. Il évoque adopté après l'article 2 amendements. 10. Alors même Gosselin. Merci madame la présidente. Cet amendement vise à. Accélérer les procédures d'expulsion. Locataires qui aurait arrêté de payer leur loyer depuis au moins 6 mois consécutif et contrer les locataires d'un meublé de tourisme qui n'aurait pas quitté le logement. Une semaine après le terme prévu de la location, c'est tout simplement parce que le nombre de loyer impayé est en augmentation, ces dernières années et que l'on parle de plusieurs millions de manque à gagner par les pour les petits propriétaires. Merci. Merci. L'avis de la commission sur un portable. C'est malheureusement un avis défavorable, chers collègues. Cet amendement entend rendre applicable. La procédure d'évacuation forcée sous l'égide du préfet prévue à l'article 38 de la loi Dalo à de nouvelles hypothèses. Le non-, paiement du loyer pendant plus de 6 mois. Et le maintien dans un meublé touristique une semaine au-delà de la date prévue. Cet amendement va à rebours de l'orientation retenue par la commission consistant à distinguer la situation des locataires défaillants de celle des squatters. La procédure de l'article 38. Ne fait pas intervenir un juge, elle est acceptable. S'agissant d'un squat. Mais pour la commission, elle n'est pas adapté à la situation d'un locataire qui doit pouvoir bénéficier d'une véritable procédure juridictionnelle. Merci. Même avis, Monsieur le Ministre. Non le. Merci madame la présidente. Le le l'avis du gouvernement, est le même que celui de de la commission qui a été parfaitement détaillé merci. Merci. Alors je mets aux voix il a retiré, merci. Alain article 2 bis. Ah ben maintenant c'est, ah ben voilà. Vous l'aurez peut-être après. 2 amendements identiques de suppression à l'article 2, le 43 Monsieur Bénard Roche. Oui je. Je comprends bien la la la vocation de cet amendement qui consiste à dire propriétaire qui peut plus rentrer dans les lieux pour l'entretenir. Parce que ces lieux sont habités par des gens qui n'ont pas il y a, tu ne peux pas entretenir ce qui paraît d'une logique absolue après la

D'abord pourquoi il a été fait cet article a été fait en réaction à une décision de la Cour de cassation. Il faut le savoir, qui a été rendu le 4 septembre, puisque la Cour de cassation confirmer la responsabilité de propriétaire d'immeuble dès lors que la. Par défaut d'entretien, même si la victime au de l'accident est un occupants sans droit et titre, bon, ça peut paraître bizarre mais c'est une décision de justice pourquoi une décision de justice parce qu'en fait avec un texte avec une loi aussi vague, l'article aussi va que celui-ci en quoi on va se trouver pris dans une sorte de Nasse, c'est si le propriétaire en fait va t'en droit de réclamer les coûts des réparations de dommages à putter aux occupants. Même après leur départ des lieux en l'absence totale d'état des lieux préalable et sans qu'il ait à prouver un lien entre l'occupation et le dommage c'est quand même grave.

Et y compris lorsque les beaux verbaux. Sont actées, comme cela est parfois le cas dans certains cas de logement précaire et donc ça risque de constituer. Une incitation au renforcement de la précarité du logement. Merci. Il avait de la commission. Monsieur le rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques, considère qu'il est anormal et même injuste qu'un propriétaire qui ne peut plus accéder à son bien et partant donc ne peut pas effectuer les travaux d'entretien nécessaires soient condamnés en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien du bien ne pas légiférer sur ce point, sur ce point reviendrait à accepter que ses propriétaires fassent l'objet d'une double peine. En outre, l'occupation illicite du logement peut entraîner des difficultés financières pour le propriétaire rendant d'autant plus difficile l'entretien de ce bien cet article, cet article 2 bis et donc bienvenue pour que l'article 12 144 du code civil qui est inchangé depuis sa création en 1804, prennent en compte le cas spécifique de l'occupation illicite de logement je précise par ailleurs que la commission a expressément exclu mais vous l'avez lu mes chers collègues exclus du bénéfice de cette exonération de responsabilité. Les propriétaires de logements indignes. Ce qui répond aux inquiétudes que vous nous avez formulé notamment en commission.

favorable à à son amélioration tels que nous les proposons dans les amendements 77 et et 87 puisqu'il faut tout à la fois protéger les propriétaires. En les déchargeant de responsabilité pour certaines. Lorsque leur logement est occupé sans droit ni titre, mais en préservant aussi. Les droits de. Pierre victime dans un certain nombre de cas d'accident et et donc les les amendements 77 et et 87 nous permet nous semble permettre répondre à vos préoccupations.

le notre rapporteur juste j'ai j'ai bien compris votre argument qui consiste à dire finalement le propriétaire s'il est condamné parce qu'il est condamné, par défaut d'entretien, en fait ça va être encore plus compliqué pour lui d'entretenir puisqu'il va être condamné à payer une amende, j'aurais aimé qu'on applique la symétrique et l'équilibre exact de ce que vous venez dire avec. Je suis d'accord avec ça mais donc le, ça veut dire aussi que le locataire qui a pas payé qui va être condamné à une amende qui va l'empêcher de payer le loyer. Ben il aurait fallu penser à ce moment-là donc on n'aurait pas dû augmenter les amendes pour les locataires. On est bien d'accord. Merci alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne sont donc pas adopté. 2 amendements identiques, le 77 Madame avec. Merci madame la présidente. L'amendement proposé précise que le propriétaire n'est pas responsable à l'égard des occupants sans droit ni titre lorsque leurs. Leur occupation a empêcher l'entretien du bien. Il répond ainsi aux inquiétudes que certains propriétaires ont pu exprimer à la suite d'une décision de la Cour de cassation en septembre 2022. Toutefois cette exonération de responsabilité ne s'appliquerait pas pour les propriétaires de logements indignes au sens de l'article 225 14 du code pénal, ce qui rejoint notamment les modifications proposées par la commission, je vous remercie. Merci le 87. Monsieur le ministre, hein. Il est défendu. Merci l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur.

Elle partage la volonté des auteurs de ces amendements d'éviter tout effet d'aubaine en faveur des marchands de sommeil, on l'a dit en commission, nous avons adopté un amendement excluant ces derniers du bénéfice de l'exonération de responsabilité telle qu'elle est prévue à cet article 2 bis de la PPL, pour le reste. La commission constate que ces amendements créerait un régime d'exonération de responsabilité, seulement à l'égard des occupants illicites alors que le problème reste le même pour le propriétaire qui ne peut accéder à son bien et ne peut donc procéder aux travaux d'entretien même vis-à-vis des tiers. S'il s'agit en effet d'un point sur lequel nous pourrions travailler travailler ensemble dans la suite de la navette. Ces amendements n'apporte pas de solutions viables aux problèmes qui les identifie. En tout état de cause, ces amendements aurait pour conséquence première de rendre illisible et plus aléatoire. Le bénéfice de l'exonération de responsabilité en s'appuyant sur la notion d'empêchement qui reposerait sur l'appréciation du juge. Il en résulterait vraisemblablement des procédures contentieuses longue qui nuirait à la lisibilité du dispositif puisqu'il ne fait guère de doute que les assurances des divers protagonistes essayeront d'invoquer ou de contester cette notion, donc je répète à vie défaveur. Monsieur le Ministre vous vous savez dit défendu. Je pense que vous avez un avis favorable sur votre merci. Donc je mets aux voix ces deux amendements identiques, dont l'un et du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Est pour.

Oui merci madame la présidente, alors j'interviens sur cet article 2 bis puisque tout à l'heure l'amendement qui a été retiré, a été l'occasion d'évoquer un problème qui aujourd'hui n'est pas résolue et je vais vous donner un exemple très précis parce que je j'ai ce dossier en tête depuis qu'on en a évoqué dans la loi ASAP, voyez, ça, ça remonte déjà il y a à la mandature précédente. Vous pouvez avoir des gens qui louent un une un appartement sur herbe. Par exemple, des gens modestes pour compléter leurs revenus pendant qu'ils sont absents. J'ai un cas où la l'appartement était loué. Donc on est bien d'accord, il y a un contrat quand ils sont revenus les Barrier des serrures avaient été changés. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on ne rentre pas plus tôt dans à la logique du squat. Ils peuvent plus rentrer chez eux. Et il y avait un contrat et donc là on se trouve devant un vide aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de protéger ces personnes qui à l'heure à laquelle je vous parle, n'ont toujours pas retrouvé leur leur Donc l'amendement il était-il évoquer notamment ce point là, donc je comprends il était peut-être mal écrit répondait peut-être pas mais moi la question que je vous pose, Monsieur le Ministre, c'est qu'est-ce que vous allez apporter comme réponse à ce cas précis, on a un contrat, on passe ensuite dans un squat. Enfin je pense que quand on plus rentrer chez soi. C'est la définition qui semble relever du mot squat. Alors je mets aux voix donc l'article de. Ce qui est pour. Contraint. Qui s'abstient et donc adopté. Article de terre amendement 67. Monsieur Lahellec. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les dispositions. Instaurées par la loi Elan est prévue à expérimental permet de loger avec des sous baux des locataires qui paient moins cher l'installation dans un logement respectant les droits, les deux le moins de normes et avec moins de droits. Pardon. Les conventions temporaires ont l'Avantage pour les propriétaires de limiter les coûts de gardiennage et à l'inverse, rentabiliser un logement qui aurait pu rester vacant. Nous considérons que ce mécanisme ne constitue pas une réponse à la crise du logement mais a l'Avantage de permettre une mise à l'abri des personnes souvent en situation de précarité, qu'il s'agisse d'étudiants ou de personnes en attente d'un logement pérenne de droit commun. Pour autant, nous dénonçons le fait qu'aucun rapport n'a permis à ce jour de tirer un bilan ni d'évaluer ce dispositif qui conserve plusieurs lacunes par cet amendement. Nous proposons d'avoir un recul plus important sur ces beaux qui désavantage les locataires avant de pérenniser donc de le dispositif. Merci. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui, mais la présidente, je répondrais volontiers à nos collègues du CRCE que je considère plutôt cet amendement comme un amendement d'appel. Parce que comme vous, je je je regrette que le gouvernement ne se soit pas acquitté de la mission de suivi et d'évaluation de l'expérimentation relatives à l'occupation temporaire que la loi Elan lui a pourtant confié expressément. Il serait cependant malvenu de refuser la pérennisation d'un dispositif qui fait largement l'unanimité. Pour cette seule raison d'absence. De de bilan et d'évaluation, les auditions que que j'ai pu mener avec Dominique Estrosi Sassone ont par ailleurs clairement permis de dresser un bilan favorable de cette. Expérimentation selon les chiffres qui nous ont été transmis plus de 1000 bâtiments 1000 bâtiments vacants ont fait l'objet d'une occupation temporaire depuis la création de ce dispositif, ce qui a permis de loger au moins 10.000 résidents temporaires. Ce qui n'est pas rien. Ces chiffres montrent que le dispositif a trouvé son public mériterait d'être davantage connu aussi bien pour lutter contre la vacance des logements que pour proposer des solutions d'hébergement temporaire, donc c'est un avis défavorable à cet amendement de suppression chers collègues mais néanmoins je pense qu'à un moment ou un autre il faudra bien faire l'évaluation et, le cas échéant réfléchir à d'autres dispositifs je vous remercie. Merci madame la présidente. Effectivement c'est c'est un avis. Défavorable. Mais sur la, la suppression de ce dispositif. Mais un avis favorable à à sa pérennisation. C'est effectivement un, un dispositif qui est utile, qui mérite d'être plus plus connue et et plus utiliser de mettre à disposition ses ses locaux vacants et de et de travailler mieux et plus en amont avec ceux qui ont les locaux vacants et les associations qui peuvent les prendre et les mettre. En en gestion et je peux vous assurer que dans le cas de tous les travaux qu'on mène sur l'hébergement d'urgence et la capacité à avoir un maximum de de locaux vacants à mettre à disposition des des plus précaires. Nous allons. Continuer à, à évaluer et probablement à pérenniser ce ce dispositif de la loi Elan merci. Oh tirer merci. L'amendement cette. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. C'est le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors ce cet amendement cette rectifier bis. À l'initiative de notre collègue. Et plusieurs. D'entre nous. Au niveau de l'article de terre qui vise à pérenniser le dispositif de mise à disposition temporaire de logements vacants. Comme indiqué il vise aussi à. Insérer sur 4 alinéa comme indiqué et dont l'objet de cet amendement et vise aussi à adapter le dispositif de protection de préservation des locaux vacants. Parle l'occupation de résident temporaire référence et fait aussi à l'article 29 de la loi. Elan puis en citant aussi l'exemple. Des des Pays-Bas qui permet aussi de sécuriser les lieux et revêtent revitaliser des quartiers dans lesquels. Ils se situent. Par ailleurs, également dans l'objet de de cet amendement. Ils prévoient également d'exclure ces locaux convoquons occupé dans le cadre du dispositif de l'article 29 de la loi élan d'un risque de requalification en baux commerciaux ou en bon professionnel qu'elle est l'objet de cet amendement. Merci. Il avait de la commission. Monsieur le rapporteur. L'extension du dispositif d'occupation temporaire de locaux vacants aux activités commerciales et professionnelles n'est pas inintéressante, si elle permet d'éviter la dégradation de ce logement ou leur occupation illicite néanmoins une telle. d'Ivoire et pardon partiellement l'esprit de ce dispositif qui est centrée depuis 2009 sur le logement, l'hébergement, l'insertion et l'accompagnement social. Selon les chiffres qui nous ont été transmis. Un tiers environ des résidences. Temporaires étaient des personnes en difficulté. En ouvrant ce dispositif aux activités commerciales des professionnels. Le risque serait alors que les propriétaires de locaux vacants favorise celle-ci au détriment d'un public plus fragile et ce serait naturellement d'hommage une telle extension nécessitera une consultation plus large, notamment au regard des règles des beaux et locaux professionnels et commerciaux que nous n'avons pas pu mener dans le petit délai qui nous était imparti. Je constate par ailleurs que l'article L 145 5 du code de commerce de commerce ouvre déjà la possibilité pour les propriétaires de conclure des baux commerciaux dérogatoires. Aussi, dénommée de courte durée qui peuvent être une solution pour occuper temporairement des locaux vacants en conséquence l'avis est défavorable. Si l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. vie du du gouvernement sera aussi défavorable. Le le dispositif visé par l'article de terre s'inscrit résolument dans le cadre de la politique. Du logement, la la loi Elan a du reste prévu une inflexion en prévoyant de manière claire sa vocation sociale sont visés explicitement. Des fins de logements d'hébergement d'insertion et d'accompagnement social. À ce titre, le dispositif est aujourd'hui conçue comme devant accueillir des résidents personne physique et pour une occupation à usage d'habitation, besoins existants en en matière d'hébergement et de Legend, il convient de préserver cette dominante au dispositif qui au regard des retours d'expérience offrent des solutions temporaires de logement ou d'hébergement qui justifie sa pérennisation. Comme j'ai dit tout à l'heure les baux commerciaux étant par ailleurs régi par une autre réglementation. Or la rédaction proposée ouvrent la porte à une forme de détournement vers des occupations. Commerciales et les précisions apportées par la norme réglementaire apparaissent aujourd'hui trop large néanmoins. Je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir à occuper bien évidemment des des pieds d'un immeuble par un local commercial y compris associatif d'ailleurs mais il me semble nécessaire de garantir que la vocation initiale du dispositif sera préservé donc tout il me mobilisé en occupation temporaire reste occupé en grande majorité par du logement et que l'utilisation commerciale soit réservé à quelques cas précis. par exemple des des pieds d'immeubles. Nous pourrions donc envisager d'y travailler, au cours de la navette à à venir s'il est démontré que cette disposition aiderait à mobiliser davantage de locaux vacants. J'aimerais par ailleurs mais je l'ai dit tout à l'heure qu'avec les associations compétentes nous mettions désormais en place un objectif de mobilisation pour dépasser les 1000 locaux. Et aujourd'hui utilisé dans cette vocation temporaire et dépasser les les 10.000 personnes accueillies depuis le début de de ce dispositif. Mais je reste à ce stade défavorable à cet amendement. Merci. Oui merci madame la présidente. Bah au vu des explications très complète à la fois tant de Monsieur le Ministre que dure rapporteur ben je retire cet amendement. Alors je mets donc aux voix l'article de terre qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Article additionnel amendements 68 à monsieur Lahellec. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est un amendement qui propose au fond que les locataires bénéficient du dispositif mentionné par là l'article de De la présente loi afin que puissent être inclus dans les protections permise par la trêve hivernale. D'autres catégories, autrement dit un élargissement de ce dispositif. Merci. L'avis de la commission je important. L'intention de cet amendement est légitime. Mais celui-ci aurait pour effet probable de décourager les propriétaires de logements vacants pour te courte période à intégrer ces logements au sein du dispositif d'occupation temporaire, ce qui apparaîtrait naturellement se disposition est par nature temporaire et donc spécifique à notre égard, il doit rester souple afin d'inciter les propriétaires concernés à conclure en plus grand nombre des contrats de résidence. Sont. Temporaires et permettre à un public soit en difficulté soit très mobiles mais. C'est pas. Comme le disait tout à l'heure Monsieur le Ministre sur un amendement précédent. Ce n'est pas interdit de réfléchir à des possibilités d'améliorer ce dispositif. d'occupation temporaire. À l'avenir et pourquoi pas pendant la navette à ce. À l'heure actuelle, à ce moment, c'est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, monsieur. Même avis que la commission, madame le président. Merci alors je mise aux voix donc la maman 68 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient donc pas adopté.

Qui s'appelle sécuriser les rapports locatifs et nous pensons. Je lisais la discussion générale l'que de sécuriser quoi que ce soit en fait ces articles et ce chapitre, les articles de ce chapitres vient de rompre l'équilibre qui a été patiemment élaborée par le législateur depuis des années toutes tendances confondues politique entre les droits des propriétaires d'une part et la protection des locataires d'autre par. De nombreuses associations de lutte contre la précarité, 12 ans. Doux Bob du Sénat sur ce sujet. quand d'autres avant que les dispositions envisagées vient de mettre en cause l'équilibre des rapports locatifs, mis en place en 1989. Patiemment améliorée depuis par tous les acteurs institutionnels privés publics ainsi que toutes les solutions proposées par les dispositifs de prévention des expulsions Penser au seul et unique profit des propriétaires et de la propriété. Le texte altère considérablement le corpus de normes visant à apporter des garanties à la partie réputée la plus faible et met en oeuvre ce que le Secours catholique appelle une industrialisation de l'expulsion locative. De son côté, la Fondation Abbé Pierre estime que ces dispositions vont provoquer jusqu'à 30.000 décisions d'expulsions supplémentaires soit autant de personnes qui risquent de se retrouver à la rue mises Boutabout ces différentes mesures permettent d'expulser un locataires en difficulté ma passagère en moins de 3 mois à partir de la constitution de la payer de loyer et supprime la possibilité pour le juge d'accorder d'office des délais supplémentaires, avec des délais aussi réduit le locataire de sera en mesure dit de payer sa dette locative ni d'obtenir des rendez-vous avec les services sociaux, ni de bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement ni d'obtenir de l'aide d'une association. En d'autres termes, le texte supprime toute possibilité pour locataire défaillant temporairement de régulariser sa situation ou de trouver une situation de relogement, ce durcissement sans égal des rapports locatifs traduit une déco d'action des situations de vie dramatique des locataires mais également des attentes des propriétaires eux-mêmes

Les auteurs de cet amendement en disant que je ne peux pas donner un avis favorable bien sûr. À cet amendement qui parce que simplement il ne tient pas compte des avancées du texte notamment ceux. Apportés par la commission. Nous nous avons, faut-il le rappeler, mais on en parlera tout à l'heure. Permis au juge de continuer à se saisir d'office des dossiers ne pas attendre que le locataire lui en fasse la demande. Nous avons ajouté deux semaines ou des les minimum entre le commandement de payer l'assignation et Nous avons considérablement renforcé l'accompagnement social. Je regarde les amendements, les articles additionnels introduit par la commission des affaires économiques. Nous avons donc vraiment. Tenter. De trouver un équilibre entre l'accélération de la procédure contentieuse. Hé hé hé. C'est la raison pour laquelle j'franchement ce serait dommage de, de, de revenir sur tout cela en modifiant. Simplement un titre. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, vous ne serait pas étonné que le gouvernement est défavorable à à ce changement de titre puisque l'essence même. De de ce texte et le travail que vous menez depuis le début, c'est bien de trouver un, un équilibre entre les rapports entre les les propriétaires. Et et les locataires proprio. Le locataire, le propriétaire et le droit de jouir paisiblement de son logement et et le locataire puissent être propre protéger en cas de difficulté, lorsqu'il est de, de bonne foi, ça sera donc un avis défavorable pour ce changement de titre. Merci alors je mets aux voix l'amendement 44 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Et pour. Qui est contre qui. Il s'abstient et pas adopté l'article 3 reste supprimer article 4. 3 amendements identiques de suppression de 46 Monsieur Bénard Roche. suppression par cet amendement de suppression. Nous souhaitons nous opposer à l'article 4 qui s'emploie à précipiter la résiliation du contrat qui lie le bailleur et le locataire en difficulté financière, dans le seul et unique objectif de pouvoir mettre ce dernier dehors le plus rapidement possible la systématisation de la clause de résiliation prévues par cet article est une mesure à la fois inutile et restrictive de liberté inutile car la majorité des baux d'habitation contiennent une clause de résiliation à droite d'ores et déjà restrictive de liberté car elle pour directement à tête à la liberté contractuelle des 2 parties prenantes au détriment du seul locataires. ça oblige aussi le propriétaire. Mais cette clause, même s'il ne le souhaite pas, telle que modifiée en commission l'article ne prive plus le juge de son pouvoir de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative et de la décence du logement. Ce dont nous nous réjouissons, monsieur le rapporteur. Toutefois, la nouvelle version de l'article n'est pas satisfaisante car elle conditionne l'octroi de délais supplémentaires à la reprise du versement du loyer et des charges à avant l'audience. Cette mesure est injuste car l'exclut de fait les locataires les plus précaires de la possibilité de disposer de délais supplémentaires alors que ce sont précisément ceux qui en ont le plus besoin. Maladie séparation, perte d'emploi. Retards de versement ou délai de versements sociaux et par ailleurs resterait de la possibilité d'octroi de des supplémentaires, on revient à méconnaître l'intérêt que représente ces délais pour le propriétaire, lui-même, vous le savez, tous les chiffres le mode de très nombreux dossiers font l'objet de règlement de la tête grâce à ces délais supplémentaires, ce qui permet aux propriétaires de retrouver les sommes dues et aux locataires de se maintenir dans les lieux, ce qui est après tout tout l'objectif recherché par les 2 parties plus généralement notre groupe dénonce la défiance à l'égard du juge exprimée par ce texte, je l'ai dit tout à l'heure une dette qui faut, d'une décision d'expulsion doit être vérifiée en toutes circonstances, par le juge en toutes circonstances resterait de la marge de manoeuvre du juge revient à restreindre l'échange les chances pardon pour qu'une solution satisfaisante et acceptable pour toutes les parties soit trouvée. Merci de 69 monsieur Lahellec. Oui madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Effectivement, le dispositif envisagé par cette proposition de loi en plus d'encombrer les tribunaux ni la capacité des locataires à pouvoir reprendre le paiement d'un loyer. Après une courte période d'arrêt. Et prévoit de fait leur expulsion systématique. Voire leur potentiel. Emprisonnement. Pardonnez-moi mais c'est un peu le retour à la prison systématique pour dettes qu'on avait connu, en d'autres temps.

Merci madame la présidente. toute la période de suspension des effets de la clause résolutoire en plus du paiement de la dette locative cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement, dans un contexte économique et social particulièrement mal choisi pour fragiliser encore davantage les personnes les plus vulnérables au delà de l'efficacité des mesures proposées. On peut s'interroger sur l'opportunité politique de ce 1er texte du quinquennat concernant le logement quand les difficultés d'accès et de maintien dans le logement persistent, voire s'aggravent. Notre ambition collective n'est-elle pas de loger tous les Français de permettre le maintien dans le logement. Faut-il le rappeler, que les personnes confrontées à des difficultés de paiement sont bien souvent des personnes qui travaillent et particulièrement encore plus aujourd'hui. Or la réduction de la précarité, l'accès au travail commence par une stabilité dans le logement. Notre groupe demande donc la suppression de cet article IV. Je vous remercie, merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. L'avis de la commission à l'égard de ces trois amendements identiques est défavorable. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les bailleurs et les locataires précise déjà que l'octroi de délais de paiement par le juge n'est possible que si le locataire et je cite en situation de régler sa dette locative. Le conditionnement de l'octroi de délais de paiement par le juge à la reprise du versement du loyer courant avant la date de l'audience va dans ce même sens et ne représente aucunement un changement de paradigme tout au plus une précision. Cela permettra en outre de démontrer la bonne volonté du locataire. Je rappellerais par ailleurs que cette condition doit déjà être réunis dans le cadre des procédures de traitement du surendettement les apports de la commission ne font qu'aligner la procédure pour impayés de loyer sur celle du surendettement. Je le répète, avis défavorable à ces trois amendements. l'article 4 pose la question du rôle du juge dans les impayés locatifs les débats en commission. Notamment sous l'égide des rapporteurs. Ont permis de préciser et de renforcer la dimension de prévention et de travail social. Je crois qu'il est encore nécessaire de compléter ses ces réflexions, par un travail sur le plan des Liens juridiques qui existe entre un propriétaire et un locataire et que le juge régie très largement aujourd'hui. que l'article 4 et il faudra donc le conserver contient des précisions positives notamment sur la clause de résiliation. Je crois aussi que des modifications importantes et pertinentes ont été introduites en commission en particulier concernant la capacité du juge à se saisir d'office. Nous avons encore un, un travail effectué. Nous allons continuer à travers d'autres amendements sur lesquels le gouvernement donnera un avis favorable mais nous sommes défavorables à un retrait total de cet article 4. Merci. Alors je vais mettre aux voix, donc ces trois amendements identiques, 46 69 79 qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne sont pas adopté l'amendement 49 monsieur Bena Roche. Alors porte sur le même article, et donc c'est un amendement de repli puisque l'article 4 et des amendements de suppression n'ont pas été voté donc cet amendement propose de supprimer la ni l'alinéa 2 de cet article. Alors c'est quoi cet alinéa de c'est celui qui systématise. J'en ai parlé tout à l'heure la clause prévoyant la résiliation de la droit d'un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Systématiser la clause de résiliation des baux d'habitation est une mesure qui, en fait je l'ai dit, porte atteinte à la liberté contractuelle sans atteindre l'objectif poursuivi par l'auteur de la proposition à savoir augmenter l'effectivité d'une clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, la majorité des baux d'habitation quand il a déjà une clause de résiliation. Ce qui rend inutile cette systématisation en fait je dirais qu'il est plutôt étonnant alors que. Nous défendons. Très souvent, les contrats. Pris par entre entre entre 2 parties. Il est étonnant de vouloir protéger en fait les bailleurs qui ne souhaite pas être réduire cette clause dans les beaux aujourd'hui de leur imposer contre leur gré. En leur ôtant donc une partie de leur liberté contractuelle le cette clause dans tous les contrats. Je comprends pas la logique. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable également les clauses résolutoire de plein droit apporte une sécurité juridique aussi bien aux bailleurs qui peut plus facilement récupérer son bien en cas de manquement du locataire à ses engagements contractuels. Colocataire qui est protégé contre les résiliation unilatérale sans motif légitime cette généralisation au sens de la commission est d'autant plus souhaitable que le secteur locatif, a déjà largement intégré cette pratique puisque actuellement, seules 1 à 2% des dossiers contentieux porte sur des beaux ne comportant pas de clause résolutoire, selon l'estimation qui nous a été fourni par l'association nationale des juges, la protection du contentieux, la limitation de la liberté contractuelle des bailleurs et des locataires seraient donc dans les faits très marginal par rapport aux pratiques actuelles. À notre sens la généralisation de ces clauses doit être. Avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. La présidente. Même avis. C'est beaucoup. Alors j'ai mis aux voix donc cet amendement 49 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. C'est pour. Qui est contraint. Ils s'abstiennent donc pas adopté 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Trois amendements identiques le IV monsieur la. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues donc. Amendement 4 rectifié bis à l'initiative de Stéphane Sautarel et plusieurs. D'entre D'entre nous. Alors concernant. Des dispositions de l'article 4 et cet article 4. Qui concerne la systématisation. Dans les contrats. De bail. De la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d'en suspendre les effets sur la. Néanmoins un risque important d'augmenter. De façon importante. Les expulsions

Et seulement 60% des locataires se rendent actuellement l'audience donc et alors il est, il est important. Cet amendement. Des fonds surtout la bonne information pour que. S'assurer que cette information soit bien transmise aux locataires intéressés sous la. Responsabilité de représentants de l'État, donc les préfets. En liaison avec les services du département où vu pour l'accompagnement social. Telle est l'objet de cet amendement. Merci le huit monsieur

Oui donc toujours un amendement de repli sur une partie de de cet article 4, en l'occurrence sur l'alinéa 3, celui qui vise. Et nous visons donc l'amendement vise à supprimer la condition relative à la reprise du versement du loyer et des charges avant la date de l'audience pour que le juge puisse accorder des délais supplémentaires. Telle que modifiée en commission l'Arctique maintenant permet au juge effectivement. D'exercer son pouvoir de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative et de la décence du logement et je dis merci à la commission et merci à notre rapporteur. Mais la nouvelle version de l'Arctique nous paraît toujours satisfaisante. En effet, à l'exclu. De fait, les locataires les plus précaires de la possibilité de bénéficier de délais supplémentaires que leur octroierait le juge alors qu'ils sont ceux qui ont le plus besoin de temps pour reprendre le versement des loyers. Le raccourcissement des différents délais opéré par cette proposition aggrave la difficulté donc pour ses locataires précaires de reprendre le versement des loyers avant la date de l'audience et diminue d'autant leur chance de pouvoir se battre lire dans le logement. Nous nous opposons donc à cette réduction des pouvoirs. Du juge par la réduction des délais. Octroyer à un certains nombres à périmètre de personnes moins large alors que le juge pourrait prendre toute la mesure de la situation et trouver lui une solution satisfaisante en exerçant son métier c'est-à-dire jugé. Merci l'amendement 25, monsieur Madame la présidente. C'est un amendement qui est déposé par notre notre collègue Emmanuel Capus. La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus peut être significativement allongé par des délais de paiement accordée par le juge dans un délai de 3 ans. Le juge ne peut accorder un tel délai locataire qu'en situation de régler sa dette locative cette faculté accordée aux juges, entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s'appliquer de facto. Il n'apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concerne pas et ne saurait le concerné. C'est pourquoi cet amendement vise à modifier l'article 24 de 1989 afin de supprimer cette faculté du juge d'accorder des délais de paiement pour des locataires en défaut de paiement. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Sur les 3 premiers amendements 4 8 et 22, ce sera une demande de retrait ou à défaut avis défavorable. Pourquoi, parce que ces amendements sont satisfaits. La commission des lois a rétabli les pouvoirs d'office du juge pour l'octroi de délais de paiement et pour la vérification des éléments constitutifs de la dette, ainsi d'ailleurs que la décence du, du logement, ce qui n'est pas rien. Il n'est donc pas nécessaire d'alourdir d'alourdir davantage la procédure en prévoyant un rôle supplémentaire d'information confiée au préfet cela risquerait d'introduire d'ailleurs hein. Un risque. De de vices de procédure si l'obligation n'étaient pas remplies et donc de rouvrir une procédure contentieuse, qui est déjà qualifiée de trop longues. L'amendement 47 lui. Rejoint ce que j'ai déjà pu dire tout à l'heure lors de la discussion des amendements de suppression de l'article IV. L'article 24 de la loi du six juillet 89 précise déjà que l'octroi de délais de paiement par le juge n'est possible que si le locataire est en situation de régler sa dette locative le conditionnement de l'octroi de délais de paiement par le juge à la reprise du versement du loyer courant avant la date de l'audience va dans ce sens ne représente aucunement un changement de paradigme. Je l'ai dit tout au plus une précision. Le donc sur celui-ci, c'est un avis défavorable sur les 47, et enfin sur le 25 rectifié bis. De monsieur kaput et de ses collègues qui va dans un sens pour le coup, totalement contraire la suppression des expulsions conditionnel qui nous est proposé porterait préjudice aussi bien aux locataires qui seraient expulsés même lorsque sa situation financière est viable. Mais. Porte préjudice également aux bailleurs qui pourrait plus difficilement voir ses créances locative rembourser le maintien des rapports locatifs, reste pour nous la solution à privilégier lorsque le locataire est de bonne foi et que sa situation financière le permet. J'ajoute d'ailleurs pour rassurer nos collègues du groupe indépendant que la commission a conditionné l'octroi de délais de paiement à la reprise du versement du loyer le courant avant la date de l'audience et que ces délais de pays m'en prendrai automatiquement fin dès le premier. Aussi bien du loyer que du plan d'apurement de la dette, le locataire locataire fortement incités à régulariser sa situation, donc avis défavorable sur l'amendement 25 rectifié vice. 4 8 et et 22 le l'avis du du gouvernement et est un avis favorable parce que nous pensons que même si c'est une condition qui n'est pas. Suffisante. La la la dimension de l'information des des locataires et est une dimension nécessaire. On sait que les publics en grande précarité et en difficulté souffrent souvent de ce déficit d'informations et, et donc la la proposition. D'accompagner mieux c'est cette information nous paraît pertinente. Toutefois, comme j'y reviendrai. Lors de la l'article suivant le le le 47 celui de. Monsieur Roche pour lequel le gouvernement émet un avis favorable. Puisque. Vous avez raison, il nous semble majeur que le juge, le juge pardon puisse se saisir lui-même en cas d'impayés locatifs sans. Demande du du locataire. Pour les mêmes raisons, puisque souvent les familles dans cette situation sont dans des situations de grande précarité, moins de 40% des locataires. Se présente avec un, un avocat. Lors de l'audience, alors que le bailleur lui vient toujours représenté. Lors, lors de l'audience et donc, nous donnons un avis même très favorable. À l'amendement 47 et évidemment pour des raisons de de parallélisme, d'une certaine manière, de l'avis du Gouvernement sur l'amendement 25 sera défavorable. Merci. Alors je vais mettre aux voix les amendements identiques, 4, 8 et 22 qui ont reçu donc un avis défavorable de la commission un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. adopté. L'amendement 52. Avis défavorable de la commission. Avis favorable du gouvernement qui est pour.

Qui s'abstient. Est adopté. Et le 25 tombe. Mais je vois l'article IV. Qui est pour.

Merci madame la la présidente. En fait une démesure qui nous apparaît. La plus. Comment dire. Une de celle contre laquelle nous opposant le plus fortement. C'est celle qui consiste à, à réduire systématiquement les différents délais de la procédure contentieuse. Du litige locatif. En fait. L'objectif bien entendu je je comprends qu'on veuille réduire les délais mais là il y a un objectif très clair, c'est. Ce expulsés. Quoi qu'il en coûte de plus rapidement possible les locataires sans leur laisser le temps de payer leurs dettes locatives. C'est ça qui doit heurte les délais qui sont remis en cause par sa tactique par cet article permettent pourtant d'éviter les expulsions, laissant le temps aux locataires. De payer leurs dettes l'Arctique est ici. Écoutez favorise en fait le phénomène du sans-abrisme sans favoriser le propriétaire, c'est-à-dire je comprendrais qu'on veuille favoriser le propriétaire et qu'on prenne des risques pour le faire mais là en l'occurrence, on prend des risques énormes et favorise pas le propriétaire dans l'intérêt de résoudre de de réside que très peu souvent dans une expulsion du locataire mais dans le recouvrement. Du montant de ses loyers. Il se fonde cet article sur le préjugé qu'il s'agit d'un choix volontaire quelque part de tous les locataires de ne pas payer des loyers alors qu'ils le peuvent. Au surplus, les nouveaux délais ne répondent à aucun besoin du côté du bailleur, jamais un délai de 3 ans n'est octroyée aujourd'hui lorsqu'un bailleur et lui-même en difficulté financière, ou si l'occupation des pas paisible ces délais importants sont rares et ne soient octroyés par le juge que lorsque propriétaire n'a aucun projet sur le bien. Par conséquent, cet article ne fait qu'affaiblir encore le droit des locataires sans répondre aux problèmes auxquels il prétend s'attaquer. Les auteurs de cet amendement des dans dans une tentative de fluidifier le marché du logement aux seuls bénéficiaires de propriétaires bailleurs et au risque de provoquer l'aggravation de la crise du du logement. L'abbé Pierre, je le rappelle, estime que cette disposition provoquera 30.000 expulsions supplémentaires soit autant de familles qui risque de se retrouver à la rue. Merci. Le 80 monsieur Bois-d'. oui ça c'est bon. Oui oui je je j'ai vu c'est j'ai du mal à m'adapter. L'article 5, réduit les délais de procédure de la procédure d'expulsion en amont de la procédure ramenant de 2 mois à six semaines, le délai entre le commandement de payer et l'assignation en justice ainsi qu'entre l'assignation et l'audience la prévention des expulsions des déploie des dispositifs de suivi et d'accompagnement pour la reprise des paiements avec des délais suffisants pour répondre à cet objectif. Cette période en amont de la procédure judiciaire et donc une étape clé pour assurer la coordination des acteurs pouvant intervenir et prévenir ainsi l'aggravation des situations la réduire dans le temps et totalement contre-productif. Il est constaté qu'une partie non négligeable et des locataires paient dans le délai de deux mois pourquoi réduire les délais et perdre ainsi des chances que la dette soit payé, ce n'est dans l'intérêt de personne. Ces mesures entrave. Par ailleurs, le travail des services sociaux, placé en première ligne et l'action des acteurs de la solidarité en leur laissant moins de temps pour réaliser le diagnostic social et financier de la famille et mobiliser les aides, trouver des solutions amiables et organiser la reprise des paiements. Les dispositions de cet article si elles étaient votées en l'état impacterait un grand nombre de ménages de bonne foi et en situation de fragilité en totale contradiction avec la politique affichée du gouvernement de maintien dans le logement et du logement d'abord. C'est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l'article 5. Merci. Merci madame la présidente. Je, je comprends que l'accélération de la procédure contentieuse locatif puisse à première vue interroger. Je reste néanmoins favorable à l'exigence de célérité de cette procédure. Il faut préciser qu'il s'agit naturellement de délai minimum légaux et non des délais effectifs constaté sur le terrain. Il est en effet anormal que ces procédures s'étale sur plus d'un an, voire deux et même parfois trois ans d'après les informations que nous ont transmises les juge des contentieux de la protection. Il est pense la Commission. Aussi bien dans l'intérêt du bailleur que dans celui du propriétaire que cette procédure gagne en clarté et en efficacité et que les jugements puisse être rendue dans des délais raisonnables permettant aux 2 parties d'agir en conséquence pour nous. L'article 5 doit être maintenu.

entre l'assignation et l'audience et ont amélioré l'accompagnement social des locataires en difficulté notamment en agissant plus en amont et en renforçant le rôle et les prérogatives des CAPEX en les sollicitant plutôt et sans allonger la procédure judiciaire. Nous avons ainsi permis aux services sociaux de disposer d'un délai total de 3 mois pour rédiger les DSF contre deux mois dans le droit en vigueur. Cela devrait donc rendre plus systématique l'élaboration de ces DSF les juges pourront alors mieux apprécier la situation sociale et matérielle du locataire défaillant, tandis que les CAPEX pour proposer des solutions d'accompagnement plus approprié pour ces raisons j'émets un avis défavorable à ces deux amendements de suppression. Merci Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Merci madame la la présidente. Le le gouvernement et émettra un avis défavorable sur la presse. La suppression pardon. De cet article, puisque cet article vise à à répondre aux craintes de de certains propriétaires qui ont pu. Être choqués par des procédures particulièrement longue, alors même que la situation des occupants ne paraissait pas juste. Ratifier ce délai néanmoins vous connaissez notre attachement à la prévention des des expulsions locatives et et très rapidement je vous je ferais un bilan du 3ème plan interministériel de lutte contre ces expulsions. Au cours du du tri du 2ème trimestre 2023. Néanmoins, nous nous soutiendrons un certain nombre d'amendements qui seront présentés. Même si comme cela vient d'être rappelé le le le à la commission a déjà fait un très gros travail. D'amélioration et d'équilibrage de. De ce texte. Notamment pour les les la situation d'impayé de locataires de bonne foi. Et qui doivent être accompagnés. Donc moi je vous propose de retirer. Cet amendement sinon j'émettrai un avis défavorable au titre du gouvernement et nous continuerons à travailler dans les minutes qui viennent sur son amélioration, merci. Merci alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques, 51 80, qui ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues par cet amendement. Nous dénonçons le fait que plusieurs dispositions de cet article des grandes la possibilité de remboursement. Pour le locataire dont les mensualités établi dans un plan d'apurement seront multipliés par trois puisque les délais possibles pour le juge serait réduit de 3 ans à un an. De plus, nous considérons que le fait de systématiser les expulsions sans tenir compte des situations départementales et locales notamment de saturation de l'hébergement d'urgence et de la tension autour du logement ni du niveau des loyers comme le souhait de l'imposer la l'alinéa 16 est une grave atteinte à la protection des locataires. Par cet amendement. Donc nous proposons que l'article 5 concerne uniquement des ajustements rédactionnels et améliore la visibilité sur la situation socio-économique des locataires en situation d'impayés de loyers. Merci. Merci. Le 76 n'est pas défendu quatre amendements identiques. Le 18 monsieur lévrier. Merci madame la présidente. L'amendement identique à nombres de nos collègues rétabli le délai initial de deux mois entre le commandement de payer et l'assignation en justice au lieu des 6 semaines proposée par la Commission. Ce délai permettra d'éviter le recours à la procédure judiciaire en locataires permettant au locataire de rembourser sa dette locative dans le délai prévu et bien évidemment de se saisir de dispositifs publics d'apurement de la dette. Je vous remercie.

rehausser le délai par rapport au texte qui nous venait de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que. L'idée de cet amendement, c'est de revenir au délai initial de deux mois. Pourquoi. Tout simplement parce que on sait que dans ce délai de 2 mois même si on sent bien la volonté de raccourcir au maximum effectivement s'temps intermédiaire. Il permet quand même à deux tiers des problèmes d'un plaid d'impayés d'être résolue à l'amiable et la crainte qu'il y a derrière tout ça, c'est que quelque chose qui peut se régler à l'amiable dans ce temps qui est quand même pas quand on parle de 3 ans de procédure globale de moi c'est peu et dans ces deux mois si pour raccourcir de semaines fin de de semaine ou quatre semaines. On prend le risque de judiciariser des situations qui pourraient se régler, c'est quand même un peu dommage 2 tiers des situations se règlent à l'amiable dans ce délai. Merci le 53 monsieur Bena Roche. Écoutez c'est une parfaite des faces par Madame Létard en fait. La commission des affaires économiques a travaillé là-dessus, je le comprends bien, je pense que la commission des lois aurait dû arriver au même résultat. En fait, on est sûr de moi, ce qui est pas un délai excessif, on vient de le montrer. Pour résoudre 2 tiers des affaires et on passe à 6 semaines, j'ai envie de dire pourquoi six semaines passent 5 semaines et demie pas cette semaine. Pourquoi changer en fait je veux dire très clairement. Bien sûr vous. La commission des lois, augmenter le, le délai est vraisemblable qui avait été mis dans le texte par l'Assemblée nationale mais 2 mois ça résout 2 tiers des problèmes. Qui et sur quelles études. Peut-on se baser pour dire on va réduire le délai, ça va être mieux alors qu'on sait que ça va être pire. Merci le 88. Monsieur le Ministre. Si vous avez quelque chose à ajouter. On est sur une mensualisation des paiements des des loyers et donc il paraît parfaitement logique de rester sur des mois complets pour reprendre. La situation et et et la reprise des des paiements ou en tout cas le travail social nécessaire, on est pour beaucoup d'entre nous tous des des élus locaux. Nous avons des centres communaux d'action sociale et nous savons aussi les difficultés qu'ont les assistantes sociales départementales pour mettre en oeuvre des des procédures et il faut au moins c'est deux mois et donc le l'avis du enfin la vie l'amendement du gouvernement et est totalement parallèle et en phase avec ce ceux qui ont été présentés de le passage de 6 à 8 semaines. Merci le 80 hein. Voilà. Cet amendement de repli est proposé par le l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales particulièrement préoccupé par cette proposition de loi et notamment son chapitre de pour les conséquences qu'elle entraîne pour le logement des familles rencontrant des difficultés économiques les délais en amont de la procédure judiciaire doivent rester un temps utile d'accompagnement social avec le diagnostic social et financier de la situation du locataire réalisé par les services sociaux du département, face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l'accompagnement social ne doit pas être sacrifiée au nom de la nécessaire réduction des délais dans la procédure contentieuse du litige locatif, l'écart de deux semaines entre le délai actuel et le délai prévu par la proposition de loi n'est pas de nature à léser les droits du bailleur mais doit être un temps utile pour l'accompagnement social du locataire. La réduction du délai de paiement de la dette locative n'est pas compatible avec des délais concrets d'intervention des acteurs de la prévention. Comment en effet dans des délais aussi contraints pourra-t-on continuer de réaliser le diagnostic mobiliser les acteurs, mettre en place un accompagnement social et au besoin envisager un relogement cet, cet amendement propose ainsi de conserver le délai de deux mois après un commandement de payer. Merci. Alors 4 amendements identiques, le cinq Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans le même esprit hein. À l'initiative de notre collègue sauterelles plusieurs. D'entre nous. Je ne rappellerai pas l'objet mais en insistant aussi sur. Sur les tensions du marché locatif et des difficultés à trouver une solution de relogement pour les locataires qui rencontrent des difficultés financières, il y a le volet humain qui est très important et l'accompagnement social qui ne doit pas être sacrifiée. Au nom de la nécessaire réduction de délais de la procédure contentieuse du litige locatif, telle est l'objet de cet amendement.

Madame la présidente. C'est un amendement qui est déposé par notre collègue Emmanuel Capus visant à réduire le délai de six semaines à un mois. Partant du fait. Qu'un délai en semaine introduirait une confusion dans les procédures.

Merci. Il vise à supprimer la disposition qui prive la personne susceptible d'être expulsé de délai de deux mois suivant le commandement à payer lorsque le juge constate que celle-ci serait de mauvaise foi. On perçoit l'intention du législateur qui consiste à distinguer les personnes en situation de détresse sociale et dans l'incapacité de payer des autres locataires et effectivement. Le on le perçoit. On la comprend. Par contre ce qui nous inquiète, c'est toujours dans l'écriture. Encore une fois là et dans ce que ça peut laisser. Prospérer comme. C'est le caractère flou de l'expression locataire de mauvaise foi. Il y a. Qu'est-ce qui est locataire de mauvaise foi, s'il n'est pas défini le Secours catholique la digue bien d'ailleurs le caractère imprécis de cette expression comporte un risque d'arbitraire et comporte juge comporte un risque qui serait lié au fait que d'abord le juge pourrait être insuffisamment informés de la situation de la personne. Et que rien n'interdit dans l'expression de mauvaise foi au juge de considérer que des personnes qui subissent une situation de grande précarité serait nécessairement de bonne foi. C'est donc pour éviter de crue d'insécurité. Juridique. Que nous souhaitons en fait supprimer cette disposition de l'article 5. En ce qui concerne l'abonnement. 48. Il remplace là idée 37 par un certain nombre d'autres à l'. Et en fait l'objet et de demander de suspendre l'expulsion des personnes reconnues prioritaires Dalo et devant être logé en d'urgence. Bien entendu la reconnaissance d'Allos d'annule pas le jugement d'expulsion mais elle fait obligation de relogement et la menace d'expulsion et souvent trop tardivement considéré comme effectif ce qui ferait que les recours Dalo sont pris au code après intervention de la force publique familles et propriétaire d'Allos et prioritaire Dalo à la rue sans proposition de relogement. Alors qu'une proposition de relogement est prévu. Et la procédure donc telle qu'encadrée par la loi doit aboutir à un logement ou un relogement des reconnus prioritaires Dalo la responsabilité de l'État de concourir aux expulsions au nom du droit de propriété doit être concilié avec l'obligation de l'État résultant du droit au logement et de peut décemment pas aboutir à mettre des personnes et des familles à la rue. Nous proposons donc d'accorder sursis sur expulsions des prioritaires Dalo tant qu'une solution de relogement n'a pas été trouvé. Et, dernier des 3 amendements. C'est le 45 rectifié et le 45 rectifié a pour objet de demander à ce qu'aucune expulsion des locaux entre que des domiciles ne soient effectué lors de la trêve hivernale. Selon l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels en 2021 64 % des 1330 expulsions ont eu lieu en trêve hivernale, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. Le rappel ce n'est pas par choix eux par nécessité que les personnes sans logement choisissent d'occuper des terrains ou des immeubles inhabités alors par le biais de logements inoccupés à des terrains ou immeubles inhabités. Le constat du phénomène du mal-logement et du sans-abrisme est sans appel de ce, de 623 personnes sont mortes dans la rue. En 2021, 30.000 personnes sont sans domicile fixe 1700 forts le 115 refuse chaque jour chaque soir un hébergement à plus de 6000 personnes dans 1700 enfants et ça touche des familles des retraités. Bon je veux pas citer d'exemple face à l'incapacité de l'État de proposer des solutions de relogement, y compris de logements d'urgence à des familles précaires nous demande Docks à minima de ne plus effectuer d'expulsion pendant la trêve hivernale j'ai dit bien autre que celle des domiciles de de de monsieur Bénard. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Sur l'amendement 70. Cet amendement revient sur les réductions de délais de la procédure contentieuse locative et sur les critères de qualification du squat. Pour toutes les raisons que nous avons déjà évoqué en discussion générale et lors des amendements précédents il est contraire à la position exprimée par la commission j'émettrai donc un avis défavorable. Sur les amendements suivants, c'est-à-dire les. Le 76 étant tombée sur le 18 rectifier bis le 28 rectifié le 53 et le 88 rectifier 4 amendements identiques. Le constat de lenteur de la procédure pré-contentieuses et contentieuses en cas d'impayés locatifs a été reconnus ou à défaut non. Par l'ensemble des personnes que avec. La rapporteur de la commission des affaires économiques. J'ai interrogé cette procédure. On le sait peu s'étaler jusqu'à 3 ans, selon les juges des contentieux de la protection qui sont a priori les interlocuteurs objectif sur ce sujet. Cette procédure doit donc être accéléré, ce qui est l'objet de l'article 5 de ce texte. Néanmoins les auditions que nous avons menées ont démontré que le délai contentieux entre la délivrance du commandement de payer et l'assignation en justice était utile puisqu'il permettait de résoudre les 2 tiers des difficultés. lors de l'examen en commission des lois, nous aurons fixé ce délai à six semaines contre un mois dans le texte de l'Assemblée nationale et de moi dans le droit en vigueur ce délai et je voudrais vraiment insister là-dessus. Ce délai est compatible avec le délai de 5 semaines que l'Agence nationale pour l'information sur le logement estime elles-mêmes nécessaires pour initier l'accompagnement social, les locataires. Cette solution ne semble un bon compromis entre le souci de célérité de la procédure d'expulsion en cas d'impayés et le souhait de maintenir les rapports locatifs lorsque le locataire est encore en mesure bien sûr de s'acquitter de son loyer. Elle a en outre le mérite d'apporter de la cohérence avec le délai de six semaines, délai identique que le texte prévoit déjà entre l'assignation et l'audience pour toutes ces raisons j'émettrai un avis défavorable à ces quatre amendements.

et et. Dominique Estrosi Sassone. Rapporteur de la commission des affaires écho. Nous avons essayé de trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la procédure contentieuse, qui est naturellement trop trop longue puisqu'elle peut attendre trois ans et une meilleure prise en charge des locataires en difficulté par les services sociaux et les excès, c'est pourquoi. Lors de l'examen en commission, nous avons renforcé le rôle et les prérogatives des CAPEX. Nous avons également rendu plus précoce et centré l'accompagnement social sur les locataires qui rencontrent le plus de difficultés. En parallèle, nous nous laissons plus de temps aux services sociaux pour réaliser le diagnostic social et financier et ainsi identifier les difficultés des locataires. Je l'ai dit tout à l'heure, ils disposeront de 3 mois contre 2 mois actuellement. Et pour en l'initié dès le commandement de pays. Dans ces conditions, nous avons considéré que la réduction du délai entre l'assignation et l'audience et non seulement acceptable mais souhaitable pour éviter que les procédures ne s'allonge au détriment des bailleurs comme des locataires défaillants qui resteraient soumis à une procédure contentieuse longue qu'il les maintiendrait dans l'incertitude quant à leurs perspectives d'hébergement. J'ajoute enfin que le délai de six semaines entre l'assignation et l'audience est cohérent avec le délai de six semaines entre la remise du commandement de payer et l'assignation en justice pour répondre à l'amendement de nos collègues du groupe indépendant qui souhaite réduire ce délai à un mois ce délai de six semaines nous semble le bon l'Anil donc l'Agence nationale d'information sur le logement dont vient de parler, nous ayant indiqué qu'un délai minimal de 5 semaines étant nécessaire pour pour engager les procédures d'accompagnement social des locataires. C'est donc un avis défavorable sur ces amendements de la part de la commission. S'il vous plaît monsieur le rapporteur. Vous étiez partis sur l'amendement 80. Et là vous nous citez vos amendements donc je ne sais pas 80 vous êtes défavorable.

Hé 48 j'en suis au 48 avis défavorable également. Et 45 rectifié avis défavorable également, j'en suis au bout oui. Merci monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Si madame la présidente. Je vais essayer d'être aussi clair que monsieur le rapporteur. Donc sur le l'amendement 70. le gouvernement émet un avis défavorable. Sur les amendements 18 rectifier 28 53 et celui du gouvernement évidemment favorable, je l'ai déjà expliqué. Sur celui le 80 hein. Qui permet effectivement de débuter le le diagnostic diagnostic social et financier avant l'audience et donnera désormais un délai de 3 mois pour élaborer le donc on on salue ces avancées et on estime qu'il y a pas de raison de le modifier. L'avis est défavorable. Sur le cinq rectifier 9 rectifier 14 rectifier 21 rectifié comme. Même avis que que la commission et donc un avis défavorable. Sur le 26. La réduction cette fois-ci du DSF un avis défavorable. Le 56, comme la commission un avis défavorable. Le 48 là aussi comme la commission un avis défavorable et enfin le 45 comme la commission un avis défavorable. Merci madame le président. Je vois que le gouvernement. A au moins essayer de d'avancer un petit peu sur ces délais de mois plutôt que les. Six semaines. Je voudrais dire à nos collègues du groupe républicain. il peut toujours dire qu'en moyenne, ces cinq semaines. Mais il y a des départements. Où pour obtenir le moindre accord du FSL. Qui est quand même souvent nécessaires. Pour voir comment on peut apurer la dette. Et ben c'est la croix et la bannière. Parce qu'il y a embouteillage des services. Donc se donner quelques semaines auront c'est moi j'ai pas l'expérience que c'est souvent au dernier moment dans la dernière quinzaine que se joue la possibilité de régler au mois d'avancer vers le règlement. Donc honnêtement sur l'ensemble de la procédure. Ça fait pas énormément de de rallonge parce que comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est pas les quelques semaines comparé au à ce que vous donnez comme exemples de trois ans de litige. D'ailleurs faudrait quand même se. S'interroger. Sur les raisons de ces trois en litige. Pourquoi aujourd'hui on met trois ans. C'est c'est pas parce que le local, le propriétaire ou locataire sont de mauvaise foi. C'est que la justice elle-même se donne pas les moyens de régler les problèmes. Et alors comme c'est, on veut accélérer. Au lieu de faire fonctionner correctement la justice. Ont fait augmenter la pression sur les gens qui sont engagés. D'un côté ou de l'autre de la procédure. On devient fou. Par la loi, on essaie de régler des choses et je je vous fiche mon billet qu'il y aura encore des procédures longues, bon donc il suffit de reporter l'audience d'une énième et etc. Il faut quand même s'interroger et ça nous ramène à la question pourquoi encombre nous les tribunaux.

Oui je, je ne vais revenir que sur ces quatre amendements identiques. Patriat l'État ben arrange gouvernement en fait j'ai j'ai bien compris, dans la réponse argumentée de notre rapporteur que cela a été fait en, en raison d'une moyenne et pour rendre cohérent. Bon, en l'occurrence permettez-moi je rapporteur de vous dire que c'est arguments que je conçois volontiers, mais ce qui me semble plus important c'est l'efficience la réalité le le l'efficacité en fait voilà et donc ça me ça vraiment très dangereux de passer d'un délai de deux mois qui fonctionne dans 2 tiers des cas. cas. Délai réduit à 6 semaines d'autant. Tout laisse à penser que ça ne permettra pas de faire mieux dans la résolution puisqu'il a beau temps mais que ça risque de déséquilibrer et de faire moins bien et donc, comme l'a dit très bien, Marie-Noëlle Lienemann

Alors je vais mettre aux voix donc. Qui a monsieur le rapporteur. Oui bien sûr. Oui comme j'étais. Je voudrais vraiment rappeler que le le but de la commission était de trouver un juste équilibre entre le souci de rapidité dont on a parlé.

Mais en fait, dès lors que. Désormais, les CAPEX. Pourront être. Saisis plutôt que le DSF pourrait être saisie dès le départ, dès le lendemain du commandement de payer, c'est bien. Une augmentation du délai permet aux services sociaux pour réaliser le DSF qui in fine et et proposé donc au lieu des au lieu des deux mois disponible jusqu'à présent aux services sociaux pour faire ce DSF c'est désormais 3 mois 6 semaines plus 6 semaines de telle façon à ce que lorsque le l'audience. Sera sera. Tenu le juge puisse vraiment disposé non pas seulement dans 30% des cas, comme c'est le cas à l'heure actuelle mais. je ne peux pas naturellement dire ce qu'il en sera l'avenir, mais d'un plus grand nombre de DSF, voire de la totalité des DSF puisque les services sociaux ont eu trois mois au lieu de deux pour élaborer ces ISF j'essaie de vous faire comprendre ça donc in fine J'ai le sentiment qu'on est on est parvenu à un bon équilibre quand même on réduit certes le délai mais in fine et les services sociaux. En plus de temps pour faire les, l'ISF. Merci, merci. Alors je mets aux voix l'amendement 70. Qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. S'abstient pas adopté, je mets aux voix donc quatre amendements identiques, 18 28 53 88, dont celui du gouvernement et qui ont reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ne sont pas adoptés. Le 81 voilà. Avis défavorable de comme ceux du gouvernement qui est pour. Qui est contrat qui s'abstient ne pas adopté. 3 amendements identiques, 5 9 21. Monsieur la

Qui est contre. Qui s'abstient. Pas adopté. Le 26. Avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Adopté le 56 défavorable commission gouvernement qui est pour. Qui est contraint. Qui s'abstient pas adopté. Le 48, même avis même vote. Le 45, même avis même vote. Merci le 29. Madame la présidente. L'État. Pour une meilleure réactivité et permettre de rentrer en contact avec la personne concernée par un autre moyen que l'envoi d'un courrier il apparaît pertinent de communiquer les coordonnées téléphoniques et adresses mails. C'est pourquoi le présent amendement propose dans le respect des personnes concernées que cette transmission de coordonner soit indiqué dès la rédaction du bail écrit qui permet à la personne d'être au fait de la communication de sa situation dès lors qu'elle rencontrerait un problème de paiement cette transparence peut faciliter l'entrée en relation des intervenants sociaux et juridiques avec le locataire et ainsi favoriser la relation d'aide cette rédaction permet ainsi de préciser le contenu de la transmission sous et qui figurait d'ailleurs dans l'objet de l'amendement madame Estrosi qui vient être précisée. Cette précision a paru utile à la commission, elle rejoint les recommandations du rapport des moulins, publié en 2020 et qui constatait qu'il était difficile de joindre les locataires pour les informer de leurs droits et leur proposer un accompagnement social. La vie est favorable. Si l'avis du ministre. Même avis favorable que la commission. Si donc je mets aux voix l'amendement 29, il a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement. Et pour qui est contraint donc adopté l'amendement 93 monsieur le rapporteur. un amendement. Logistique, pardon. Simple simple correction. Le gouvernement favorable. Merci. Je me vois donc l'amendement 93. De la Commission, avis favorable du gouvernement qui pour qui est contre qui s'abstient donc adopté. Je me vois l'article 5. Pour un contraint. Qui s'abstient n'donc adopté. Après l'article 5 2 amendements identiques, le 50 Monsieur Bénard Roche. Oui merci madame la présidente. Cet amendement fait. Demande la suspension des effets du commandement de quitter les lieux. Lorsque le ménage ou la personne. Qui fait l'objet d'un jugement d'expulsion saisi la commission de médiation départementales. C'est les prioritaires Dalo en fait qui sont concernés par des commandements de quitter les lieux et qui peuvent faire recours à la commission de médiation départementales d'ailleurs en 2018, il y en a eu. 55.000. Je crois qu'il a été déposé devant le huit commissions de médiation les comètes. Et le nombre de recours a tendance à attends en augmentation. Ça a un effet puisque cette commissions de médiation départementales. En fait, contribue assez. De manière assez considérable, assez conséquente à lutter contre la précarité locative et donc nous pensons que suspende cette procédure d'expulsion. Donnerait de meilleures chances à une mise en oeuvre effective du Dalo. C'est une proposition, il faut le dire, qu'est issu de l'association Droit au logement.

Même amendement puisque nous proposons de suspendre les commandements à quitter les lieux tant qu'une reconnaissance de priorité droits logement n'est pas établie. Donc c'est. La même chose que l'amendement qui a été fort bien défendu par notre collègue merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Un avis défavorable, l'accompagnement social des locataires en difficulté ne doit pas commencer à l'issue de la décision judiciaire, mais dès les premiers impayés. C'est le sens des amendements que nous avons porté Dominique Estrosi Sassone et moi-même lors de l'examen du texte en commission en l'état. Mes chers collègues, vos amendements risquerait non seulement de ralentir une procédure d'expulsion locative déjà très longue qui peut s'étaler, on l'a dit. Jusqu'à trois ans mais pourrait en outre engorger les commissions de médiation par les effet signale qu'ils engendraient. La fumée. Si l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Bien évidemment les l'État est tenu de prêter ce concours l'exécution d'une décision. De justice et donc pour ces raisons le où cette raison le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Merci. Merci alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques, 58 72, qui ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui. Pour. Qui. Vous vouliez prendre la parole.

avec plaisir. Merci Valérie. La présidente. Le présent amendement donc les 55 a pour objet d'interdire toute expulsion locative lorsque des personnes mineures sont présentes dans le logement et que la famille n'a pas obtenu de propositions de relogement, c'est-à-dire il faut que les 2 conditions soient remplies qu'il y ait des mineurs et qu'il y ait aucune proposition de relogement. Cette mesure a pour objet de lutter contre les expulsions, locataire de familles. Avec des enfants. Bon je vais pas rappeler tout le chiffre 4 millions de personnes mal logées, 600.000 enfants, selon le rapport 2021 sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, j'ai pas entendu les chiffres du du rapport 2022 qui était remis hier ou avant-. Hier j'étais ici, donc j'ai pas pu y aller mais enfin on doit les avoir aussi je pense pas que ça ait baissé. Autant d'enfants qui vivent dans la rue ou qui sont hébergés chez des tiers, ou qui sont à l'hôtel ou qui sont dans des squats ou qui sont dans des structures d'hébergement collectives en tout cas qui sont dans des situations où. Leur leur intégrité physique et morale et forcément attaqué beaucoup plus facilement. La FCPE, le collectif des associations unies et le collectif jamais sans toi ont alerté sur le fait que plus de 4 à 6% d'enfants scolarisés enfin que le nombre d'enfants scolarisés qui dorment dans la rue, a augmenté de 4. Pour ça, je dis bien 4 assis pour ça depuis le début de l'année 2022 par rapport à 2021. certaines Fabien arrête de payer le loyer pour protester contre les conditions insalubres dans lesquelles elles vivent. On a vu beaucoup de cas médiatisés là aussi à la télé comme les cas de squat d'ailleurs il y en a autant. De moisissures qui empêche les enfants de respirer de Balco qui risque de s'effondrer de trou dans le plafond et cetera. Donc pour ces raisons-là doux souhaitant que on ne puisse pas. Avoir recours à une expulsion locative lorsqu'il y a des mineurs et que la famille n'a pas obtenu de propositions de relogement. Le 52. Porte sur un autre. Un autre souci enfin dans le cas qui nous cause problème. C'est. Le fait qu'on puisse en fait. Faire jouer un effet de clause de résiliation de. La droit du contrat de location. Alors que le bailleur de respectent pas l'encadrement des loyers dans les zones tendues, c'est-à-dire qu'en fait on a un. Dispositif une disposition dans dans l'article 140 de la loi et Elan qui permet d'encadrer les loyers, vous le connaissez dans certaines zones dit de flux tendu. Dans ces villes les loyers étant normalement encadrés. Un certain nombre de bailleurs de respectent pas cet encadrement et sont en infraction. Il détermine des loyers qui sont trop élevés par rapport à la règle. Et donc ce que nous disons nous. Comment peut-on. Permettent à un bailleur qui lui même état d'infractions. Et qui demande donc un loyer qui ne devrait pas demander en fonction de la loi de résilier le contrat de location parce que le locataire de lui pas soigner ça nous paraît du de contradiction totale. Donc nous demandons donc que lorsque le propriétaire ne respecte pas ces clauses d'encadrement de loyer, il ne puisse pas faire jouer cette clause et donc de résolution du bail et expulsé demandé l'expulsion sur le locataire. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. en affirmant qu'ici nous le partageons tous néanmoins je ne pourrais pas donné un avis favorable à cet amendement telle qu'il est proposé en 1er lieu, il convient de rappeler que les demandes de concours de la force publique ne sont pas une compétence liée du préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pendant lequel il s'informe auprès des services sociaux et des services de police, de la situation économique et sociale et, bien entendu. Notamment de la composition du foyer des personnes à expulser. Aucun texte ne limite son pouvoir d'appréciation, tout au plus a-t-il précisé à l'article L 153 tirer 1 du code des procédures civiles exécution que le bailleur a droit à une indemnité si le préfet lui refuse l'octroi du concours à la force publique. Il n'est ainsi pas rare que les demandes de concours de la force publique soit refusé d'après les chiffres de la Cour des comptes en 2019, les préfets ont instruit 52.860 demande le concours de la force publique, parmi lesquels 35.208 ont été accordés. Les 17.652 demande restant ayant été refusé explicitement ou implicitement supprimer le pouvoir d'appréciation du préfet qui prend déjà en compte les conséquences sociales qu'aurait une expulsion avec le concours de la force publique permettrait à des parents de mauvaise foi, il en existe peut être de se maintenir de façon indéfinie sans droit ni titre dans un logement sans qu'aucune solution d'expulsion ne soit possible en outre l'amendement mentionne le relogement des familles, alors qu'il pourrait s'agir de groupes d'opposants illicite mêlant des adultes et des mineurs sans qu'un lien familial ne les lie véritablement dans ce cas est telle qu'il est rédigé cet amendement ce groupe pourrait se maintenir indéfiniment dans le logement, malgré la décision judiciaire d'expulsion. Je rappellerai enfin que le juge peut par ailleurs déjà accorder des délais différents des délais différents l'expulsion en prenant en compte la situation de famille tel que c'est prévu dans le code des procédures civiles d'exécution donc avis défavorable sur le 55 sur le 52, avis défavorable et également parce que la mesure que vous nous proposez, cher collègue. Paraît disproportionné mais aussi favorable à une explosion des contentieux. Par ailleurs et comme nous avons déjà pu en discuter, lors de la discussion de l'article quatre tout à l'heure en cas de contentieux locatif, le juge peut d'ores et déjà vérifier d'office les éléments constitutifs de la lettre de la dette locative et notamment aussi le caractère descend du logement. Donc là aussi, avis défavorable. Merci madame la présidente pour l'amendement 55. La vie du, du gouvernement et est défavorable pour les mêmes raisons que celles de la commission, et tenu de prêter son concours à l'exécution d'une décision de justice. Néanmoins nous avons comme la commission confiance d'abord dans la saga cités du juge puis celle de du préfet de de de faire l'évaluation sociale telle qu'il telle qu'elle est prévu mais donc l'avis est défavorable pour le pour le 52 dans la mesure où nous cessons de le dire, cette loi est est équilibré entre le droit des, des locataires et et le droit des des des propriétaires. Eh bien le gouvernement émet un avis favorable. Si effectivement le propriétaire ne respectent pas. Les réglementations de la ville dans lequel elle s'applique et donc l'encadrement du du du loyer il se met en faute. Et et donc nous trouvons cet amendement intéressant et nous émettons un avis favorable. Je ne céderai pas davantage sur le 2ème amendement puisque le gouvernement donne un avis favorable. J'espère que nos collègues du groupe républicain pourrait quand même comprendre l'importance de l'égalité, puisqu'on est dans un jugement équitable. Mais quand on dit il faut laisser le préfet. Choisir décider. Le problème du préfet, c'est le crédit. Ce que j'ai été ministre. Des préfets m'ont dit je ne peux plus. Car je n'ai plus les crédits inscrits. Pour payer le loyer. En m'opposant à la force publique. Qu'à la limite du choix du préfacé ça c'est son budget. Or il s'agit d'enfants. Quel avenir faisons-nous à notre République. Si les enfants déjà 25% des enfants. Vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Si en plus une partie de. Comme image de la République. L'expulsion même si leurs parents sont pas des des des saints. Quelle image ils ont de la protection républicaine sans relogement et là il s'agit pas d'exiger le relogement mais une proposition de relogement. Si les parents sont de mauvaise foi, il y a eu proposition de relogement. Je vous assure, on est en train de de de de se donner des des effets sociaux et politiques avec des boomerangs terrible. La contestation des principes mêmes de notre République. Vont être accrue dans une partie de la jeunesse la plus paupérisées. Or on a besoin de leur adhésion. Franchement c'est pas dramatique de trouver une solution de cette nature. Et puis s'il faut doubler les crédits pour éviter les expulsions dans, dans ce cas-là franchement comparé à tout ce qu'on gaspille ici ou là, il me semble se ferait bien plus utile à notre République. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement 55 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui ça tient pas adopté. L'amendement 52. Avis défavorable de la commission. Avis favorable du gouvernement qui est pour. Pas adopté.

Alors, article 6 à mon en 89. Monsieur le Ministre du gouvernement. Merci madame la la présidente. L'amendement proposé par le gouvernement. Propose l'indemnisation des des propos l'indemnisation des propriétaires bailleurs est un élément important de l'équilibre entre le droit des propriétaires et des locataires Excusez-moi. Et comme tout le monde un peu fatiguée. La, l'article 6 visent à à modifier l'article L 153 1 du code des procédures civiles d'exécution en disposant que que les modalités d'évaluation de la réparation due aux propriétaires en cas de refus du concours à la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont sans préciser par décret en Conseil d'État, l'article 153 hein et l'article 153. du CP-CE1 pardon pose d'ores et déjà le principe de la réparation en cas de refus de concours de la force publique comme ça été rappelé tout à l'heure par Madame Lienemann dès lors que la loi elle-même prévoit une réparation intégrale du préjudice. Un décret d'application est inutile puisque tous les chefs de préjudice doivent être indemnisés. Tant que les chefs de 10 indemnisables que les modalités de leur évaluation sont déterminés par la jurisprudence administratif et ses principes sont applicables de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisie par le bailleur, dans l'hypothèse où la préfecture fera une proposition d'indemnisation insuffisante. Enfin si la motivation de cet article se font sur le postulat selon lesquels seuls 54% des propriétaires font une demande d'indemnisation en raison de la complexité du dispositif et de la disparité entre les règles appliquées par les procès Un décret en Conseil d'État, précisant les modalités d'évaluation de la réparation due aux propriétaires serait sans incidence sur la méconnaissance par les victimes des droits dont il dispose, l'article 6 est donc à notre avis pas nécessaire et peut donc être supprimés. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas convaincu par l'argumentaire du gouvernement, au contraire je pense qu'un décret permettrait d'harmoniser les pratiques et de rendre plus lisible le cadre normatif qui régit l'indemnisation des propriétaires qui se voient refuser le concours de la force publique tout gain de lisibilité favorable à son appropriation par le public concerné, quel qu'il soit l'avis est donc défavorable. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 99 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour.

À l'article 7 2 amendements identiques, le 19. Madame avez. Merci madame la présidente. L'article 7 s'appliquera en l'état à l'ensemble des procédures d'expulsion sans distinction de la nature et de l'affectation des lieux. Objet de l'expulsion. Ainsi, au vu de l'objectif poursuivi qui est de permettre au CAPEX d'assurer un meilleur suivi des locataires expulsés et que nous partageons. Il nous semble opportun par cet amendement de limiter la communication des informations relatives aux seuls expulsion de locaux habités nous procédons également à une mise en conformité en prévoyant la transmission dématérialisée au préfet et à la CAPEX par le commissaire de police, de justice pardon du procès-verbal qu'ils réalisent lors de l'expulsion d'un lieu habité, je vous remercie. Merci l'amendement 90. Monsieur le Ministre du gouvernement. Est défendu. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Ces deux amendements identiques, nous paraissent superfétatoires puisque l'article 7 prévoit déjà que l'époque CAPEX ne sont compétentes qu'en matière de prévention des expulsions locatives, ce qui exclut les situations de squat qui pourrait concerner des locaux commerciaux, des entrepôts ou des box de Parking. La commission émet néanmoins un avis favorable puisque la transmission dématérialisée des procès-verbaux d'expulsion de lieux habités au préfet et au Cap ex-par les commissaires de justice est une précision utile. donc je mets aux voix l'amendement. Les 2 amendements, 19 et 90, dont celui du gouvernement et avec un avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient.

sur des éléments qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion ce point sécurise le partage d'informations et le respect des personnes accompagnées parce que cela est important. Tendez. Déontologiquement qu'éthiquement le présent amendement précise que ces informations seront communiquées par les professionnels sociaux et médico-sociaux, avec l'accord du locataire cette pratique doit s'inscrire dans une relation de confiance, engagé dans le respect de la personne accompagnée le cadre permet aux professionnels d'être en cohérence avec les principes éthiques de la relation d'aide et d'être transparent avec le locataire en difficulté. Cette précision est d'autant plus importante que les réalités de terrain démontre que les personnes rencontrent des difficultés à aller au devant des institutions et des professionnels qui sont pourtant engagés dans une démarche d'aide, il existe des représentations une peur, une honte pour le locataire d'exprimer ses difficultés qui relève de l'intime. méfiance le partage d'informations doit être le plus lisible possible pour les personnes car il y aura des répercussions directes sur la mise en lien et la relation de confiance on entre les professionnels et le public qu'ils rencontrent. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Bien que nous comprenions largement votre préoccupation chers collègues je ne peux donner un avis favorable à cet amendement pour 2 raisons. En 1er lieu la soumission des membres de l'AKP que ce secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal semble déjà une garantie suffisante. Il est en outre dans l'intérêt des locataires que les CAPEX et les services sociaux disposent des informations nécessaires à l'appréciation de leur situation afin de les orienter vers les bons dispositifs d'accompagnement et ainsi éviter l'expulsion mais en second lieu, cet amendement ne me paraît pas viser le bon dispositif juridique il conviendrait plutôt d'ajouter le conditionnement de l'accord du locataire à la ligne à 14 qui traite de la transmission au CAPEX des données confidentielles par les professionnels de l'action sociale et médico-sociale plutôt qu'à l'alinéa 15 qui traite de la transmission de ces données des CAPEX vers les services sociaux qui élabore les DSF. Avec regret un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Le gouvernement estime que cet amendement. Est déjà satisfait en, en l'état actuel. Du droit la transmission entre l'AKP que et les travailleurs soucieux sont soumis aux aux règles. De et aux normes de de la RGPD garantissant la prise en compte du droit du du locataire, donc en l'état, nous n'émettons un avis défavorable. Merci madame la présidente. je voulais quand même redire quelque chose qui est important pour les travailleurs sociaux qui m'ont suggéré d'ailleurs cette proposition d'amendement, c'est qu'ils sont tenus quand même par le secret professionnel. La relation de confiance à établir entre une famille un ménage et les travailleurs sociaux, c'est toujours compliqué et ça participe quand même. D'une relation qui font maintenir et c'est pas pour alourdir le processus mais croyez-moi, la relation de confiance elle l'essentiel et donc attention quand même à l'avenir à voir si on ne peut pas dans la navette regarder cette question. vous retirez l'amendement. Merci. Alors 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 92. Monsieur le Ministre. Pour le gouvernement. Merci madame la présidente. L'enjeu de de cet amendement déposé par le le gouvernement et de répondre plus rapidement aux besoins du locataire comme du Bayer du bailleur en matière de résolution des impayés locatifs et de prévention de ces expulsions, la dématérialisation des alertes effectuée par les partenaires locaux de la prévention des impayés permettra de simplifier les modalités de saisie administrative des CAPEX et d'accélérer le traitement des informations qu'elles contiennent, par les services déconcentrés de l'État. Parallèlement, l'objectif de cet amendement est de permettre à la CAPEX de saisir les dispositifs adaptés pour traiter le plus rapidement possible les dettes locatives dont elle a connaissance au bénéfice du bailleur et de solliciter en fin de procédure, les dispositifs d'hébergement pour éviter les éventuelles mises à la rue des locataires en situation. Si si je vous remercie. Merci monsieur Capo Canellas pour le 57. Merci madame la présidente. L'intention est la même que celle du gouvernement, je crois que sa rédaction et plus précise. Donc je m'Irakli volontiers. Donc vous retirer votre amendement. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Je voulais donner un avis favorable au 92 une demande de retrait au 57 puisque le 57 et retirer l'avis favorable 92 emporte. Merci donc je m'envoie l'amendement 92 du gouvernement dans l'avis favorable de la. Commission qui et pour qui est contre qui s'abstient et donc adopté. 2 amendements identiques. L'amendement vents monsieur Merci madame la présidente. Notre amendement propose de réécrire de pardon de réécrire l'article L 824 tiré de afin de définir précisément le rôle respectif de la CAF et de la CAPEX en cas d'impayé d'un allocataire et de garantir que la CAPEX soit effectivement décisionnaire en la matière. Merci le 91 identique. Monsieur le Ministre, s'est défendu merci l'avis de la commission, monsieur le rapport. Ces amendements apportent des précisions rédactionnelles pertinente ils évitent toute confusion entre le rôle des CAF et les CAPEX tout en maintenant le pouvoir décisionnaire de ces dernières en matière de versement des APL en cas d'un payé de loyer. J'aimais donc à la vie enfin favorable à ces deux amendements. Merci donc je mets aux voix ces deux amendements identiques, 20 91. Dont celui du gouvernement. Avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient et c'est

35. Monsieur Bénard Roche. Oui oui je vais le défendre, vous inquiétez pas.

Ça me paraît être une sorte de publicité. Peu voilà et délicate, on va dire ça comme ça et. Vous avez vu les positions que nous avons descendu défendu. Vous avez bien compris dans l'opposition sur ce projet de loi je passe et donc nous pensons sincèrement que même modifié par les rapporteurs par la commission des lois par la commission des affaires sociales qui ont emporté quand même des vieux considérable modifié par quelques-uns des amendements qui ont été votées, y compris certains de notre groupe, nous pensons malgré tout que cette loi de correspond pas à une loi qui répondrait au titre qu'il y a été donnée et donc d'une manière. On va dire pour éclaircir les choses. Nous avons proposé de l'appeler par ce que nous. Être les conséquences de cette loi c'est-à-dire condamné les plus précaires à la rue. Donc la proposition de loi devient, proposition de loi condamnant les plus précaires à la rue. je ne vous étonnerai pas si effectivement la vie est défavorable. Nous ne partageons pas le jugement très négatif que portent nos collègues du groupe écologiste sur cette proposition de loi, elle a été vraiment singulièrement améliorée enrichi. Donc j'ai la prétention de dire que là pour le coup, le titre correspond assez au contenu. vous proposons, naturellement, de maintenir le le titre de cette PPL telle qu'il est. Merci Monsieur le Ministre, ma, ma vie. ma vie. Madame la présidente. Merci donc je mets aux voix l'amendement 35, il a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient donc pas adopté, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de de loi. Madame Estrosi Sassone pour explication de vote. Merci beaucoup madame la présidente. remercier encore une fois. Notre rapporteur au fond André Reichardt lui dire que je suis très heureuse d'avoir travaillé de concert avec lui. On a fait un, un fin travail de déminage on a conduit un certain nombre de notions en commun dans un calendrier qui était particulièrement contraint mais je pense que ce qu'on a voulu faire à travers le texte qui est présenté ici au Sénat, a été atteint. Je voudrais également remercier l'ensemble des administrateurs tentent de la commission des lois que de la commission des affaires économiques qui nous ont accompagnés tout au long de nos auditions et pour la, la rédaction de nos amendements. Alors dans ce texte, ce que nous avons voulu faire bien sûr c'est renforcer le Vodé contre le squat et lutter contre l'usage dilatoire des procédures par des locataires qui serait de mauvaise foi mais nous avons voulu également et je crois que ça a été souligné à plusieurs reprises assuré véritablement une distinction entre d'un côté les squatteurs et de l'autre côté, des locataires en difficulté locataire défaillant, ce qui n'était pas du tout le cas lorsque le texte est arrivé de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, je pense que vous en êtes bien conscients et nous avons voulu sur la partie lutte contre le squat effectivement réintégrer un certain nombre de mesures que nous avions fait voter ici au mois de janvier 2021 dans une proposition de loi que j'ai donc j'avais écrit quitter compte pour garantir la propriété immobilière contre le squat. Et donc c'est du temps qui a été perdu. On l'a dit, on l'a dénoncé. Parce que si effectivement cette proposition de loi que nous avions déjà voté il y a 2 ans de cela, avait été présentée. Par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Eh bien aujourd'hui, ces mesures seraient déjà en application. Pour autant, j'espère que, elles le seront maintenant assez donc rapidement, nous avons voulu aussi favoriser le développement du logement intercalaires débloqué surtout la prévention précoce des impayés de loyers. Merci. Tout au long des échanges, il nous a été expliqué qu'il était donc inadmissible. De rentrer chez soi et de trouver quelqu'un qui s'y étaient installés. C'est vrai. Mais et c'est ce que condamne déjà nos lois existence et ce qui a d'ailleurs justifié 170 concours de la force publique délivré en 48 heures durant l'année 2021. Vous l'aurez remarqué aucun de nos amendements ne proposer de revenir sur ces dispositions qui permettent déjà donc l'intervention de la police et des peines de prison. Nous regrettons cependant que le mal ne soit pas traitée à la racine et que les logements vides passe donc. Mais les logements vides ne face par exemple jamais l'objet de réquisitions, contrairement à ce que la loi permet ce que nous regrettons, encore davantage, c'est que ces quelques situations de squat 170 donc serve de prétexte pour légiférer alors que les 300.000 personnes sans domicile sont encore dans l'attente de l'ombre d'une loi les impayés qui conduisent à la suppression d'un bail sont d'abord causer, je l'ai déjà dit par l'absence de politique publique ambitieuse en matière de logement, rien n'est fait pour limiter le prix des loyers dont la part augmente considérablement dans le budget des ménages pris ont pris en étau entre la hausse de prix et la baisse du pouvoir d'achat, 5,8 millions de personnes subissent un effort financier excessif pour se loger. Selon le 28ème. Rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a d'ailleurs été présenté hier. Monsieur le Ministre, mardi soir, vous vous êtes satisfait d'une augmentation du nombre de places des ben on ne d'hébergement de 1% quand le nombre de personnes sans domicile a lui augmenté de 10%. Nous restons donc dans ce même rapport de un à 10 au même titre que l'on compte Guy logements vacants pour une personne sans domicile fixe. Il faudrait donc faire 10 fois plus mais il faudrait pour cela s'attaquer réellement aux inégalités d'accès au logement.

Merci. Monsieur le rapporteur. La commission des Lois pardon en la personne du président François Noël Buffet et les des collègues et puis de façon globale. Toutes celles et ceux qui ont bien voulu contribuer à améliorer ce texte, on va le dire comme ça à améliorer ce texte qui méritait quelques. À tout le moins modifications améliorations que je n'sais pas d'ailleurs à appeler amélioration. Je voudrais aussi. Remercier pour la qualité des échanges et puis. Mais c'est d'usage ici la civilité des interventions des uns et des autres. Ah en disant aussi, Monsieur le Ministre que. Félicitant que il va pouvoir il va pouvoir il y avoir une deuxième lecture. Sur ce texte et ce à n'en pas douter à travers cette 2ème lecture nous pourrons encore peut être amélioré l'un ou l'autre point sur lequel nous étions un peu quoi. Dans ce court laps de temps qui les là qui nous a été attribué pour faire ce travail, je vous remercie. Avant de donner la parole. Je vous signale que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains pour vous puissiez aussi vous vous préparez. Monsieur Salmon. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme vous tous les matins et tous les soirs je je croise de nombreuses personnes à la rue. Ces personnes-là, à un moment sans doute, elles ont eu hein ah logement. Et les vicissitudes de la vie les ont amenés là où elles sont aujourd'hui. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce que cette loi va aller dans le sens. De d'avoir moins de personnes à la rue. Je n'en suis pas certain, je pense même clairement que c'est le contraire parce que le but est bien là, d'accélérer les expulsions. On parle d'équilibre. Effectivement, j'ai bien vu que dans, au niveau de la commission on a essayé de rendre cette loi un peu moins implacable et un peu moins déséquilibré en faveur des des bailleurs et que l'on n'a pas considéré de la même manière les squatteurs et les locataires qui avaient des soucis pour payer leur loyer. Effectivement j'entends bien qu'il a eu quelques avancées mais. Au fond, cette loi va quand même dans le sens. 2 rigidifier ce qui était possible avec des juges. On a déjà tout un arsenal qui était là. Il faut faire en sorte que lorsqu'il y a une décision de justice elle soit appliquée. Il faut que le préfet a jusqu'au bout qu'il ait, dès qu'il puisse reloger également, on est dans un moment où ça fonctionne, on peut le dire, très mal et je pense que cette loi va aller dans une aggravation de la situation donc c'est pour ça qu'avec notre groupe, nous voterons contre bien entendu cette loi. Merci ma progression. Merci madame la présidente. Je voudrais féliciter la Commission les rapporteurs pour le travail qu'ils ont effectué de cette distinction qui a été fait clairement entre les squatters et entre les locataires vous le savez, moins ça fait 16 ans je suis le dossier des squatters et j'ai redit au Ministre comme je l'ai dit à tous les ministres, ils l'ont précédé sur ces bancs, depuis 16 ans. Il y a déjà une loi il y a ce fameux article 38 élaborée. Effectivement en pleine nuit. Mais si la justice et les préfets avaient appliqué la loi depuis ses 16 ans, ne serait peut-être pas contraint à devoir remodifier et à chaque fois repréciser des choses donc plusieurs des ministres ont dit oui on va vérifier et on va faire en sorte que ce soit appliqué. Je vous assure que pour depuis 16 ans, suivre en tout cas à l'application de l'article 38 de la loi Dalo. Le nombre de le nombre de préfets qui y aurait un certain nombre de dispositions, j'en ai eu eu et j'en ai vu beaucoup donc pour que la loi soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée et je reçois je rejoins en cela monsieur Gondard, s'il a été appliqué, on n'aurait peut-être pas besoin de légiférer de nouveau. Merci. Même la présidente Valérie d'État. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. À mon tour de féliciter évidemment nos deux rapporteurs. Qui ont vu arriver ici sur le bureau du Sénat et dans les commissions. Un texte. Que nous n'aurions peut-être pas en tout cas pour notre groupe Union centriste voter en l'état et certainement pas pour ma part. Car effectivement la façon dont été traité d'une part les squatteurs et d'autre part les locataires défaillants. N'était absolument pas acceptable et et absolument pas envisageable ce rééquilibrage que vous avez permis madame et monsieur les rapporteurs était absolument indispensable et d'ailleurs nous vaudra de voter favorablement ce texte nourri et enrichi par le travail par aussi effectivement Madame Estrosi. Sassone. La proposition de loi, vous l'avez rappelé que vous aviez initié il y a bien longtemps maintenant nous aurait permis peut-être d'avancer plus rapidement mais en tout cas, on le voit un gros travail a été menée pour apporter des outils dans la gestion des impayés sur la prévention des impayés de loyers. Parce que c'est vrai que la première des solutions à trouver. C'est déjà celle de ne pas laisser ces familles en difficulté et s'embarquer dans cet engrenage, réduire les délais, être plus efficace en amont. Favoriser les échanges entre tous les acteurs de la gestion des impayés de loyers, c'est absolument essentiel, le travail aussi et les initiatives par un moment qui ont été posées sur tous les bancs et par tous les groupes ont permis d'enrichir et du gouvernement aussi, Monsieur le Ministre. D'enrichir aussi le travail des rapporteurs et je pense qu'on peut. Alors chacun avec sa sensibilité chacun avec peut-être un vote différent mais reconnaître que le Sénat a fait plus qu'oeuvre utile et qu'aujourd'hui sort en texte de cette assemblée Un outil qui va permettre à mon sens d'améliorer la gestion, la situation des propriétaires d'une part des locataires. D'autre part et évidemment aussi de faire une distinction telle qu'elle doit l'être entre squatteurs d'un côté locataires en fragilité de l'autre il me semble que, aujourd'hui, le Sénat a joué son rôle.

Une fois que vous aurez sorti un squat. Par une décision là je parle pas du squat occupé à pas de domicile hein on est tous d'accord que ça c'est le sujet à traiter. Hé ben 15 jours après. Il reviendra. Et rebelote. Ce sera pas les mêmes rebelote parce que si on s'attaque pas à traiter ces sujets autrement. Ce ne sera pas réglée. Et puis ce que le, le ministre de la justice ou Denis grande leçon hier. Je voudrais bien qu'il fasse une circulaire aux procureurs. classer ils arrêtent de classer sans suite quasiment tous les litiges. Qui a qui mettent en cause des propriétaires qui ne sont pas corrects. Le nombre de fois où le logement décent classée sans suite. Protestations sur telle ou telle des gens qui font des vous savez des travaux dans la cage escalier pour virer les gens pour rendre invivable logements classée sans suite. Et même je l'ai dit d'ailleurs quand tu des squatter dans des logements HLM. Je connais des organismes HLM qui ont déposé plainte auprès du procureur parce que justement les réseaux qu'on veut combattre s'était installés les réseaux de de squat unique et ben classée sans suite. Alors on se fait. Des énormes d'écran de l'éclat ration et ben qu'il nous fasse une circulaire qui rectifie le fait que le droit au logement, c'est fondamental et qu'on arrête de classer sans suite, parce que ça sert à rien de faire des lois et on constatera après que n'étant pas appliquée, on va encore les durcir. Je regrette ces attitudes. Merci. Alors donc quand je vous l'ai dit, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin clos. Alors résultat du scrutin. 343 votants exprimés, 343 pour 252 contre 91, le Sénat a adopté.

l'ensemble des des sénatrices et sénateurs présents sur l'ensemble de Vauban. Je je crois que le le le travail qui, qui a été fait est un travail de, de qualité, il a concouru à améliorer comme ça a été dit. Le texte. Ah le rendent en encore plus équilibrée, en tout cas. J'en suis intimement convaincu et et donc encore une fois, merci à tous et le travail pourra continuer comme ça a été dit en en en deuxième lecture pour encore améliorer enrichir ce ce texte merci. Merci. Alors, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mardi 7 février à 14h 30 pour l'examen de la proposition de résolution exprimant le soutien du Sénat à l'Ukraine, condamnant la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie et appelant au renforcement de l'aide fournie à l'Ukraine. La séance est levée.